La séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du mercredi 25 janvier. A été publié sur le site internet du Sénat. Y a-t-il des observations. Le procès verbal est donc adopté. Madame la Ministre, mes chers collègues. Avant d'aborder notre ordre du jour. Je souhaite. Salué la mémoire d'un grand résistant. Qui fut aussi un fonctionnaire exemplaire de notre institution. Jacques Bloch. Directeur honoraire du service des commissions du Sénat. Nous a quittés le 28 janvier dernier. Né dans une famille qui avait quitté l'Alsace Lorraine. Pour rester française. Il était entré. Dans la résistance à l'âge de 20 ans. Joue un rôle de 1er plan. Dans la libération notamment. De la ville de Guéret. Grièvement blessé, il fut capturé. Livré à la Gestapo. Torturé. Avant d'être déporté à Buchenwald. Parvenant à s'échapper, il puis rejoint les forces armées américaines. Et revenir. Intégrés au Conseil de la République. Dès 1946. Il a servi l'administration sénatoriale pendant plus de 40 ans. Jusqu'en 1990. Recueillant les éloges unanimes de nos prédécesseurs et de ses collègues. Pour son dévouement et la qualité de son travail. Pour ces actes. D'héroïsme. Jacques Bloch fut nommé commandeur de l'or de la Légion d'honneur par décret du général De Gaulle. Même si vous ne l'avez pas connu. La cérémonie aux plaques. Du 11 novembre. Jusqu'en 2020. Il fut toujours présent. Petite silhouette. Celui de ces tortures un bras pour partie au moins. Il était toujours fidèle à cette cérémonie et à cet engagement. Alors je voulais. Au nom du Sénat d'aujourd'hui au nom du Sénat tout entier. Rendu hommage à la mémoire d'un homme. Qui incarnera à tout jamais le courage. Et l'abnégation au service de la France. Et de valeurs que nous portons ensemble dans notre diversité.

chers collègues. Oh non au au regard du nombre d'amendements déposés sur les textes inscrit à l'ordre du jour de cet après-midi. Et en accord avec le gouvernement et les commissions concernées. Nous pourrions, d'une part reporté à demain soir, mercredi 1er février l'examen de la provision de loi visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des 25 années d'assurance des plus avantageuses. Examen, initialement prévu en dernier point de notre ordre du jour. De la journée. D'autre part. D'ouvrir la nuit de ce soir et prévoir une éventuelle. Suite de l'examen de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite le jeudi 2 février après-midi. À l'issue de l'espace réservé au groupe écologiste solidarité et territoires et éventuellement le soir. Y a-t-il des observations sur l'organisation de ce débat pour nous permettent d'examiner ces différentes propositions dans les meilleures conditions possibles. Je n'en vois point il en est les. L'ordre L'ordre du jour appelle les explications de vote, des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Je rappelle que la procédure accélérée a été engagée sur ce texte et je donne immédiatement. La parole et pour 7 minutes. À Dali Wattebled pour le groupe les indépendants République et Territoires. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le président, madame Nice, mes chers collègues. Le 26 juillet 2024. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques marquera le début d'une grande fête populaire. Célébré dans tous les territoires ruraux comme urbains. Tous les Français seront au rendez-vous. Elles ne seront pas les seuls. athlètes. Athlète paralympique et 10.500 athlètes olympiques s'affronteront dont 4 milliards de téléspectateurs. Au-delà de son ampleur et de attendent qu'il génère. Cet événement est inédit à plus d'un titre. il mort inédit par l'immense défi que représente la Serbie d'ouverture en plein air. Il a ensuite inédit. Par son exemplarité écologique. Puisque nous accueillerons les premiers jeux alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris. Cet événement est enfin inédit. Par son exemplarité en matière de parité et d'inclusion. Déjà. En 1924 les Jeux de Paris marqué l'histoire en ouvrant pour la première fois les portes. Aux athlètes féminines. 100 ans plus tard, la France se démarque encore en leur dans les premiers jeux strictement paritaires. Je souhaite également faire un clin d'oeil aux prises nos 2 mascotte. Par partisan jument technique nous rendons notre droit conforme pardon. Pour la première fois les mascottes olympiques et pro-olympiques sont identiques. Avec une prothèse visible pour la seconde. Malgré les apparences, cela n'a rien à Loudun. Nous on pouvait de joie et d'émotion à accueillir, pour la première fois, aussi en France. Ces jeux et admirer la tête concourir au Grand Palais pour l'escrime fauteuil au château de Versailles pour les épreuves de para-équitation ou encore au Champ de Mars pour le rugby fauteuil. En aimant des jeux ce texte propose de nouvelles dispositions en matière de lutte contre le dopage. De sécurité, d'adaptation à l'Outre-mer ainsi que des mesures sanitaires. Par ces ajustements techniques, nous rendons notre droit conforme aux exigences du comité international olympique. Les apports du Sénat vont dans le bon sens et permettent d'apporter quelques précisions nécessaires, nous pouvons nous en féliciter. Dans le cas de la lutte contre le dopage. Le Sénat à favoriser la collaboration avec l'Agence française de lutte contre le dopage et de la cellule de renseignement financier national. Nous avons aussi pérenniser la Poste et de procéder à des tests génétiques et c'est une bonne chose, car le vent adapter nos méthodes de détection aux pratiques dopantes qui rivalisent d'innovations. disant identifieront pleinement et plus facilement ce qui serait brisé le serment olympique. Le Sénat a voté plusieurs mesures de simplification. Parmi elles, nous avons facilité l'accès aux autorisations de stationnement spécifiques. Pour les taxis aux abords des jeux, des endroits des Jeux olympiques. Il est essentiel également d'être partisan exigeant sur la question d'accepter aux équipements et aux épreuves. Le Sénat a également simplifier cette procédure permettant de déroger au repos dominical. Cette adaptation temporaire au droit du travail permettra aux commerces concernés de bénéficier pleinement de l'afflux de des visiteurs. Durant les prochains mois. La France va accueillir du plusieurs événements de grande ampleur. Ces jeux bien sûr olympique et par. Sont parmi les plus regardées. Pour l'image d'autres pays. Mais aux aussi et surtout pour le concitoyen et pour les visiteurs. Nous devons assurer qui se déroulent en toute sécurité. Nos forces de l'ordre sont pleinement mobilisés dans la préparation de ces jeunes. Elles auront besoin de renfort. La sécurité privée constituera à cet égard un atout précieux. En plus d'effectifs suffisants et nous semble nécessaire que ceux qui nous protègent puisse employer les meilleurs outils. le traitement algorithmique et la de la vidéoprotection. A suscité beaucoup de débats. Nous pensons qu'elle constitue une avancée majeure pour la détection des troubles à l'ordre public. Que ce soit des mouvements de foule ou des menaces terroristes. Comme toute technologie, il y en a néanmoins nécessaire d'encadrer strictement son utilisation pour protéger au mieux la liberté a du duel de nos concitoyens. Nous nous félicitons que la CNIL soit étroitement associé à son développement. monsieur Hermier. Par ailleurs, le texte renforce également les sanctions concernant les intrusions dans les stades. Nous saluons ces mesures, il faut cesser d'instrumentaliser le sport à des fins politiques. C'est un espace de rassemblement où il faut mettre en avant ce qui nous rapproche. Plutôt que ce qui nous divise. Pour ces différentes raisons. La modification au Sénat de l'intitulé du texte désormais plus ouvert permet de rendre compte de la diversité des dispositions prévues pour permettre aux Jeux de se dérouler dans de très bonnes conditions. Enfin. Si les joueurs en eux-mêmes représente un événement majeur. Que nous sommes fiers d'accueillir. Il est essentiel de préparer la suite. La politique d'héritage et sa durabilité dans le temps sont essentiels. En effet. Quelle meilleure occasion que ces jeux pour faire de la France une nation sportive. Il a-t-il rappelé. Madame le Ministre. Que l'acte physique et sportive a été érigée en grande cause nationale en 2024. J'en suis heureux. Pour nos jeunes. Pour qui l'augmentation du temps dédié au sport dans les écoles primaires et les collèges mais aussi. Pour la commission du passeport sont d'excellentes nouvelles également heureux pour le moins jeunes si j'ose dire car nous connaissons les vertus de la pratique sportive pour la santé. En 2024, la France avec Jérôme des 38 médailles dont 13 en or en 2024. Nous sommes certains. En 2024, certains que nos athlètes olympiques et paralympiques représenteront fièrement nos couleurs cette confiance que nous pouvons leur adresser nos encouragements pour le dernier mois de préparation. Les Jeux olympiques ne sont pas seulement des compétitions sportives. Ce sont aussi des temps, des temps de fraternité, d'échange et de découverte des temps d'émerveillement aussi. Nous devons relever ce défi ensemble. Aussi les groupes d'importants votera ce texte et appelle à la position de tous pour célébrer ensemble le sport ses valeurs et ses adeptes dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Et maintenant notre collègue Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre madame. Et monsieur le rapporteur, chers collègues. Les semaines et les mois passent et envolée sécuritaire de ce gouvernement ne retombe jamais. L'examen en séance de ce projet de loi a démontré par bien des aspects les réels motifs d'un véhicule législatif dans le but n'est pas tant l'adaptation de certaines de nos règles pour un déroulement seraient des épreuves des Jeux olympiques mais bien essentiellement la mise en oeuvre de nouveaux outils sécuritaires poursuivant la dérive de ce gouvernement. Vers une société de surveillance. Nous l'avons déjà exposé mon collègue Thomas Dossus a défendu avec cohérence et sincérité. Quel est le coeur de ce projet de loi. Une mise en concordance du droit de la santé pour des questions de dopage. Une réécriture du code de l'urbanisme pour le développement futur du sport dans nos territoires dès les Jeux. Non, il n'en est rien. Nous aurions pu être à vos côtés madame la 10 pour soutenir les fédérations et le sport amateur comme professionnel, qui voit dans les JO. La vitrine qui sort accélérer la pratique sportive dans toute sa diversité. Nous aurions aussi hé bé débattent sérieusement de la Pac de cet événement sur d'autres tissus de festivals et d'événements culturels sur les surcoûts et les difficultés pour les organisateurs ou les collectivités sur l'utilisation culturelles, sportives. De l'Exposition offerte à d'autres nations par cette vitrine ouverte sur le monde nous aurons une France sous cloche comme le craint ma collègue Monique de Marco La vie les autres activités continuera pendant ces Jeux et la sécurisation de ces autres événements outre surcoût pour leurs organisateurs souffrira de risque de précipitation et de formation insuffisante. Nous avons eu l'occasion de le dire quel étrange texte centrée sur les JO et sur les Jeux paralympiques, qui compte plus de 80% de mesures pérennes. Car à des aspects les plus remarquables des articles les amendements étudier et voter quand six dans la mise en oeuvre sur un temps long de mesures censées d'être nécessaire que pour le bon déroulement des Jeux. Cette loi est bien plus loin que l'organisation des Jeux. Qu'en est-il de ce cheval de Troie sécuritaire. Notre groupe regrette une nouvelle fois une vision débridée et si éloignée des valeurs de l'olympisme. La disproportion des mesures pour la sécurité en jeu dans ce texte cache de réels atteinte aux droits des personnes qui s'inscrivent bien au-delà du temps des jeu j'ai pu l'exprimer tout ce déploiement de la vision sécuritaire n'recours massif et presque à différencier à la vidéosurveillance ont augmenté. Proche de nombreuses questions. Durée de l'expérimentation. Finalité de l'expérimentation à venir des apprentissages de ces machines contrôle de mécanismes algorithmique dangereux potentiel mise à disposition pour d'autres opérateurs non nationaux plus ou moins respectueux des droits de leurs citoyens. La CNIL dit dans son positionnement plus que prudent sur ces technologies qu'sont susceptibles d'affecter les garanties fondamentales apporter aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. C'est bien une vision sécuritaire technologique qui se dévoile et que deux jugeant d'autant plus des fast-et inefficace. Aubert complètement le terrain. Car sur le terrain. Que se passe-t-il. Le recrutement, la formation des agents de sécurité n'a pas été anticipé. Nous allons manquer de personnel, publics et privés. Le recours à l'armée Madame la Ministre ne va pas tarder à être annoncés. La Cour des comptes estime qu'il faudrait employer 22.000 à 33.000 agents de sécurité privés par jour pour véritablement sécuriser l'ensemble des épreuves. Ces chiffres-là dépasse largement les capacités disponibles dans des entreprises de la région et du pays. Les craintes de voir sur le terrain des gens peu formés face à des événements d'une telle ampleur laisse inévitablement ressurgir le spectre du fiasco du Stade de France. Il est vrai qu'il est difficile de retenir les leçons d'un événement que le gouvernement a toujours considéré comme bien bien préparé ce déni. Coupable ne doit pas être l'occasion de manquer de remettre en cause et de faire progresser les tactiques de matière, de l'ordre et de la gestion des flux de population. Au-delà. Des craintes de la mise en place de mesures Sécurité disproportionnées rien dans ce texte vient éloigner le doute d'une explosion des coûts comparables à l'expérience londonienne. Ce texte ne s'attarde pas et ne s'inquiète pas de l'étude du triste héritage financier et budgétaire que pourrait laisser les Jeux olympiques et paralympiques. Le dernier rapport de la Cour des comptes alerte pourtant clairement sur un budget qui n'est toujours pas connue. Qui des précisément pas établi, mais on nous a dit que ça allait là. Bientôt, et rien ne rassure vraiment les collectivités autre d'événements sur les garanties financières que devrait leur apporter l'état. Il est également regrettable que les collectivités qui se sont engagés pleinement dans le projet olympique soit mise de côté pour des décisions pratiques comme nous l'avions demandé par exemple au travers de l'exercice temporaire de pouvoir de police de circulation et de stationnement. Décision qui permettrait de limiter la pacte environnemental des Jeux. L'impact environnemental. Annoncé comme cheval de bataille de ce gouvernement. Mais que n'a-t-il pas été à danser sur ce terrain par Emmanuel Macron et ses gouvernements depuis bientôt 6 ans, sans être suivi de mesures à la hauteur des enjeux vitaux. Impact aussi sur la qualité de vie des riverains des jeux qui en plus de ne pas être sûr de pouvoir participer et assister à cette fête devra subir l'invasion de la publicité dans un cadre anormalement dérogatoire aux règles du droit commun en vigueur. Les entreprises partenaires sont ainsi autorisés à afficher sur les bout du historique les espaces naturels et à peu près tous les éléments qui leur conviennent dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site d'organisation des Jeux olympiques. Partenaires. Dans certains pour en faire feu sans retenue, alors qu'ils sont notoirement répertoriés pour leur action néfaste à l'environnement et au changement climatique. Est-ce vraiment des jeux pour l'environnement. Part essentielle du d'incitation à consumérisme débridé ses affichages ont des conséquences environnementales que nous n'acceptons pas en temps normal. Alors que nous avons en fait réussi à limiter la pollution visuelle des panneaux lubies de ces dérogations prise au bout. Où l'État incite à la sobriété énergétique n'ont pas de sauce. À croire que nous pouvons mettre tout cela entre parenthèses, le temps des Jeux quelle hérésie. Nous avons tenté au travers de plusieurs amendements de recentrer la loi sur ce qu'elle devrait être. L'encadrement des JO et non sur ce qu'une dérive sécuritaire pérenne au détriment du droit des citoyens. Certaines positions, a été entendu par la commission et par le gouvernement. Très peu, trop peu. La plupart ne leur pas et l'équilibre du texte n'a pas été modifiée, nous maintenant une analyse de texte trop dangereux pour les libertés individuelles aux objectifs réels qui aurait nécessité une concertation une confrontation sereine 2 visions différentes sur la sécurité globale de notre société en fait sur d'autre modèle de société. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre ce projet de loi. monsieur le Président Madame la Ministre Mesdames messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le compte à rebours est lancé dans 542 jours 4h et 9 minutes. Une fête unique débutera dans notre pays, celle des Jeux de 2024. Une aventure sportive incomparable qui fera la fierté des Françaises et des Français et plus encore s'il arrive à la hauteur de nos ambitions, à savoir une fête sportive populaire dont l'héritage deviendrait le symbole d'un nouveau modèle de jeu sobre durable et inclusif, les jeux n'étant pas un événement sportif comme les autres. De nombreuses questions se posent, se pose. Quant à son organisation. Raison pour laquelle nous devrons prendre toutes les précautions pour assurer son bon déroulement, c'est je crois l'esprit de ce projet de loi, un texte qui répond à de multiples enjeux et qui ne mérite par conséquent. Pas l'appellation de texte sécuritaire. Une fois encore, les arguments soulevés par le groupe écologiste sont tout à fait contestable exprimé des inquiétudes ou des désaccords. Quant à la vidéoprotection et à ses usages, c'est une chose mais qualifié ce texte de copies techno sécuritaire, c'est autre chose. Résumé ce projet de loi, un texte qui ne traiterait que de la sécurité et faux et d'une certaine manière c'est même injuste. Alors certes, il est question de sécurité dans ce projet de loi. Le texte vient renforcer nos dispositifs de sécurité avec l'expérimentation d'un dispositif de vidéo-protection ayant recours à l'Intelligence artificielle non la ligne rouge de la reconnaissance faciale n'a pas été franchie exigences du recours au contrôle humain, système de gestion des risques, accompagnement et contrôle de la CNIL dans le développement et l'application des traitements, autant de garanties supplémentaires adoptée par notre assemblée qui permettront. D'éviter les dérives liberticides que vous craignez tout autant que nous. Oui, le projet de loi permet de mettre en place des scanners corporels à l'entrée des enceintes qui accueilleront plus de 300 spectateurs à l'image de ce qui existe déjà dans les aéroports parce que c'est une mesure intrusif, là encore, nous apportons des garanties supplémentaires à l'image de l'amendement porté par mon collègue Dominique Théophile exigeant de recueillir obligatoirement le consentement Express des personnes contrôlées par ces scanners. Un amendement adopté qui apporte une garantie non négligeable. Une garantie parmi d'autres, tels que l'impossibilité matérielle de reconnaître un visage ou encore l'interdiction du stockage et de l'enregistrement des images. Oui, le projet de la renforce notre arsenal juridique pour assurer la sécurité de tous et la tranquillité des épreuves olympiques et paralympiques. Nous devons tirer les enseignements des incidents passés afin d'éviter qu'ils ne se reproduise. Raison pour laquelle. L'obligation de présenter un titre d'accès pour rentrer dans une enceinte sportive et l'obligation pour les organisateurs des manifestations les plus importantes de recourir à des billets nominatifs dématérialisée et infalsifiable, sont à mes yeux des mesures justifiées et proportionnées, par conséquent, non, nous ne sommes pas dans la surenchère sécuritaire. Il s'agit d'apporter des précisions juridiques utiles aux juges qui appliqueront et respecteront les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines. ce projet de loi met en oeuvre des moyens nécessaires afin d'assurer la sécurité des Jeux des participants et du public. Rappelons également que ce texte traduit certaines des recommandations figurant dans le rapport d'information du Sénat sur les incidents survenus au Stade de France en mai dernier. Mais comme l'ont démontré nos débats, mes chers collègues, ce texte répond aussi à des enjeux liés à la santé, au sport et à l'organisation des Jeux. Sur le plan sanitaire d'abord en proposant une une adaptation de l'offre de soins et de premiers secours. Je pense à la création de la polyclinique olympiques et paralympiques 100 centres de santé unique au coeur du village. Je pense également aux professionnels de santé étrangers qui pourront bénéficier d'une autorisation d'exercice dans le cadre des jeux ou encore la possibilité pour d'autres acteurs que les axes, les associations agréées de la sécurité civile de délivrer des formations aux premiers secours. Ce texte protège également les valeurs de l'olympisme à travers la lutte contre le dopage en autorisant le recours aux tests génétiques des tests réalisés par le laboratoire antidopage français de l'université de Paris-Saclay qui seront utilisées par l'International Testing Agency à qui. Le CIO a confié la mission de contrôle contrôle antidopage. Mes chers collègues. Le projet de loi apporte aussi des réponses aux enjeux liés à l'organisation des Jeux, pensons à la mise en oeuvre de la dérogation au repos dominical qui sera, je le rappelle conditionné au respect du volontariat des salariés, ainsi qu'à l'octroi des contreparties légal prévue dans le code du travail. Les communes situées à proximité des sites de compétition ont été intégrés à juste titre pour éviter tout risque de rupture d'égalité entre les entreprises, notamment les communes qui sans être limitrophes aurait pu avoir une affluence de touristes. Je pense également à la mutualisation des moyens de la Solideo avec ceux de Grand Paris Aménagement je pense enfin à l'attribution de nouvelles autorisations de stationnement pour les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant alors oui mes chers collègues. Il est bien il est. Bel et bien question de sécurité dans ce projet de loi mais n'oublions pas de préciser qu'il est aussi question de sport de santé et d'organisation. En témoignent les modifications bienvenues qui ont été adoptée par notre assemblée en commission séance parmi les apports du Sénat, soulignant la clarification du statut des règles dérogatoires de la polyclinique ainsi que la possibilité pour les volontaires olympiques et paralympiques de participer aux missions du Centre de santé je pense également à l'autorisation des échanges d'informations entre l'Agence française de lutte contre le dopage et Tracfin, la cellule de renseignement financier dans France-française. Je pense au droit pour les personnels affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les Jeux de retrouver leur affectation antérieurs. Une fois l'événement achever notre assemblée a également voté des mesures significatives en matière de lutte contre le dopage. À l'image de la pérennisation des tests génétiques aux fins de lutte contre le dopage permettant de mettre en conformité. Notre code du sport avec le code mondial antidopage. Une lutte qui sera renforcé en Polynésie française grâce à l'extension de certaines mesures d'enquête. Saluons enfin la proposition du rapport de la Cour des comptes sur l'organisation, le coût et l'héritage des Jeux qui permettra de mettre en lumière le travail colossal qui est menée en la matière et de suivre son évolution. En définitive, mes chers collègues, nos débats ont je crois, permis de préserver l'équilibre de ce texte tout en l'enrichissant sur de nombreux aspects, loin de toute polémique. Le groupe RDPI votera donc pour ce projet de loi qui nous rassemblera sans doute sur un point l'impatience d'assister à ces Jeux olympiques et paralympiques qui s'annonce d'ores et déjà historique. Si mon cher collègue. La parole est à d'autres collègues Jérôme Durain pour le groupe socialiste. Écologiste. Vous avez Vous avez la parole. Le Sénat s'était prononcé à l'unanimité en faveur de l'adoption de ce 1er texte cette unanimité témoignait de la volonté, quelles que soient les bancs de réussir, Paris 2024. 5 années plus tard et un an et demi avant les Jeux de Paris. Voici le Parlement à nouveau saisi d'un projet de loi. S'il était initialement affublé du même titre, le Sénat a accepté nos demandes on ajoutant à son intitulé la précision suivante portant diverses autres dispositions. Ce n'est pas anodin. Nous souhaitons toujours comme l'ensemble des sénateurs et sénatrices de cet hémicycle, la réussite des Jeux. Cette réussite passe-t-elle par l'adoption de ce texte. Alors il y a bon nombre de mesures très utile. Présente dans les 24 articles de ce projet de loi ainsi les adaptations nécessaires en matière d'offre de soins, de formation aux premiers secours sont compréhensibles, on perçoit bien la nécessité d'avoir un centre de santé au sein du village olympique, tout comme la possibilité de former davantage de monde aux premiers secours. Le chapitre consacré à la lutte contre le dopage est d'importance. L'autorisation de l'examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison des empreintes génétiques pour les analyses antidopage a provoqué de vifs débats dans l'hémicycle. Nous nous félicitons de l'adoption de l'amendement de notre collègue Lozach, qui prévoit un échange d'informations entre l'Agence française de lutte contre le dopage et Tracfin. Le chapitre 5 évite le recours aux ordonnances pour l'application en outre-mer cela devient une habitude légistiques sénatoriale et c'est un progrès indéniable. L'un des enjeux principaux mis en avant par le gouvernement concerne la sécurité de ces Jeux olympiques. Alors que notre pays reste confronté à des menaces d'envergure. Nous comprenons que l'exécutif consacrent beaucoup de ressources à cette problématique. Nous comprenons la recherche d'efficacité, en donnant plus de pouvoirs aux préfets nous comprenons la mise en conformité du régime de la vidéoprotection avec le droit européen sur la protection de données. Nous sommes donc prêts à comprendre beaucoup de choses mais cela ne veut pas dire que nous soyons prêts à tout accepter. Ce qui nous intéresse dans ce texte, ce sont les Jeux olympiques et les Jeux para-olympiques pourtant plusieurs mesures qui sont présentés comme étant des expérimentations temporaires sont amenés à être pérennisés au-delà de la seule échéance des Jeux cela et le fait de la volonté du gouvernement, mais c'est aussi le résultat de plusieurs évolutions porté par la majorité sénatoriale. Le Sénat a retiré tout caractère expérimental à la possibilité pour le laboratoire antidopage français de procéder à des tests génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs. Pourtant, la mise en oeuvre de ces mesures qui déroge aux dispositions du code civil issu des lois bioéthiques aurait mérité un débat approfondi et une expertise pluraliste que l'unique rapport d'évaluation envisagé par la majorité sénatoriale ne peut suffire à combler sur la vidéo surveillance automatisée. La position de la majorité sénatoriale aboutit à préjuger de la pérennisation de cette technique de contrôle qui constitue un véritable tournant en matière de sécurité publique. En votant la durée de l'expérimentation, bien au-delà de la période des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En annonçant d'ores et déjà sa reconduction, voire son application définitive ce texte olympique défini dans notre pays un nouveau standard de sécurité même rendu plus précis par les travaux de notre chambre même en prévoyant un droit d'information du public renforcé. Nous considérons qu'il ne s'agit pas du bon véhicule législatif pour porter des choix aussi lourd. Par ailleurs, l'organisation des Jeux olympiques de 2024 constitue un prétexte pour apporter une solution sécuritaire à des problèmes de maintien de l'ordre au sein des stades et renforcer démesurément les peines applicables. Alors même qu'un groupe de concertation entre représentants des supporters et des ministères concernés est à l'oeuvre des associations de supporters dont on peut considérer qu'ils sont des amis du monde sportif ont ainsi exprimé leurs plus vives inquiétudes quant au contenu de cette loi les articles 12 et 12 bis sous l'initiative de la droite sénatoriale sont d'autant plus malvenue que l'exécutif souhaite restaurer le dialogue avec les supporters, ces dernières années. Faut-il donc envisager des peines de prison si des militants envahissent le Stade de France pour porter un message politique. Au groupe socialiste. Nous sommes conscients que parfois la politique s'invite dans le sport. À l'inverse du président Macron et nous ne pouvons pas accepter des dispositifs proposés qui nous paraissent inutilement durcie. Quant au chapitre IV consacré aux dispositions diverses reconnaissons qui a abouti à des discussions parfois Cavaliere pourtant plusieurs de nos amendements qui avait un lien Direct avec la réussite des Jeux olympiques ont eux aussi été jugée irrecevables les transports en commun parisiens, la taxe de séjour dans les hôtels de luxe des villes hôtes le travail le dimanche dans les communes concernées par les Jeux l'affectation renforts humains pour insécurité là Autant de sujets dont nous n'avons pas pu débattre alors qu'ils auraient enrichi utilement nos débats. Le groupe socialiste, écologiste et républicain est entré dans la discussion parlementaire de manière constructive souhaitant je le répète, la réussite des Jeux, nous le souhaitons toujours mais le texte déposé par le gouvernement comme la discussion en commission, puis dans l'hémicycle, non pas levé tous nos doutes des inquiétudes légitimes, notamment autour de l'article, sept ont beaucoup crispés et nos doutes demeurent. Le bilan est donc mitigé face à l'accumulation d'expérimentation que nous considérons mal encadrés et pas assez restreinte. Nous faisons le choix de l'abstention exigeante à ce stade de l'examen du texte. La réussite de Paris 2024 ne justifie pas que l'on accepte des reculs présents ici ou là, dans cette loi. Nous suivrons avec vigilance la navette parlementaire, espérant notamment être rassurés sur les moyens mis à disposition de ces jeux sur la préservation de l'agenda culturel 2024 et espérant surtout que les expérimentations. Dans ce texte seront davantage encadrées. La parole est à madame la présidente. Éliane Assassi. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. madame la présidente. Face à des enjeux réels de sécurité mais aussi de rayonnement international, vous avez subrepticement introduit un florilège de dispositions attentatoires aux libertés et droits fondamentaux. Le problème est bien que ces dispositions sont voués à être pérennisés. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Pourtant, le gouvernement a décidé d'être sourd. Mon groupe rappelle que l'exception doit demeurer temporaire et nous regrettons qu'avec ce projet de loi l'exception soit banalisé et rentrera finalement dans le droit commun. Nous refusons d'adhérer à la vision que vous nous proposez des JO et des J. O. P sous prétexte de sécuriser l'événement, ce texte ouvre la boîte de Pandore ou à des atteintes aux droits les plus fondamentaux. Avec les nouvelles technologies que vous nous proposez. L'heure est au détricotage du RGPD. Nous passons un cap, nous sommes face à un laboratoire juridique et sécuritaire que nous rejetons fermement jusqu'où pouvons-nous aller dans l'atteinte aux libertés individuelles sans mettre le moteur des expérimentations que vous nous proposez. Les droits fondamentaux sont niées par la vidéosurveillance algorithmique et nos fortes réserves n'ont pas été prises en considération. Cela est bien regrettable. La France étant jusqu'ici en pointe dans le domaine du RGPD. Les droits fondamentaux ne doivent pas s'effacer au profit d'expérimentation sécuritaire n'oublions pas. Que l'utilisation de la, de l'Intelligence artificielle et pour l'heure dépourvues de cadre légal, même si un règlement européen est en cours d'élaboration. N'oublions pas non plus que l'expérimentation ne nous garantit aucun résultat. Comme son nom l'indique, on teste, on essaie mais on ne connaît pas son efficacité. Le droit au respect de la vie privée qui balayé d'un simple revers demain je suis au regret de vous dire qu'on ne balaie pas ainsi les droits fondamentaux en procédant de la sorte vous entaché la popularité des Jeux olympiques de Denis 24 cette magnifique et belle compétition porteuse de valeurs universelles. C'est pourquoi nous nous sommes opposés à votre durcissement sécuritaire tout azimut et ce même. Et ce même dans le cadre des manifestations sportives. Nous avons proposé de proportionnée certaines mesures comme le pointage ou encore vous montrez méthodiquement comment le tout répressif non notamment en matière d'engins pyrotechniques. En plus d'être inopérant va même à l'encontre du but poursuivi, à savoir la sécurité des supporters. Pour nous, le sport et ces manifestations constituent des moments festifs et de joie spontanée, bref une communion populaire à l'état pur. Or, votre penchant sécuritaire dans l'encadrement des manifestations sportives directement inspirée de la gestion des Coupes du monde en Russie au Qatar de feront que saper un élan populaire spontané pour un événement sportif majeur de plus. Comme nous l'avions dénoncés dans notre motion d'irrecevabilité, le recours aux agents de sécurité privés pour encadrer ces JO ne sera pas à la hauteur des enjeux. La sécurité privée ne doit pas être confondu avec la sécurité étatique au risque de se solder par un cuisant échec tels qu'essuyés par les JO de Londres en 2012. Cette délégation n'honore aura ni l'événement ni les professions de la sécurité publique. Par ailleurs, ce texte aurait dû constituer un engagement du gouvernement pour entreprendre une politique volontariste en matière de sport. L'héritage économique et social des Jeux fut au mieux survoler durant les débats pour ne pas dire totalement évacué et pourtant pourtant. Quel meilleur moment que celui où se tiendront les Jeux pour casser les barrières sociales territoriales ou encore celles liées au handicap entre usagers et pratique sportive le sport Madame la Ministre c'est un enjeu culturel et ce, tant au niveau professionnel qu'au niveau amateur. Si effectivement les jeux met à l'honneur. Nos athlètes de haut niveau et à travers nos fédérations sportives ne pas réfléchir à l'après-en matière d'accessibilité de la pratique sportive pour tous et toutes. Je vous le dis, Madame la Ministre c'est du gâchis. Enfin, s'agissant de l'accueil des Jeux dans des jeux. Notre groupe a posé la question. Lors des débats de l'anticipation des besoins en matière de capacité d'accès aux soins des hôpitaux avec la présence de milliers de supporters du monde entier. L'afflux de patients dans les hôpitaux de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, dont 15% des lits sont actuellement fermés par manque de personnel paramédical, nécessite une anticipation des besoins par l'État. Les besoins supplémentaires en lits d'hôpitaux et de recrutement de personnels doivent être immédiatement suivi de mesures tout en garantissant le niveau d'accès aux soins pour les patients franciliens. Si les besoins ne sont pas suffisamment anticipé l'agence régionales de santé devra déclencher le plan blanc pour mobiliser l'ensemble du personnel hospitalier, cela entraînera de facto la suspension des congés pour le personnel hospitalier, comme cela est d'ailleurs prévue pour les forces de l'ordre. N'oublions pas que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques va également impacter fortement la vie des fonctionnaires, mais également des salariés auxquels il sera demandé de travailler les dimanches autour des sites de compétition alors même que l'évaluation de la loi Macron de 2015 qui à déréglementer le travail du dimanche dans les zones commerciales les zones touristiques, les zones touristiques internationales et les gares à démontrer que l'ouverture du travail le dimanche n'a entraîné aucune aucune hausse de l'emploi ou de l'activité. Nous soutenons que la remise en cause du repos dominical pour les salariés est un geste d'antijeu sur nos droits sociaux le groupe CRCE considère que ce projet de loi libérale et sécuritaire ne respectent pas le juste équilibre entre sécurité et protection des libertés et droits fondamentaux il n'honore pas les Jeux olympiques et son esprit de fraternité en ce qui le porte de graves atteintes aux libertés publiques. Ainsi vous ne serait pas surprise. Madame la Ministre le groupe CRCE votera contre ce projet de loi.

Vous avez la parole. Elle comprenait déjà un certain nombre de mesures visant à répondre aux contraintes de l'organisation d'un événement d'une telle ampleur et à moins de deux ans des Jeux olympiques, il était nécessaire d'adopter plusieurs mesures complémentaires. Particulièrement en matière de dopage, de sécurité, de santé et quelques autres mesures d'ordre divers. Le groupe Union centriste est favorable à l'adoption de ce texte qui a été. Perfectionné par le travail de la commission des lois et des 2 autres commissions, saisie pour avis. Celle des affaires sociales, celle de la culture et puis bien évidemment perfectionner dans cet hémicycle, à l'article IV la rapporteure Agnès Canayer a eu la la subtilité de nous proposer un compromis qui prend en compte la nécessité d'une mise en conformité pérenne du droit français avec le code mondial antidopage tout en conservant la prudence nécessaire en matière d'examens des caractéristiques génétiques. preuve a fait oeuvre constructive. Concernant l'article 7 sur la vidéoprotection qualifié d'augmenter puisqu'il s'est vu consolidé tant en commission par l'introduction de garanties supplémentaires à tous les moments du développement et du déploiement de ces dispositifs que dans l'hémicycle par l'adoption de 2 amendements de nos collègues du Rhin et Tabarot qui vise à plus de transparence des fournisseurs en exigeant une déclaration d'intérêts et du personnel pour le recrutement. En discussion générale. Je me suis réjoui que le gouvernement et la commission des lois et eu là justement l'Intelligence de ne recourir à sept a qu'à titre expérimental. De manière limitée, limitée dans le temps limité dans l'espace limité à un cadre restreint et sans aucune utilisation de données biométriques. Il n'y a là aucune atteinte aux droits fondamentaux. Les données personnelles sont protégées puisqu'elles ne sont ni traité ni stockées ni collecter. Néanmoins, cela ne nous dispensera pas et c'est l'objet de la proposition 22 de la mission d'information sur la reconnaissance biométrique. Menée conjointement avec Jérôme Durain et Marc-Philippe Daubresse. De créer au-delà des Jeux olympiques. Un cadre juridique expérimental pour recourir à la reconnaissance biométrique en temps réel sur la voie publique sur la base d'une menace pré-identifier éventuellement, il nous faudra déposer une proposition de loi afin de permettre un débat serein, apaisé enfin sur ces sujets et démocratique. Bien sûr, sur ces questions d'avenir parce qu'il est nécessaire de nous protéger face au développement des usages aujourd'hui non régulé. Je tiens également à saluer le travail du rapporteur Claude Kern qui a intégré le principe de l'obligation de recourir à des titres d'accès infalsifiable afin de mieux lutter contre les fraudes perpétrées en recourant à de faux billets. Désormais les billets devront être nominatif dématérialisée et infalsifiable pour les manifestations sportives de grande ampleur, dont la jauge sera fixée par décret en Conseil d'État. Autre avancée de la commission culture, qui me semble importante à signaler. Le rapport de la Cour des comptes. À l'issue des jeux olympiques qui apparemment et paralympiques qui devra faire le bilan de l'Organisation du coup et de l'héritage de cet événement et être remis au Parlement dès le mois d'octobre 2025. Ce rapport devra également retracer l'ensemble des coûts engagés par l'État et les collectivités. Ce qui est. Ce qui permet bien sûr une transparence et nous la devons à nos concitoyens. Et je conclurai par là je je veux simplement saluer l'amendement proposé par la rapporteure Canayer et que nous avons adopté en séance qui prévoit expressément l'application du projet de loi dans les territoires ultramarins sont renvoyés à une ordonnance ce c'est notre collègue là natte et tout. Annie particulièrement rassuré par ses dispositions pour la Polynésie. Pour toutes ces raisons qui ont permis d'améliorer sensiblement la qualité de votre projet de loi Madame la Ministre le groupe Union centriste votera favorablement. À ce ce texte. Je vous remercie, cher collègue de votre attention. de votre attention. Notre collègue Jean Louis Masson. Pour la réunion administrative des sénateurs qui ne figure sur la liste. D'aucun groupe.

Madame le Ministre, chers collègues. Ce ce second texte que nous examinons puisque il y a plusieurs années, nous avons déjà eu un vote sur l'organisation des Jeux olympiques. Et je l'espère, le dernier, j'espère que maintenant. Les choses seront bouclés. C'est un texte qui n'est pas fondamental mais qui apporte un certain nombre d'ajouts et. Qui incorpore. Également un certain nombre. De dispositions à caractère plus ou moins expérimental qui s'ajoutent finalement. Ah je dirais aux problèmes spécifiques des Jeux olympiques, ces mesures que l'on ajoute sont des mesures qui sont supplémentaires et qui viennent je dirais. Compléter finalement l'arsenal alors. Je voudrais insister simplement sur la problématique. des aspects de sécurité. Je pense pour ma part que si pour les Jeux olympiques. On estime qu'il y a un certain nombre de dispositions à caractère sécuritaire qui doivent être prises en matière sportive, hé bien il est logique, il y a une certaine cohérence à ce que ces dispositions ne s'applique pas seulement aux jeux olympiques et donc moi je ne vois aucun inconvénient

C'est tout particulièrement le cas de la vidéo surveillance et. Ce ce texte apporte un petit complément et je dirais. Renforce finalement les aspects de sécurité, on a vu à de nombreuses reprises dans les stades et on il faut on n'a pas été obligé d'attente des Jeux olympiques pour voir qu'il y avait des problèmes et donc. A fortiori ce qui sera fait pour les Jeux olympiques, je me réjouis de ce que cela puisse être étendue. Ceci étant, il y a quand même un aspect on oublie trop souvent que les jeux Olympiques ne se passeront pas seulement à Paris mais se passeront également dans un certain nombre de villes où il va y avoir une sorte de décentralisation soit pour l'entraînement soit carrément pour l'organisation de certaines épreuves et dans ces villes, ce n'est pas toujours dans les villes c'est parfois même dans des des petites villes qui sont en bordure de grandes agglomérations d'agglomération et il y a une problématique car on parle d'installer la Wii sans surveillance de. De faire des investissements mais il est évident que la problématique. Pour Paris et la région parisienne n'est pas obligatoirement la même que la problématique pour les petites communes et les. Je dirais qu'ils sont en province et lesquels peuvent être confond Pour les petites communes et moyennes communes. Lesquelles. Si elles ont un équipement. Peuvent être confrontés à des difficultés. Or il y a quand même un point qu'il serait un important d'examiner, c'est le financement des équipements de vidéo-surveillance car il y a à un moment donné, il va y avoir des dépenses et les communes vont être obligés de faire des dépenses et ce qu'il faut savoir c'est que ces dépenses seront faites pour des Jeux olympiques, donc pour quelque chose à Caracas à caractère national. Et il est important que les régions puissent les subventionner et malheureusement. Actuellement les régions n'ont pas le droit de subventionner l'équipement des communes ont plusieurs conférences c'est un, c'est je pense un problème important. J'ai pas assez de temps pour pour m'expliquer depuis longtemps mais ça suffira.

Alors certes, contrairement à mon collègue Bernard Charlès intervenu pour notre groupe, dans la discussion générale. Je ne suis plus un grand sportif. Même s'il a été quelque peu de manière. Et surtout. Surtout, il continue à suivre avec assiduité, les performances des 2 sportifs nationaux. C'est l'occasion de saluer le parcours de le handballeur lors du dernier championnat du monde qui s'achevait ce week-end à Stockholm. Qui suit de près l'épopée de footballeurs à décembre Nous prenons le Tour l'habitude de perdre les finales. Espérons donc. Qu'Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France. Sortira vainqueur l'Automne. Et qu'une pluie de médailles. Ça va de 16 tombera pour les Jeux Olympiques. Vous comme dans mes chers collègues, je me réjouis que notre pays soit organisateur des Jeux olympiques et para-olympiques. Même si d'un point de vue strictement sportif. J'aurais quelques regrets dans le choix opéré par le CIO. Notamment au sujet des nouvelles disciplines a introduite. Le skateboard plutôt que le karaté. Le break Dance plutôt que la pétanque. Je n'aurais pas cacher ma ma satisfaction si ça avait été l'inverse mais sans doute. C'est une question de génération plutôt banlieues que ruralité. Toujours est-il que chacune a c'est-à-dire conscient du défi que représente l'organisation d'une TVA un tel événement pour notre pays et qu'il est impératif que Paris et la France accueille sans accroc. Vainement. Un accueil sans accroc de sport Steve d'abord c'est une nécessité qui vaut le sur le plan des soins avec l'installation d'un centre de santé dans le village olympique a pas olympique est une nécessité qui vaut également du point de vue de la lutte contre le dopage. De nouvelles techniques d'analyse demande donc être autorisé à la création des jeu c'est une bonne chose. Nous considérons que le dispositif proposé 100 relativement équilibré et que leur pérennisation comme on le prend pas le texte du Sénat n'est pas là pas être craignent. Un accueil sans accroc également pour la sécurité et la sécurité des personnes. Je ne vais pas refaire le débat articles que ce projet toutefois. Un attire particulièrement l'attention. Qu'on demande dans cet hémicycle, nous avons des craintes quant aux discussions de l'Arctique La peur d'une société sous surveillance automatisée à la mode en Willy elle est agité de manière excessive, mais il y a des fois où l'épouvantail se justifie, c'est le cas ici parce qu'en même temps que les algorithmes et autres Intelligence artificielle. S'affirme avec l'espoir de plus de sécurité. L'e-mail s'face et et sans discernement aussi. Bien entendu. Le projet présenté mesuré il marque même une satisfaction puis s'il n'y aura pas, pas question de reconnaissance faciale mais on consomme trop bien c'était méthode des petits pas. Nous savons comment les choses progressent par palier. L'introduction c'est-à-dire artificielle risque d'être une première en marche jusqu'au jour où, sous couvert de nouvel aménagement que les algorithmes seul n'aurait pas pu prévoir. Il faudra aller au-delà. Seulement, je ne crois pas que j'ai dispositif. Aurait permis d'éviter les drames qui ont eu lieu dans notre pays. Je pense à l'assassinat de Samuel Paty aurait Tam-Tam Charlie-Hebdo ou la nuit du 13 novembre 2015. Pas plus que l'algorithme ne l'aura empêché au mois de mai dernier lors du stade du match Stade de France c'est un. Un Chevènement des causes imprévisible pour reprendre les mots de la préfecture. Plus encore, je vais sentiment. Profond que l'idée présentant l'innovation technologique comme une solution évidente demeure une chimère potentiellement dangereuses. On me rétorquera peut-être que comme pour le choix entre la break Dance et le la pétanque. Ce n'est qu'une affaire de génération Auquel cas j'espère c'est un psy en manque. Vous aurez raison mais accordez-moi le privilège de douter. Vous comprenez donc mes chers collègues, que même si nous voterons ce texte nous ferons avec une certaine retenue. Notre groupe RDSE rappelle souvent son attachement à la liberté et aux libertés, nous savons qu'nos limites d'ailleurs nous avons déposé une série d'amendements visant à durcir les conditions d'usage par l'administration du mécanisme de surveillance Al Gore rythmiques nous tant qu'il n'est pas trouvé. D'ici favorable au sein du Sénat toutefois nous ne sera pas obtus, si nos amendements n'ont pas convaincu. D'autres ont été retenus et participeront à mieux garantir les droits et libertés de nos concitoyens. Au regard de ces tous ces éléments, l'article 7 remodeler offrent davantage de satisfaction que sa rédaction initiale, malgré les réserves que j'ai vu une évoquer sur notre sujet, ce projet de loi introduit la possibilité de mettre en place des scanners corporels entrer enceintes. Dans lesquelles est organisé une manifestation sportive ou récréative ou culturelle. Nous sommes satisfaits du travail du Sénat qui aille à suis améliorer le dispositif initial, notamment avec l'adoption en commission de la manne de masse de notre collègue Maryse Carrère je dirais également un mot du volet pénal de cette ce projet. Le texte initial qui nous a été soumis, renforcer les sanctions des violences commises à l'occasion d'une manifestation sportive enfin semblait s'est positionné en faveur du davantage de fermeté. J'y trouve mon compte, je ne crois pas qu'il faille admettre. De souplesse particulière notamment au regard de la nature médiatique et. Systématique et des violences dans le sport et en particulier dans les stades avec et cela achèvera bon propos j'aimerais dire notre satisfaction à l'adoption de la même de l'amendement de notre collègue Nathalie Delattre que le groupe RDSE soutenait largement. Elle nous a partagé sa crainte de voir disparaître. Des plages à l'issue des jeux Olympiques. Le corps du maîtres nageurs sauveteurs CRS. La position du gouvernement, cette question nous rassure et nous retrouverons les CRS donc maître nageur sur les plages en 2025. Et si pour toutes ces raisons, vous comprendrez que le groupe RDSE dans sa grande majorité votera en faveur de ce projet de loi. Je vais donner la parole de notre collègue Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, rapporteur du texte. Je m'exprimerai aujourd'hui en tant que membre de mon groupe. L'organisation de ces Jeux présentera des défis considérables, tant sur le plan de la sécurité que de l'organisation des compétitions ou encore de la lutte contre le dopage. Les jeux de Paris 2024. Après plus d'un siècle d'attente devrait rassembler près de 13,5 millions de spectateurs, 4 milliards de téléspectateurs. Et se tiendront sur 37 sites à travers la France des berges de la Seine aux rivages du Pacifique en Polynésie française. En outre, ce projet de loi nous parvient, quelques mois à peine après les événements de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai 2022. Ces événements avaient alors conduit la commission des lois et de la culture a consacré une série d'auditions sous l'égide des présidents buffet et la font. Le rapport qu'il rédigeait alors prenait un ensemble de réflexions et préconisations utiles qui contribuèrent grandement à guider nos travaux actuels. C'est donc avec une conscience des enjeux et un esprit de responsabilité, que nous avons abordé ce texte déposé par le gouvernement. Ce dernier comprenait 3 pans principaux le 1er concerné les problématiques de santé et de dopage. Le second, les questions de sécurité et le dernier un certain nombre d'ajustements plus varié. Premièrement, sur la question du dopage, il nous faut il nous fut initialement proposé de déroger à la législation française pendant la durée des Jeux. Afin de nous conformer aux exigences du CIO en matière de lutte antidopage, c'est-à-dire de nous aligner sur le code mondial antidopage. Après avoir soigneusement étudié la question, nous avons privilégié une mise en conformité plus durable du droit français aux normes internationales entourée de garanties appropriées à la nature des examens des caractéristiques génétiques dont il est question. Grâce à cela, la France sera en conformité avec le droit international pour les futurs événements sportifs. Après tout ces jeux n'ont pas vocation à être la dernière compétition internationale à se tenir dans notre pays avant d'éventuels nouveaux jeux au siècle prochain. Toujours dans le domaine du dopage. Nous avons également fait en sorte de conforter les dispositions spécifiques à la Polynésie française en bonne intelligence sénatoriales avec la collectivité de Polynésie et le gouvernement. Le 2ème pan du texte qui fut plus discutée consacré à la question de la sécurité. Cette dernière est un enjeu majeur d'autant plus que certains événements tels que la cérémonie d'organes d'ouverture organisé le long de la Seine nécessiteront un déploiement inédit de nos forces de police et de de gendarmerie afin d'en garantir le bon déroulement. l'expérience récente du Stade de France doit nous servir de piqûre de rappel et prévenir de toute menace. Il nous faut être exigeant et au rendez-vous attends c'est pour cela que nous avons retenu l'utilisation de traitements algorithmiques pour les images des caméras, l'expérimentation de ce dispositif de vidéoprotection intelligente pourrait constituer un atout indéniable dans l'identification et la neutralisation rapide des risques liés aussi bien aux terroristes qu'au mouvement de foule inopinée naturellement nos débats tout au long des travaux autour de ce texte, l'ont montré l'emploi de telles technologies a pu générer des inquiétudes que nous comprenons. Le rapport de nos collègues Daubresse de Belenet et du hein. C'était d'ailleurs abondamment penché sur les tenants et les aboutissants de cette technologie. Pour cette raison nous avons perfectionné le dispositif en affinant son objet en améliorant l'information du public et en entoura en entourant l'usage des données collectées de garanties supplémentaires. Dans ces conditions, l'expérimentation de la vidéoprotection intelligente devrait simultanément permettent de contribuer à la sécurisation des jeux et nous permettent d'évaluer en situation réelle. Les mérites de cette technologie. Notre démarche similaire pour d'autres dispositifs quel tels que le recours aux scanners à ondes millimétriques ou la mise en conformité avec le droit européen de la protection des données personnelles. Par ailleurs les travaux menés avec la commission de la culture, autour des outils de lutte. Contre les entrées frauduleuse ou violence en récidive dans les enceintes sportives ont également permis de renforcer considérablement le texte initial. Une question importante a également retenu notre attention dès les auditions. Même si elle demeurait nécessairement peu présente dans le texte lui-même la question des coûts et de l'héritage. La candidature parisienne se voulait offrir comme les plus sobre. Et écologique de l'histoire récente grâce à l'usage d'infrastructures existantes et à la mise en place d'un héritage durable et utile dans les mots mêmes de madame la Ministre devant notre assemblée. C'est effectivement un impératif si nous souhaitons conserver l'adhésion des Français à l'organisation des Jeux, c'est pour assurer cette transparence démocratique, que nous avons prévu la remise par la Cour des comptes d'un rapport sur les coûts et l'héritage des Jeux. En outre, et cela relevait presque autant de la rigueur juridique que de l'esprit olympique et para-olympiques. Nous avons souhaité élargir la possibilité d'obtenir de nouvelles autorisations de stationnement pour les taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nos travaux ont donc permis vous le voyez de grandement consolider le texte initial en le rendant à la fois juridiquement plus solide et cohérent et plus protecteur sur le plan des libertés individuelles. Et si cette tâche est effectivement ardue. Nous ne pouvons qu'encourager tous les acteurs des Jeux olympiques et para-olympiques de 2024. En leur rappelant les paroles du baron Pierre de Coubertin chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. 542 c'est le nombre de jours qui nous séparent de la grande fête universelle du sport soyons au rendez-vous vous l'aurez compris, notre groupe votera donc ce projet de loi. Merci ma chère collègue. Chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 de notre règlement au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi dont l'intitulé. Est modifié, projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. Le scrutin est ouvert. Mais je vous invite. Ah insérer votre carte de vote dans le terminal. Et de l'laisser jusqu'à la fin du vote.

Plus personne ne demande à voter donc.

Le scrutin est clos.

Résultat du scrutin 113 nombre de votants, 338. Nombre de suffrages exprimés, 273 pour l'adoption, 245 contre 25. Le Sénat a donc adopté.

Mesdames, et messieurs les sénateurs, je voudrais évidemment au nom du gouvernement et avec mes collègues, Clément Beaune, notre ministre des Transports me fait. L'amitié d'être présent à mes côtés pour ce moment important également au nom du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Je voudrais vous remercier pour cette adoption la saluer, vous dire que c'est évidemment un jalon indispensable dans notre préparation aux Jeux olympiques et paralympiques évidemment l'ensemble des membres des commissions qui ont été très à la à la manoeuvre dans l'amélioration de ce texte dans cette adoption. Merci Agnès Canayer. Merci Claude Kern merci Florence là s'arrêtent pour la minutie, avec laquelle vous avez travaillé. Et votre engagement derrière tout ça. Ainsi pour la richesse de nos échanges des apports importants de la part du sénat je pense à la mise en place de cette billetterie infalsifiable dématérialisée. Je pense aux équilibres trouvés sur la prévention de toutes les formes de violence dans nos stades ainsi que le renforcement de notre dispositif contre le, contre Certes pas réussi à vous convaincre tous mais je sais que tous vous êtes engagés derrière la réussite de ces Jeux olympiques et paralympiques et je voulais aussi vous dire que j'avais été très attentive à vos interventions pour aussi placé plus largement que les Jeux olympiques, la place du sport un peu plus au coeur de notre société. Monsieur le Sénateur requis, y compris le rugby. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Je vais maintenant suspendre la séance elle sera reprise. À 15h 50. Pour l'examen de la proposition de loi visant à régulariser le père lui de la communauté de communes du Chablais.

Chers collègues, la séance est reprise.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, madame la rapporteure madame la présidente de commission, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi déposée avec ma collègue Sylviane Noël ainsi que pour l'avis favorable de la commission des affaires économiques et sa rapporteure maintien d'RTL pour le travail effectué. Si j'le qu'il est inhabituel. Ce texte est d'une importance capitale pour notre département de la Haute-Savoie et tout particulièrement pour le territoire du Chablais. En ce qui permettra la réalisation d'une autoroute reliant à Thonon projets structurants est attendu depuis des années par les Chablaisiens. Pour replacer le contexte de cette proposition de loi, il faut rappeler que le Chablais très attractif à la fois du fait de sa proximité avec la Suisse de son dynamisme économique à et de son potentiel touristique. Cette activité entraîne logiquement d'importants flux de véhicules et ce malgré les efforts faits pour développer le ferroviaire et les modes de circulation alternatifs. Je pense par exemple au Léman Express inaugure en 2019 ans dans l'objectif de 50.000 usagers par jour, été largement dépassé et qui transport désormais plus de 65.000 personnes quotidiennement au RER Sud-Léman ou encore au vélo route des 5 lacs dont je préside les Covid et les copines pardon et qui sont en cours d'étude. J'espère d'ailleurs Monsieur le Ministre que vous tiendrez le RER Sud-Léman pour son inscription au CPER. Il ne peut donc de fait le reproche de privilégier la route au détriment du train et je tiens à souligner et félicité la pleine mobilisation des élus du Chablais en faveur de l'inter modalité. Le report modal est évidemment un objectif louable et nécessaire, qu'il faut encourager. Mais j'estime qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature et qu'il conduisent à empêcher des projets routiers pourtant totalement nécessaire. Il faut rester réaliste. Certains automobilistes n'ont tout simplement pas la possibilité de prendre les transports en commun pour des raisons d'accessibilité ou tout simplement car les horaires ne correspondent pas à leurs besoins. En outre, la liaison Bachy tenons est exemplaire d'un point de vue environnemental, son impact sur la consommation de terrains sera compensée et il est prévu d'intégrer des innovations permettant de réduire les émissions de CO2 tels que le développement de mobilité flux libre électrique ou encore le covoiturage. Ce projet d'autoroute est nécessaire et même urgent car le Chablais n'est reliée que par des routes départementales. Le réseau routier n'est donc pas à la hauteur des enjeux rencontrer. Il en résulte un enclavement très important du territoire qui entraîne le passage d'un nombre excessif de voitures et de poids lourds dans les centre-villes bourgs et hameaux et qui conduit à des embouteillages très conséquent. Ces passages engorgement incessants pose de graves problèmes de sécurité et de tranquillité publique et engendre une forte pollution. Rendez-vous compte que certaines communes du Chablais, de 4000 à 5000 habitants voit chaque jour passé jusqu'à 22.000 véhicules à proximité des écoles, des commerces et habitations. Certaines, à l'image de Brenton sont tout bonnement coupé en 2 par la départementale tandis que d'autres s'inquiètent du risque d'accident à leur passage à niveau. En heure de pointe. Un trajet qui devrait durer 40 minutes en prend le double, soit près d'une heure et demie et consomme bien plus de carburant qu'un cas de circulation fluide. Dans ce contexte, l'État, les collectivités, mais aussi et surtout les habitants du Chablais qui soutiennent massivement le projet d'autoroute. Ont de longue date souhaité remédier à la situation. C'est ce qui a à conduire dès la fin des années 80 à étudier la création du tronçon autoroutier qui nous occupe dans le but de désenclaver le territoire. Le projet a cependant été perturbé à maintes reprises et ce n'est qu'à partir de 2015, qui a pu voir lieu un développement significatif avec la publication du projet. Chacune des étapes de procédure prescrites par la loi ont par la suite était avec diligence, qu'il s'agisse des consultations et enquête publique ou des études environnementales et ce jusqu'à la déclaration d'utilité publique intervenue fin 2019. Mettant aux compatibilité les PLU des communes concernées par le tracé. Pourquoi alors ce n'est aujourd'hui devant vous avec ma collègue Sylviane Noël pour vous demander d'adopter cette proposition de loi visant à sauver ce projet structurant pour le département. Si l'ensemble des prescriptions a été suivi à la lettre. Car concomitamment à la procédure de déclaration d'utilité publique, la communauté de communes du Bachabélé a prescrit en 2015, élaboration d'un 1er PLU intercommunal le contenu de ce pays lui a été arrêté définitivement en juillet 2019, soit avant l'intervention de la DUP qui a eu lieu le 24 décembre de la même année. De ce fait, même si la future autoroute est prise en compte dans d'autres composants du pays lui telle que la stratégie de mobilité et les enjeux environnementaux les zonages retenue ne font pas apparaître l'emplacement réservé au projet et le règlement ne comporte pas les règles écrites nécessaires à la réalisation des travaux puisqu'il n'était pas possible d'inclure un projet non encore définitivement arrêté par le biais d'une DUP. Il en résulte donc que malgré le fait que la déclaration d'utilité publique visait justement à mettre en conformité les documents d'urbanisme, l'adoption du pays lui après la publication de la DUP a entraîné une primauté du pays lui empêchant la réalisation du projet d'autoroute faut dit avoir fait figurer les éléments requis. Il était impossible pour le PCI de corriger le Tir une fois la des huppés publiée qui a le droit de l'urbanisme n'autorise aucune modification du projet de document. Une fois celui-ci a arrêté il n'y avait donc pas de moyen d'inclure le projet sans que la communauté de communes ne commettent un vice de forme. Entachant la procédure d'il y d'illégalité. En l'état le projet autoroutier donc irréalisable alors même que toutes les études et procédures nécessaires ont été mises en oeuvre, que les collectivités concernées sont toutes favorables et ont d'ores et déjà investi pour sa réalisation, que l'ensemble des autres documents d'urbanisme tels que le Scott et Le Strat dette prennent en compte le projet et ont mis en oeuvre les coûteuses études nécessaire que tous les documents sont purgées de recours et que 90% des habitants du territoire sont en faveur de la création de cette autoroute. Cette situation résulte d'un véritable casse-tête juridique combiné à un concours de circonstances et est tout bonnement impossible de trouver une solution autre que législatives sans mettre en danger l'intégralité du projet. En effet un nouveau décret pourtant déclaration d'utilité publique serait considéré comme un détournement de procédure et une révision du P. lui ou attendent adoption du nouveau pays lui de la communauté d'agglomération prendra environ 3 ans. Or cette échéance n'est pas compatible avec les délais requis pour l'appel d'offre et entraînerait une remise en cause du projet dans sa totalité. C'est pourquoi la proposition de loi que vous examinerait aujourd'hui vise tout simplement appliquer la mise en compatibilité prévue par le décret au pays lui du Bachabélé. Elle s'inspire du mécanisme de validation législative. La seule différence étant qu'il n'a pas d'effet rétroactif. Ce qui la rend bien moins susceptibles de porter atteinte à la sécurité juridique. Elle respecte par ailleurs en tout point la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de validation législative telle que je voulais des qui était, Mais avant je souhaite ouvrir une parenthèse sur le fait que la problématique rencontrée par les élus du Chablais doit nous conduire plus largement à nous interroger sur la complexité du droit de l'urbanisme et les obligations contradictoires que celui-ci fait peser sur les collectivités. Car si des lois telles que celle que nous étudions aujourd'hui, ils peuvent être admises exceptionnellement, je suis bien évidemment conscients qu'ils ne doivent pas se multiplier. Or c'est ce qui nous attend si nous ne faisons pas en sorte de réduire l'amas des textes législatifs et réglementaires ayant trait à l'urbanisme. Je referme la parenthèse et revient sur les raisons pour lesquelles une proposition de loi respecte la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui prévoit plusieurs critères cumulatifs. Que la loi poursuivent un objectif d'intérêt général. Qui ne me connaissent pas de principes à valeur constitutionnelle, à moins que l'objectif d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle qu'il respecte les décisions de justice et enfin que la portée de la validation soit strictement définies. Premièrement, elle répond à des objectifs d'intérêt général de préservation de la République d'abord qui lui même un objectif de valeur constitutionnelle. On sait que la réalisation de l'autoroute permettra de remédier à un problème de sécurité et de tranquillité publique. Économique de par an, ce qui évitera aux collectivités à l'État de réengager de coûteuses études, qui ont déjà été faites. Écart un retard dans la réalisation du projet en tiendra une forte hausse des coûts. Enfin, l'objectif est également environnementales et de santé publique hein puisque cette liaison permettra de réduire la pollution due aux bouchons et passage incessant de véhicules. Il est en effet pas prévu d'augmentation du trafic seulement un report hors des centres-villes. De même le droit au recours est respectée puisque tous les recours ont été purgés enfin à la portée strictement définies puisque la proposition de loi vient de manière très précise mettre en compatibilité le pays lui sans laisser aucune porte ouverte. En outre, aucun objectif de valeur constitutionnelle n'est méconnu. Certains pourront arguer que c'est le cas pour l'objectif de protection de l'environnement. Or le projet de Toulouse vise au contraire à atteindre cet objectif et la consommation d'espace sera compensé. Je pense qu'un sincèrement que sur le long terme, ce projet sera plus bénéfique pour l'environnement qu'en laissant les choses en l'état et j'ai oublié mes chers collègues, de ne pas y formuler une opposition de principe. Uniquement car si il sait car il s'agit d'une autoroute. Je ferais enfin une dernière au Mac à part une poignée de locaux qui s'y opposent et c'est le jeu, on ne peut pas mettre absolument tout le monde d'accord, je ne vois que des personnes étrangères au Chablais se positionner contre le projet. En revanche je ne crois pas avoir entendu l'un d'entre eux. Qu'il ne faut pas du Chablais. Non, non. Les personnes qui sont comptes sont principalement de secteur d'Annecy et d'autres départements, Toulouse, Bordeaux, Lyon, mais les associer. Si on chablaisien. Écologistes n'ont pas pris position contre, en revanche je ne crois. Pas avoir entendu la tromperie rende publiquement la parole en faveur des projets. RER Sud-Léman ou vélo route des cinq lacs comme je vous dis, chers collègues, je préside ces 2 comités de pilotage et aucun soutien sur les projets ferroviaires ni d'autoroute ni de en vélo des saints. Donc je vous encourage aussi à les soutenir. Donc c'est 2 poids 2 mesures pour et c'est pour toutes ces raisons et au regard de l'immense nécessité que représente la réalisation de cette autoroute pour mon territoire et pour je cite ici les élus de Thonon agglomération ne pas les laisser de côté dans le développement de la région et ne pas créer un territoire de vitesse. Je vous invite mes chers collègues à voter en faveur de cette proposition de loi, je vous remercie. Très bien. La parole est maintenant le rapporteur, madame Martine Berthet. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues. Chacun des textes qui nous est donné d'examiner dans cet hémicycle dans cet hémicycle est toujours bien différent des précédents, c'est ce qui fait la beauté et l'intérêt du travail du Parlement. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui présentée par nos collègues Cyril belva et Sylviane Noël et peut être un peu plus atypique encore. D'aspect assez techniques de prime abord, ce texte nous adresse en fait à nous représentant des territoires français, une question très concrète, souhaitons-nous qu'un projet d'infrastructure d'intérêt général. Déjà passé par l'ensemble des étapes administratives nécessaires à sa réalisation soit mise en échec du simple fait de l'enchevêtre ment de procédures d'urbanisme parallèle. Parlementaire comme élus locaux savent que le cadre juridique du droit de l'urbanisme a été considérablement modifié et j'ose le dire complexifiée au cours des 2 dernières décennies. Les documents d'urbanisme locaux se sont multipliés les procédures formelles qui préside à leur élaboration se sont rigidifiés et allonger l'insécurité juridique qui les entourent s'est fortement accrue. Il faut désormais entre 4 et 6 ans pour élaborer un plan local d'urbanisme et peu de maires et présidents d'EPCI sont aujourd'hui en capacité de le faire sans recourir à des prestataires externes le fête intercommunale, s'il a accentué les solidarités et le dialogue territorial s'est révélé lui aussi source de complexité nouvelle au fur et à mesure des créations puis des fusions de PCI et des divers transferts de compétences écrire un PLU pour une commune comme auparavant et sans comparaison avec l'écriture d'un pays à lui couvrant 20 50 voire 100 commune. Je rappelle aujourd'hui ce contexte de complexité et d'instabilité juridique car il est essentiel pour appréhender pleinement la démarche de la proposition de loi qui nous est soumise. Dans ce cas concret, l'ensemble des collectivités territoriales du bas Chablais travaille depuis plusieurs décennies à la réalisation d'une liaison 2 fois 2 voies entre Massy et Thonon-les-Bains qui mènerait à bien le désenclavement du bassin répondrait à son développement rapide et assurerait la sécurité des riverains. En 2017, ces collectivités accompagné de l'État ont donné une nouvelle impulsion au projet de liaison routière avec le lancement d'une concertation publique la conduite d'une évaluation environnementale, puis en 2019 la prise d'une déclaration d'utilité publique afin de prendre en compte le projet dans sa globalité et de faciliter sa réalisation cette déclaration d'utilité publique a prévu comme le lui permet. Le droit, la mise en compatibilité simultanée des plans locaux d'urbanisme des 10 communes concernées par le tracé. Cette DUP a ainsi ouvert la voie à la réalisation du projet très attendu par les parties prenantes. C'est là qu'intervient le contexte particulier que j'évoquais tout à l'heure, la communauté de communes du Bachabélé avait lancé l'élaboration d'un PLU intercommunal. En 2015, c'est-à-dire avant la relance du projet de liaison 2 fois 2 voies entre temps devenu communauté d'agglomération, elle a finalisé ce PA lui début 2020. Si la déclaration d'utilité publique du projet routier avait bien prévu la modification des anciens plans locaux d'urbanisme elle n'avait pas prévu que l'adoption du nouveau lui viendrait peu après écraser ces modifications. Comble de la situation. Une fois ces difficultés identifiées. Il s'est avéré à la fois impossible pour la communauté d'agglomération de modifier son PA lui avant approbation puisque celui-ci avait déjà été soumis à concertation et enquête publique. Est impossible pour l'État de prendre une DUP modificative puisque la jurisprudence du Conseil d'État ne le permet pas, à projet constant. Qui plus est, toute modification du lui à peine adoptée devrait passer par la procédure la plus contraignante qui reprendrait une à une toutes les étapes d'évaluation de concertation de concertation d'enquête publique déjà effectué. La démarche de la proposition de loi bien qui atypique et donc très simple, elle vise à étendre les effets de la mise en compatibilité prévue par la déclaration d'utilité publique au nouveau plan local d'urbanisme afin de permettre au projet de de se poursuivre sans délai injustifié. Eu égard à son caractère atypique. Notre commission a souhaité examiner ce texte avec une exigence toute particulière en le passant au filtre de plusieurs critères concrets. Premièrement nous avons vérifié que ce texte ne vise aucunement à faire échec à des décisions déjà prises à aller à l'encontre des compétences des collectivités ou bien à restreindre des droits acquis, notamment en matière de droits de recours. Nous avons pu constater qu'il s'agit bien d'un texte, et dans et pas d'un texte de censeur. Les collectivités territoriales du bas Chablais m'ont confirmé que la situation actuelle ne relevait pas d'une volonté locale de freiner le projet mais bien d'une erreur dans la conception simultanée de la DUP et depuis du PS lui le tout dans un contexte juridique complexe. Le projet est anticipé et soutenu de longue date par tout le territoire, l'ensemble des autres documents d'urbanisme Scott sera dette notamment le prennent déjà en compte et le qualifie de projet structurant pour la région. Surtout, le projet a fait l'objet de la totalité des modalités de concertation de participation du public d'accord des collectivités et de droits de recours prévues par la loi, notamment une concertation publique sous l'égide de la Commission nationale du débat public. La déclaration d'utilité publique est aujourd'hui purgé de tout recours et les quelques contentieux ont été rejetées par la justice. L'examen de cette proposition de loi n'est donc pas l'occasion de revenir sur le fond du projet autoroutier qui a déjà fait l'objet de décisions administratives et de décisions de justice. Deuxièmement notre commission a vérifié qu'il n'était pas possible de parvenir au même objectif par une méthode alternative qui ne passe pas par la loi. J'ai notamment explorer 3 pistes une nouvelle DUP un nouveau PA lui une révision du PLU comme évoqué tout à l'heure c'est trois options n'offre pas de solution viable soit par impossibilité juridique soit par impossibilité pratique. En particulier, elles impliqueraient des délais intenables, d'une part, car la DUP existantes arrivera à son terme en 2029. D'autre part, car la situation actuelle d'engorgement du Bachabélé est source de nuisances et de risques réels. Troisièmement et pour finir, nous avons souhaité mieux comprendre l'objectif d'intérêt général de ce texte. En ce qui le permet la réalisation d'un projet d'infrastructure essentielle pour la région, dans lequel les collectivités et l'État sont déjà très engagés. Nous avons pu constater l'urgence et l'importance du désenclavement du bas Chablais dans la droite ligne des objectifs de réduction des inégalités territoriales et de développement équilibré des territoires. L'absence d'infrastructures à la hauteur des enjeux est perçue par la population et les collectivités territoriales comme une condamnation comme une relégation. Les accidents, la pollution, les nuisances sonores touche directement le coeur des villages et des hameaux. Pour toutes ces raisons, nous avons pu constater que l'ensemble des collectivités territoriales et la grande majorité de la population soutiennent ce projet d'intérêt général. La CNDP a confirmé que seuls 10% des participants à la concertation, s'il était déclaré défavorable témoignant d'un réel consensus local. Les communes concernées ont toutes rendu un avis favorable à la déclaration d'utilité publique et nous l'ont récemment confirmé enfin aucun des recours en justice contre le projet n'a abouti. À l'issue de ces travaux. Notre commission des affaires économiques a donc estimé que cette proposition de loi en dépit de sa démarche atypique poursuit un objectif qui mérite d'être soutenue. Elle vise à remédier à des difficultés concrètes d'application du droit de l'urbanisme, mettant en danger un projet d'intérêt général, soutenue par les parties prenantes sans qu'il existe d'alternative satisfaisante à cette solution législative en commission. Nous avons donc adopté cette proposition de loi sans modification et porteront dans cet hémicycle la même position. Il serait dramatique dans un pays comme la France où l'on appelle chaque jour et surtout dans cette assemblée, à la résorption des inégalités territoriales à la réindustrialisation ou encore à la simplification du fardeau administratif que nous sacrifions sur l'autel de la complexité juridique. Un projet d'intérêt général unanimement reconnue alors même qu'une solution existe. Le projet qui évoque cette proposition de loi a franchi avec succès toutes les étapes prescrite par la loi. Il faut maintenant qu'il puisse être menée à bien, car il est extrêmement attendu. Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre délégué chargé des Transports, monsieur Clément Beaune. Merci beaucoup monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Le texte qui vous est présentée aujourd'hui vise, cela a été dit à permettre la réalisation d'une liaison autoroutière entre les communes de machines de Thonon-les-Bains dans le département de Haute-Savoie. Le Bachabélé plus largement le département de la Haute-Savoie, attendent depuis longtemps, la réalisation de cette liaison pour laquelle il convient de pouvoir aujourd'hui avancer. Bien que reconnue d'utilité publique en 2019 la construction de cette liaison nouvelles et de fait aujourd'hui à l'arrêt car les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal le lui de la communauté de communes du bas Chablais adoptée en février 2020. Ça verte en l'état incompatible avec le projet d'infrastructure. Or cela été bien expliqué j'y serai donc bref dans cette intervention il ressort que cette incompatibilité entre le paie lui du Bachabélé et le projet autoroutier ne semble pas résulter d'une décision délibérée des collectivités mais plutôt d'une erreur de traduction au sein d'un document d'urbanisme, d'un projet anticipé longuement débattu et il convient donc d'y apporter une solution. Cette intervention législative qui est proposé Merci théoriquement juridiquement possible de faire évoluer le paie lui du bas Chablais par des procédures classiques, voire d'attendre qu'un nouveau lui puisse être élaboré par la collectivité. Mais les délais qu'impliquent ces procédures le par l'ensemble des nouvelles et différentes étapes à franchir serait extrêmement long pour un projet qui se trouve avoir déjà apporté toutes les procédures. Toutes les suivi toutes les procédures requises et apporter toutes les garanties demandées ce choix relève désormais de manière exceptionnelle et spécifique d'une décision démocratique, parlementaire, ce qui montre bien que là encore des garanties sont requises dont je laisserai évidemment juge le Sénat dans ce vote. Vous l'avez, je crois, parfaitement éclairés. Monsieur le sénateur Pell madame la rapporteure. J'entends évidemment cela et mon devoir de les rappeler un certain nombre d'arguments d'opposants au projet qui sur le terrain comme peut être dans l'hémicycle s'oppose à ce projet en tant que telle, en tant que projet routier. Vous le savez je partage très clairement la volonté de réduire encore et davantage l'impact environnemental de nos infrastructures de nos mobilités de décarboner au maximum et le plus rapidement possible nos transports c'est ce à quoi je m'attache en encourageant notamment les crédits du réseau ferroviaire en soutenant. Dans la sillage du rapport du conseil d'orientation des infrastructures qui sera très prochainement présenté à la Première ministre dans les arbitrages qui seront en préparation et soumis à votre assemblée à l'ensemble du Parlement pour mobiliser des crédits en faveur du report modal du domaine ferroviaire et de la transformation de nos infrastructures. Toutefois, il faut aussi être clair, réaliste et pragmatique. Tous les villages de France ne seront pas désormais demain accessible par le train ou par ce qu'on appelle mobilités douces en un instant et en un clin d'oeil, l'usage de la voiture reste évidemment complémentaires et indispensable dans de nombreux territoires, et ce tout particulièrement aux jeunes rurale ou en zone de montagne. Disons-le clairement, ce n'est pas simplement. De moins de transport routier dont nous avons besoin, c'est aussi le transport routier adapté plus durable qui permet plus de transports en commun plus d'électrification plus de partage de nos usages le covoiturage ou l'autopartage à chaque fois que cela est possible et nous l'encourageons l'ennemi de leurs l'ennemi n'est pas la voiture en elle-même la route en elle même c'est l'usage individuel et polluants des véhicules sur lesquels nous devons agir, c'est sur ces alternatives sur ces transformations que nous devons travailler et accélérer. En outre, et c'est heureux, les standards environnementaux de nos infrastructures les plus traditionnels, si je peux le dire comme la route évolue, s'améliore. Hé bien qu'une infrastructure sans impact n'existe pas. Nous avons fait beaucoup de progrès collectivement en matière de traitement de l'eau le protection de la biodiversité en particulier j'insiste donc à cet égard cela été rappelé sur le fait que le projet en question répond à toutes les garanties environnementales en vigueur par nos réglementations et législations et que le Conseil d'État d'ailleurs écarté. Cela a été précisé par décision du 30 décembre dernier, l'ensemble des contentieux qui. Rappelons enfin que la route qui existe aujourd'hui entre Massy étonnons souffre de congestion n'offrent pas les garanties de sécurité élémentaire et suffisante, ce qui est aussi non seulement un problème de sécurité mais un problème mais un problème environnemental par ces blocages ou engorgement le trafic ainsi engendré. L'État soutient depuis le départ, ce projet de liaison autoroutière qui est souhaité très largement et très ardemment par les les collectivités locales par beaucoup de membres du Sénat à l'origine du texte. Je les salue et je tiens à saluer en particulier le sénateur Pell va la sénatrice Noël ainsi que Loïc Hervé impliqués aussi dans ce projet utile au développement du territoire et répondant, je le rappelle à l'ensemble des exigences posées. Si le recours à la loi pour modifier un peu lui. Doit rester exceptionnelle, j'y insiste, il appartient au législateur au sénatrice aux sénateurs aujourd'hui rassemblés. l'apprécier l'opportunité j'en ai indiqué je crois l'importance nous donnerons donc au nom du gouvernement, un avis de sagesse à cette proposition de loi, je vous remercie. Très bien. La parole est maintenant Monsieur Salmon pour le groupe écologiste solidarité et territoires. 4 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure. Chers collègues, je suis élu de cette assemblée depuis le mois de septembre 2020. Et je dois avouer que je ne pensais pas en tant que sénateur, à voir à m'exprimer sur un texte de cette nature et en Bretagne, département d'Ille-et-Vilaine il m'appartient de me prononcer sur le document d'urbanisme d'une communauté de communes situées en Savoie je Haute-Savoie veuillez m'en excuser. Je me sens quelque peu déconcerté. Vous voyez bien que c'est un peu loin. Comme beaucoup d'entre vous, je suis également élu local et je considère que les règles d'urbanisme auxquelles sont soumises les collectivités territoriales sont les mêmes sur l'ensemble du territoire. Nous avons toutes ces tous déjà été confrontée à une révision d'un PLU ou encore la mise en conformité pour permettre à la réalisation d'un projet quel qu'il soit certaines certes, ces règles sont parfois complexes fastidieuse longue et coûteuse mais elles sont la garantie d'un aménagement du territoire, respectueux des principes du développement durable d'une gestion économe de l'espace, elles sont la garantie de répondre aux besoins de développement local en tenant compte des politiques nationales et territoriales d'aménagement et des spécificités d'un territoire. J'ajoute que ces règles sont aussi la garantie via les enquêtes publiques de fournir une information éclairée sur les projets d'aménagement aux citoyens d'un territoire et ce n'est pas négligeable. Il est pourtant d'autant plus difficile de se faire un avis sur l'origine de ce problème qui amène cette PPL que d'un côté, les auteurs de la proposition de loi plaide pour une négligence des élus et de l'autre côté, j'ai été destinataire de plusieurs contre-arguments qu'il avance que les collectivités concernées étaient pleinement informés des risques encourus. En me penchant de plus près, j'ai découvert un véritable serpent de mer revenant régulièrement dans l'actualité, à savoir une liaison autoroutière entre ma machinerie et Thonon les Bains qui fait l'objet d'un combat acharné entre ses opposants et partisans depuis plus de 30 ans. Je vais m'attacher à m'interroger sur la forme de la et la procédure. Si on nous demande aujourd'hui de faire prévaloir la Duper de ce projet autoroutier par par rapport aux pays lui c'est uniquement parce que le nouveau PLU, il crée pour le bas Châtelet ne mentionnait pas une nationale initialement ce projet d'autoroute. Malgré les demandes formulées par l'autorité environnementale et la sous-préfecture demande qui aurait nécessité la réalisation d'une évaluation environnementale et donc un rallongement des délais. La loi est ainsi faite, on peut se demander pourquoi tout cela n'a pas été pris en compte. C'est donc pour cela que nous sommes amenés à étudier cette proposition de loi pour réparer ce qui serait, selon les auteurs du texte, un oubli involontaire des élus locaux. Vous m'excuserez par avance de penser que le Sénat n'est pas le lieu pour s'émanciper des garanties propres prévues par nos règles d'urbanisme. Alors que la situation aurait pu être évitée maintes fois. Tant dès 2020 par une intégration du projet d'autoroute au lui ou lors de sa modification simplifiée en 2021. De plus, les auteurs du texte indique que cette PPL est nécessaire, faute d'alternative à ce projet d'autoroute. Je souhaite vous rappeler l'avis du conseil d'orientation des infrastructures dont parlait le Ministre tout à l'heure, qui souligne dans son dernier rapport que ce projet local n'a pas de caractère prioritaire pour le système de transport national et que la desserte du Chablais pourrait être améliorée en renforçant notamment le service ferroviaire du Léman Express train qui a prouvé son efficacité en transportant plus de 50.000 voyageurs par jour. Je terminerai mon propos en soulignant le risque constitutionnel en effet le présent texte avance pour seule justification de cette loi de validation. Le retard dans la conclusion du contrat de concession et donc de réalisation du projet. Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel et pourtant clair, cela ne constitue pas un motif d'intérêt général. En adoptant ce texte nous créerions un fâcheux précédent qui n'honorerait pas le Sénat dans sa conception de ce qu'est la loi et l'intérêt général. Donc pour toutes ces raisons, le groupe écologiste votera contre ce texte qui nous semble fort incongrue. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Bernard buis pour le groupe RDPI. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. À la lecture de la conférence des présidents. Publié le 13 décembre dernier, comme un certain nombres d'entre nous, j'ai été un peu surpris pour ne pas dire désarçonné d'apprendre que le Sénat allait examiner une telle proposition de loi. Peut être pouvait-il s'agir d'une terreur d'impression une publication involontaire de l'ordre du jour du conseil communautaire de Thonon-les-Bains. Non j'ai bien lu, c'est bien à nous parlementaires de régulariser le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bachabélé. La rapporteure que je remercie pour son travail archiver expertiser et documenté nous l'a bien confirmé en commission. Ce texte est inhabituel et concerne un cas spécifique. Dans un contexte d'inflation législative regretté par notre président lors de ses voeux. Nous pourrions considérer que le signal envoyé par l'examen de ce texte n'est pas positif. Alors, mes chers collègues. Quel est le message que nous souhaitons porter en direction des élus locaux à l'heure où la décentralisation doit être confortée par une future loi sur les libertés locales. Et puis, passé l'étonnement. Nous avons cherché à comprendre pourquoi diable passer par le Sénat pour valider un projet d'aménagement local. Le sujet porte sur un projet d'autoroute dans une zone à forte progression démographique, la construction d'un axe constitué de 2 fois 2 voies reliant initialement Annemasse puis ma Chili à Thonon-les-Bains datent des années 1980 ou des premières études ont été lancées. Inscrit au schéma directeur routier national le 1er avril 1992. La motivation politique autour de ce projet était forte de grandes figures nationales se sont alors prononcé pour soutenir ce projet je passe ainsi à Bernard Bosson ou Pierre Mazeaud. Défendu par les milieux économiques du territoire pour favoriser l'attractivité, le tourisme et la mobilité de ses habitants. La quatre 400 fut déclarée d'utilité publique le 6 mai 1995. Mais en raison d'un front uni d'opposants rassemblant mer et riverains, le projet a été rejeté par le Conseil d'État en mars 1997. Après moult rebondissements dont je vous ferai grâce. Le projet est remise sur les rails. 20 ans plus tard et une nouvelle déclaration d'utilité publique et signé en 2019 par le Premier ministre Édouard Philippe. Nous aurions pu espérer le règlement de ce dossier mais la complexité des normes d'urbanisme et l'oubli concernant la mise en compatibilité du PLU lui du Bachabélé en auront décidé autrement. Dans ces conditions, malgré les réserves émises. Ce projet doit aboutir et si cela doit passer de matières exceptionnelle par notre assemblée alors nous soutiendrons cette solution législative qui permettra d'accélérer définitivement le processus car sur le fond, ce projet a du sens. Situé aux portes de l'agglomération genevoise est bordée par le lac Léman le Chablais connaît depuis plus de 50 ans, un dynamisme démographique et économique. Sa population a plus que doublé entre 1960 et 2010 pour atteindre aujourd'hui 130.000 habitants. On regard de la documentation que j'ai pu consulter, nous avons affaire à un territoire particulièrement enclavé qui ne bénéficient d'aucune voix nationale con. Contrairement au reste du département. Élus drômois, plus précisément du Diois région montagneuse qui recouvre le sud du massif du Vercors et le nord de la Drôme provençale, je sais ce que signifie l'enclavement et ses conséquences pour ses habitants. En ce qui concerne les timbres déplacement en effet plus du tiers des actifs du Chablais travaillent en dehors de ce territoire un quart travail en Suisse, plus de 80% de ses actifs utilisent leur véhicule pour aller travailler, ce qui conduit à un engorgement du réseau secondaire et des nuisances résultante. Donc si ce projet soutenu par la population locale et une grande partie des élus du département peut permettent de faciliter les déplacements en direction de pôles d'attractivité comme le Genevois. Alors oui nous devons le soutenir, nous donnerons ainsi un point final à ce serpent de mer pour qu'enfin ce territoire puissent disposer d'un projet structurant facteur d'attractivité qui permettra de désengorger les petits bourgs et de répondre aux besoins d'économie locale. Notre groupe votera donc cette PPL. Socialistes écologistes républicains. la 100 à l'ensemble de mon propos, notre collègue Christian renonce Arazi chef de file de notre groupe sur ce texte. Une fois n'est pas coutume. Je vais exprimer au nom de mon groupe. Des explications de non vote sur cette proposition de loi visant à régulariser, ça a été dit, le pays lui de la communauté de communes du Chablais. C'est un choix rare mais qui s'impose aujourd'hui. Il va sans dire que l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de notre assemblée. De notre assemblée par la droite sénatoriale nous a grandement étonné que comportant un seul article, ces propositions de loi prévoit que les dispositions du décret du 24 décembre 2019 déclarant d'utilité publique le projet de liaison autoroutière entre Massy et Thonon et pourtant mise en comptabilité compatibilité des documents d'urbanisme prévalant sur les dispositions contraires du PLU du bas Chablais approuvé par le conseil communautaire de Thonon agglomération le 25 février 2020. L'objectif de cette manoeuvrent logistique et de permettre la construction du dernier tronçon de 16 kilomètres et demi de l'autoroute A quatre 400 qui désenclave les communes de ce territoire du Chablais. le lui du bas Chablais en cours d'élaboration au moment de l'adoption du décret n'a in fine est pas pris en compte la règle selon la réalisation de cette autoroute est annulé toutes les mises en conformité et la réservation des espaces concernés par les travaux. L'agglomération de Thonon a donc ouvert une demande de modification simplifiée du PLU lui est saisi la mission régionales d'autorité environnementale Auvergne

à générer un nouveau retard parce que Thonon agglomération souhaitent éviter une telle éventualité et de nouveaux blocages des 2 sénateurs LR de son Haute-Savoie ont donc sollicité le Sénat pour régulariser ce projet et forcé la révision de ce pays lui en invoquant un motif d'intérêt général. Mes chers collègues. Prenons un peu de recul sur une telle proposition de loi, nous avons tous dans nos territoires. Des cas particuliers ou difficiles à régler en matière d'urbanisme. On peut imaginer que chacun d'entre nous s'inspire de nos deux collègues. Imaginez un peu l'allure que prendrait alors notre ordre du jour. Plus sérieusement, cette proposition de loi porte atteinte à plusieurs principes constitutionnels et à la crédibilité de notre institution. Le but d'intérêt général évoquée par cette PPL ne présente aucune dimension constitutionnelle mais une volonté clairement affichée d'accélérer un projet en contournant les règles en vigueur relative à l'évaluation environnementale. Elle ne respecte ni l'obligation d'Iggy lance à l'égard des atteintes à l'environnement ni la participation du public induite par la procédure d'évaluation environnementale, ni le droit au recours par ailleurs requérir la procédure législative pour régler une situation strictement local est invraisemblable. Le Sénat ne dispose ne dispose pas du moindre droit d'ingérence dans des projets territoriaux de cet ordre. Comment peut-on valider un tel contournement des procédures habituelles, notamment en termes d'impact environnement et de consultation des citoyens. Comment peut-on demander au sénat chambre des territoires de passer outre les prérogatives des collectivités sur leur document d'urbanisme comment chers collègues. Croyez-vous que cette manoeuvre sera perçu par les élus locaux quelle que soit leur département, n'est-ce pas là une grave atteinte à la crédibilité de notre institution et naturellement soutenu par les deux sénateurs du département de Savoie, pas la majorité. C'est une sénatoriale mais aussi et on doit souligner par le gouvernement. En dépit de ces irrégularités. Il y a donc de fortes chances d'être adopté à l'Assemblée nationale. C'est un exemple supplémentaire du mépris du gouvernement à l'égard du Parlement. On y adopte des lois essentielles sans vote on il régularise des dossiers locaux bientôt le gouvernement de s'passera ne s'embarrassera même plus de nous consulter sur quoi que ce soit voté ce texte créera un dangereux précédent dans la rivière dans la régularisation des projets territoriaux confirmant la négation des prérogatives des communes, le peu de cas qui est fait de l'opinion de nos concitoyens ou des procédures en matière de défense de la vie alors que nous ne pouvons plus nous permettent de les ignorer. Cette manoeuvre ni enfin toute idée de participation collective à l'élaboration de projets qui concernent tournant pourtant en 1er lieu les usagers voter contre ou s'abstenir sur ce texte reviendrait à cautionner la sollicitation du Sénat en la matière et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, vous aurez compris qu'il nous est impossible. Par respect pour notre institution de le faire dans un refus de décrédibiliser le Sénat, le groupe mon groupe, le groupe socialiste, écologiste et républicain ne prendra donc pas part au vote sur cette proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues. Bien évidemment. Et et je ne reviendrai pas, je crois que comme tout un chacun notre groupe, nous nous sommes interrogés effectivement sur l'opportunité de légiférer pour régulariser. Aujourd'hui à travers la proposition de loi de nos collègues haut-savoyard. Le EPA lui d'une communauté de communes, précise le Bachabélé en l'occurrence et donc demain, peut être, ouvrant ainsi la voie à d'autres intercommunalités. Cependant et pour en avoir compris discuter. Ce week-end et puis échanger par, par différents moyens de communication avec un certain nombre d'élus de cette. De ce territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes. je crois que nous avons finalement de débat. Celui d'un projet. Qui est réelle, qui maintenant est posée depuis de nombreuses années. D'une difficulté que vivent au quotidien les habitants et les élus des 10 communes qu'on soit concerné qui effectivement l'engorgement routier quotidien dans ce territoire et donc le projet de la création d'un nouvel axe routier, c'est un, un projet et je veux le dire ici, qui est soutenu par la grande majorité des élus locaux par les habitants, mais qui effectivement a du mal à se concrétiser, comme cela a été relevé. C'était pour autant en bonne voie et je crois que d'ailleurs. Les habitants, il est élu y ont cru avec une déclaration d'utilité publique, une enquête publique purgé de tout de tout J'entends. Également les réserves qui peuvent être émises là aussi sur ce territoire et parfois à l'extérieur sur le besoin de soutenir des modes de transport alternatif notamment des transports en commun. C'est aussi bien évidemment ce que nous suggérons pour offrir la possibilité de voyager autrement que nous ne partons que nous dans les débats en matière de mobilité mais il y a aussi des réalités géographiques. Des réalités de relief qui font que demain. La seule desserte. Ferroviaire qui pourrait être en tout cas d'un point de vue environnemental. La moins polluante, ne peut être la seule réponse et que dans l'urgence, immédiatement tout de suite j'ai envie de dire dès aujourd'hui, il y a également besoin d'améliorer. Le déplacement par voie routière. Pour autant, au même titre que l'on peut considérer que ce n'est pas au Parlement d'intervenir donc sur une compétence pleinement décentralisé. Nous n'avons pas non plus vocation à opposer un projet alternatif, face aux projets retenus choisi démocratiquement, démocratiquement, Il nous est donc à travers cette proposition de loi demander de corriger ce qui s'apparente à une erreur en espérant, comme je l'ai dit que ce type de proposition de loi ne se répète pas. Ce qui est moins sûr aujourd'hui puisque le cas du Bacha Blaise nous semble symptomatique en effet de nombreuses compétences sont régulièrement transférés vers les collectivités de la loi notre avec plus récemment la loi 3DS et si ces transferts permettent parfois de privilégier des politiques publiques. Conçu dans un souci de proximité les moyens qui sont accordés aux collectivités sont malheureusement toujours en dessous de leurs besoins réels, ce qui contribue à aggraver les difficultés qu'elles rencontrent. Et je rajouterai, Monsieur le Ministre, parce que nous disons régulièrement ici au Sénat, les uns et les autres, je crois, sur à peu près tous les bancs, bien évidemment, quand l'on renforce la décentralisation, il y a également besoin d'une véritable déconcentration et donc de fonctionnaires d'État, au service des élus qui les accompagnent et qui les sécurisent dans la prise de décision. Pour autant, cela ne serait pas juste non plus de faire payer ce manque de moyens et cette erreur de mise en conformité qui en découlent, par un retard supplémentaire nous entendons la demande formulée par les élus locaux, l'attente des habitants des 10 communes concernées qui ont entendu parler, je le disais de ce projet depuis des décennies décennies mais demeure relativement mal connecté au reste du département et donc de la région, cet axe routier est une véritable opportunité en matière de développement de mobilité de réduction de la pollution sonore qu'ils connaissent au quotidien. nous nous opposerons pas au passage de ce texte comme nous ne l'encourageront pas non plus et donc, notre groupe s'abstiendra. En l'état, Monsieur le président. Monsieur le Ministre, madame le rapporteur. Mes chers collègues. Cet après-midi c'est l'avenir du Chablais qui nous réunit. Le Chablais. C'est l'une des 6 provinces de la Savoie historique. Situé sur la rive sud du Léman entre lac et montagne. Ils représentent l'essentiel du territoire de l'arrondissement de Thonon-les-Bains. Le Chablais. C'est un territoire dynamique de plus de 100.000 habitants. Qui est à la fois touristiques, agricoles et industriels. Ne buvez-vous pas de l'eau d'Évian ou de Thonon régulièrement. La géographie apparemment très favorable de ce territoire lui crée cependant des contraintes importantes en terme de desserte par les infrastructures, notamment routières. Ainsi, le quotidien des Chablaisiens ce sont les bouchons routiers quand ils vont vers Genève Annecy où la vallée de l'Arve ou qu'ils en reviennent. L'idée de la création d'une liaison routière et autoroutière de entre l'A40 et Thonon-les-Bains n'est pas nouvelle, elle a une quarantaine d'années. Alors que nous nous approchons de la mise en concession, après que tous les États voulue par la loi ont été franchi avec succès le projet est confronté à un écueil semble-t-il insurmontable qui risque de retarder durablement, ce projet qui n'a que trop traîné. Il est vrai que l'idée de régler la situation par la loi et surprenante inédites presque innovantes. Se fondant sur la hiérarchie des normes, selon laquelle une loi prévaut sur un décret qui lui-même prévaut sur un arrêté ministériel ou sur les actes des collectivités territoriales ainsi faudrait-il passer par la loi pour rectifier le document graphique du lui de l'ex-Communauté de communes du bas Chablais Alors je mets mes interrogations de côté. Et je vais vous faire confiance madame la rapporteure. Je vais faire confiance aux services. De l'État et à leur analyse Monsieur le Ministre, en apportant mon suffrage à l'adoption de cette proposition de loi. Mais mes chers collègues si la liaison autoroutière mérite absolument d'être soutenu pour être réalisé, seule elle ne changera rien et risque bien d'être saturé. Dès son ouverture dans quelques années. En effet le désenclavement du Chablais sera donc multimodal ou ne sera pas. Et la vraie préservation de notre environnement passe bel et bien par là. Monsieur le Ministre, le président de la République a annoncé sa volonté de développer des réseaux RER dans 10 métropoles dans l'agglomération franco-valdo-genevoise. Nous avons déjà le onzième c'est le Léman Express. Il nous faut plus de trains. Et aussi des trains qui vont plus vite, il faut aussi des parkings relais bien positionné qui permettent le transfert de l'automobile vers le train. Je formule le voeu que notre étoile ferroviaire autour de Genève puisse bénéficier de travaux permettant au train de reprendre toute sa place à l'ouest du Chablais entre Genève et et Évian via Annemasse et tonneau mais aussi à l'Est avec la réalisation du RER Sud-Léman qui permettrait le bouclage du lac avec la remise en service de la voie ferrée dite du Tonkin. Mais il n'y a pas que la route. L'autoroute et le train il y a aussi le bateau, en effet, la desserte des grandes villes du littoral du Léman de la Rive-Nord comme de la rive sud doit être développé considérablement. Tout comme doivent être développées. Les transports publics du quotidien autour de la ligne de bus à haut niveau de service corollaire lui aussi indispensable du désenclavement routier et autoroutier du Chablais. Enfin je me ferais taper sur les doigts si j'oubliais le vélo. Avec la ViaRhôna et les mobilités douces qui se prête très bien à la topographie comme au climat tempéré des rives du Léman. Alors pour tout cela. Nous avons besoin d'un chef d'orchestre et d'un ensemblier pour mettre en oeuvre cette vision stratégique pour fédérer les initiatives des collectivités territoriales et des élus locaux poursuivre aussi les engagements politiques pris par les uns et les autres souvent à grands coups de clairon médiatique. J'en appelle à vous Monsieur le Ministre, pour que l'État joue complètement son rôle poursuivent ces différents projets et s'assurer qu'ils sont bien menée de conserve je j'espère que vous saisirez cette occasion pour qu'un qu'un désenclavement durable soit mis en oeuvre pour le Chablais et le nord de la Haute-Savoie. Nous le devons au Chablais. Nous le devons aux Chablaisiens pour le rap porter une accessibilité digne de ce territoire. Je vous remercie. Damien. La parole est maintenant à monsieur Henri Cabanel pour le groupe. RDS. Et 4 minutes. Je remplace au pied levé mon collègue Christian Billac, auteur de cette. Discussion générale qui n'a pu se déplacer à Paris la présente, proposition de loi propose de procéder par voie législative au déblocage du projet, dit-elle. M.t. de liaison autoroutière entre ma Chili et Thonon-les-Bains en Haute Savoie projet déclaré d'utilité publique en décembre 2019 dans le tracé n'apparaît pas au sein du pays lui du bas Chablais. En cause, une complexité procès du rial due à une modification du PLU Ueli concomitante à l'évolution du périmètre de la collectivité et à la procédure liée à la DUP. L'enquête le public dans le cadre de la DUP a été menée en 2018 et porte sur des opérations de réalisation d'une voie nouvelle à 2 fois 2 voies à caractéristiques autoroutières.

La suppression de, de passage à niveau sur la route départementale centre ancien la requalification de la route départementale 903, dans les traverses de du à Chablais et Périgny bien que cette dernière ne relève pas d'une d'IUP, voici en quelques mots ses conclusions afin de ne pas retarder davantage la réalisation du projet, on propose de recourir à la loi plutôt qu'à une procédure ordinaire de modification simplifiée du PLU lui que la communauté d'agglomération avait tenté de mener avant que la mission régionales d'autorité environnementale d'Auvergne Rhône Alpes exige en 2021 une évaluation environnementale du projet. En effet le fuseau autoroutier n'a pas été intégré lors de l'élaboration du pays le lui alors que l'enquête publique sur la mise en cause hein compatibilité des documents d'urbanisme avait eu lieu dès 2018. Mes chers collègues permettez-moi de faire 2 remarques. Première remarque de principe pour commencer. Si le législateur doit intervenir à chaque fois qu'un palu, un palu oui Stradella ou tout autre projet d'intérêt local ou régional connaîtra des difficultés de mise en oeuvre. Il conviendra désormais que le Parlement siège de 52 semaines auparavant. 2ème remarque est inspiré de mon expérience d'élue de terrain. J'ai bien noté que ce projet de liaison autoroutière. S'inscrivait dans une démarche de transition écologique est exemplaire d'un point de vue de son insertion induire le mental toutefois pour avoir connu le même type de projet dans mon département de l'Hérault, alors même qu'il y ait aucune incompatibilité entre les textes existants. Le projet a dû faire face à une contestation juridique du dossier par des associations environnementales, laquelle Cossette. alors retardé le projet de plus de 10 ans. Loin de moi l'idée de souhaiter le même sort au projet elle T si le lui devait faire l'objet d'un nouveau recours à liaison a raison pardon de l'absence d'évaluation environnementale intégral le projet. Mais il y a fort à parier que sur ce projet on redécouvre tout un tas d'espèces rares inconnues souvent du grand public. Vous l'aurez compris. Mon groupe par respect pour notre rôle de législateur est exclusivement sur un problème de forme ne participera pas au vote de ce texte pour qui être utile n'est pas moyen congrue cet hémicycle Alain Alain place de motif impérieux d'intérêt général. Nous ne pouvons soutenir cette loi de validation. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole maintenant Madame Sylviane Noël. Pour les républicains et pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues, il me revient le plaisir et l'honneur de clôturer quasiment cette discussion générale relatifs à la proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui dont je suis coauteur avec six Cyril elle va. Je tiens tout d'abord à remercier vivement notre rapporteur Martine Berthet pour la qualité de son travail, le sérieux et la rigueur avec lesquels elle a abordé cette proposition de loi. Avant d'entrer dans le vif du sujet. Il me semble important en préambule de vous présenter le contexte particulier dans lequel s'inscrit cette demande de validation législative. De quel territoire parlons-nous du Chablais, la région la plus septentrionale des Alpes françaises. Un secteur de Haute-Savoie particulièrement dynamique d'un point de vue démographique tenant agglomération a connu une croissance de sa population de 16 et demi Regroupant des lieux touristiques de renommée internationale comme Thonon Évian Morzine-Avoriaz Chatel et bien d'autres stations avec 207.000 lits touristiques. Des activités économiques de 1er plan notamment la plus importante usine d'embouteillage de France et parmi les 3 plus grandes du monde, avec les eaux minérales d'Évian. Qui compte 1200 salariés, 6 millions de bouteilles qui quittent chaque jour ce site dont une grande partie. Via le réseau ferroviaire et une autre partie, par la route. C'est enfin un secteur, caractérisé par des échanges internationaux de premier ordre le Chablais étant à l'interconnexion avec Genève, le canton de Vaud et le Valais. Sur le plan politique, ce territoire fut l'un des derniers de France à être couvert par l'intercommunalité. Vous allez comprendre mes chers collègues, que cette précision et la chronologie qui l'entoure a toute son importance dans l'évocation de ce texte et des raisons qui ont pu conduire à cette incohérence de documents d'urbanisme qui nous occupe aujourd'hui. Il s'agit en effet du dernier territoire de France à être couvert en totalité par un EPCI à fiscalité propre une intercommunalité né sous la contrainte au prix de nombreux débats parfois violents CDCI. La ville de Thonon-les-Bains restera ainsi isolé de tout rattachement intercommunal jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle naîtra Thonon agglomération née du regroupement des communautés de communes du Bacha bled et collines du Léman et de la ville de Thonon. Avant l'amendement de cette communauté d'agglomération la communauté de communes du bas Chablais concernées par le tracé de cette autoroute. Ah le 17 décembre 2015, presqu'île élaboration du PL lui sur l'intégralité de ce territoire en 2017, cette communauté de communes disparaît au profit de Thonon. Qui reprend alors la main sur cette procédure le 22 octobre 2019, le conseil communautaire de Thonon agglo arrête le projet du P. lui du bas Chablais avant de l'approuver définitivement le 25 février 2020. Et dans certains dans cet intervalle, 2 mois avant le 24 décembre 2019 et signer le décret du Premier ministre, déclarant d'utilité publique le projet de nouvelle voie entre. Thonon décret portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes concernées. Cette chronologie révèle ainsi parfaitement que l'absence du tracé de cette autoroute dans le PLU du bas Chablais est incontestablement lié à un défaut de vigilance de tous les services, dans un contexte d'enchevêtrement de procédures complexes menée concomitamment et de construction d'intercommunalité. Or il s'agit pourtant d'une infrastructure absolument vital pour désenclaver le territoire chablaisien, un des derniers barreau autoroutier manquant du département. Il convient par ailleurs de souligner que des 2 fois 2 voies existent déjà aux extrémités du projet autoroutier. En amont, existe déjà, la deux fois deux fois machine chasseurs qui sera complétée très prochainement par une liaison à 40 chasseurs porté par le département de la Haute-Savoie et en aval, se trouve le contournement de Thonon également en 2 fois 2 voies et donc au milieu se trouve ce goulot d'étranglement, source de bouchons interminables aux heures de pointe c'est 16 qui ne sont pas ni au gabarit et qui supporte un trafic routier très soutenue qui traverse plusieurs communes certaines rural jusqu'à 2022, 1000 véhicules/jour enregistrée pour certaines d'entre elles. Cette situation ainsi amener l'État à prendre la décision de mettre en 2 fois 2 voies ce tronçon sous-concession autoroutière. Il est ainsi inconcevable de laisser persister un tel trafic sur le réseau routier secondaire avec tous les risques que cela comporte. L'actualité de notre département nous l'a tristement rappelé il y a quelques jours seulement, avec l'explosion d'un camion-citerne circulant en zone agglomérée engendrant de blessés graves et des dégâts matériels très importants. Il en va donc du bon sens de terminer ce projet porté par l'État dont, je le rappelle, l'ensemble des procédures ont été validés et l'ensemble des recours purgés, le Conseil d'État ayant confirmé il y a tout juste une année le rejoint le rejet des recours des opposants, la procédure de validation législative est parfaitement encadré par le législateur et elle est incontestablement adapté à ce type de situation visant à réparer une pure erreur matérielle de procédure, comme c'est le cas en l'espèce. Notons qu'il y a une vingtaine de procédures de ce type examiné en moyenne chaque année par le Parlement français sur des cas spécifiques, il nous est ainsi arrivé de légiférer sur des questions très particulière concernant la clairette de Die les règles spécifiques pour l'aménagement des Jeux olympiques et du Grand Paris ou encore des délais supplémentaires accordés pour l'élaboration des PLU ils métropolitain et parisien. Mes chers collègues. Bon nombre d'entre nous avons été élus locaux avant d'être sénateur. Nous connaissons les lourdeurs administratives immense liés à ces procédures d'. Élaboration d'urbanisme a fortiori à des stades intercommunaux et à la conduite de ce type d'infrastructures structurantes. Un projet attendu depuis près de 30 ans est fortement soutenu par l'immense majorité des collectivités locales, des entreprises, des citoyens qui souffrent de cet enclavement et des difficultés de circulation qui s'aggrave avec le temps. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur ou d'un oubli qui ne peut en aucun cas remettre en cause le bien-fondé le sérieux d'un projet porté par une dizaine d'années de concertation d'études de procédure parfaitement mené à bien et tout à fait transparente l'ensemble des taux des documents de Thonon agglomération prenant bien en compte dans dans leurs équilibre réorientation. Le projet de liaison autoroutière. Les élus de nos territoires et les citoyens déplore chaque jour notre complexité administrative source d'erreurs et de contentieux dans sa grande sagesse, le législateur a permis par le biais de ses validation législative une résolution rapide et efficace des erreurs et omissions dont nous pouvons tous être responsables, un jour ou l'autre ne nous privons pas de cette situation. Et servons-nous au contraire de cet exemple pour tenter de simplifier davantage ce type de démarche, source de contentieux, la chambre des territoires que nous sommes doit démontrer dans son pragmatisme à permettre une résolution rapide de ce type de problématique, les élus locaux n'attendent rien de moins que cela de la part de ceux qui ont le privilège et l'honneur de les représenter dans cet hémicycle. Je vous invite donc massivement à voter en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci cher collègue et. La discussion. Général va être maintenant en effet Close après l'intervention du président Maluret.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le Bachabélé était un territoire particulièrement prospère et attractif qui voit sa population augmenter considérablement. Située entre la lac vallées et montagnes. Ses habitants bénéficient de la beauté des rives du lac Léman. Sa position géographique, on fait également un lieu de passage stratégique pour les travailleurs transfrontaliers. Toujours plus nombreux à faire chaque jour le trajet entre la France et la. Face à l'augmentation rapide des flux routiers et la tension sur la lignes ferroviaire et c'est lui locaux tirent la sonnette d'alarme. Depuis des années, défendu par les autorités publiques souhaitée par les élus locaux et surtout attendu par les habitants. La construction d'une liaison autoroutière entre les villes de Massy et de Thonon-les-Bains est annoncée depuis plusieurs années. Une large concertation publique a été engagée et les recours déposé au Conseil d'État, en opposition au projet ont été examinés. Le projet en est sorti renforcé et conforté dans son caractère d'intérêt général. La construction d'une liaison 2 fois 2 voies répondrait efficacement à la congestion croissante des axes de circulation actuel. Après diverses péripéties. Ce projet a été déclaré d'utilité publique en 2019 comme cela a été rappelé précédemment. Le décret en question emporte mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes concernées. Pourtant à la complexité administrative se sont ajoutés des aléas de de calendrier empêchant le projet de liaison autoroutière de figurer dans le pays lui de la communauté de communes. Nous avons donc été saisie d'une requête à visé dérogatoire, ce qui est très habile très inhabituelle pour un cas particulier mais ce projet est important pour le Bachabélé. Au vu des difficultés présentes et des perspectives démographiques futures. Nous pouvons dans ce cas, prendre en considération les spécificités des territoires et adapter le droit aux situations locales. Aujourd'hui, nous soutenons donc ce projet d'intérêt général qui répond aux grandes difficultés de circulation et d'enclavement dont témoignent les habitants du Bachabélé. Parmi les différentes options. Le recours à la loi paraît être la solution la moins imparfaite pour répondre aux impératifs de calendrier. L'adoption de ce texte mettra un terme à cette situation de paralysie administrative. Et de joute procédurale entre les parties prenantes au nom du groupe des Indépendants j'accueille donc favorablement cette proposition de loi, tout en soulignant que le recours à la loi pour régulariser un pays lui doit rester exceptionnel. Je vous remercie. Merci monsieur le président, mes chers collègues. Comme indiqué tout à l'heure dans la discussion générale, cette proposition de loi soulève de graves difficultés sur le plan constitutionnel. Le but, invoqué par ce texte, c'est une volonté d'accélérer un projet en s'émancipant des règles en vigueur relative à l'évaluation environnementale, à savoir la méconnaissance de l'obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement. La méconnaissance du principe de participation du public induit par la procédure d'évaluation environnementale et la méconnaissance du droit au recours. À l'heure de l'urgence climatique qui n'aura échappé à personne et du nécessaire respect de l'environnement. Il n'est pas acceptable qu'un texte viennent s'affranchir de l'ensemble des garanties propres à l'évaluation environnementale. Cette loi pose question sur la forme comme sur le fond. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. Accélérer la construction du autoroute en ce début 2023, nous semble complètement anachronique et est une négation à l'urgence climatique. Il est urgent. Il faut poser les choses, il y a des procédures. Prenons le temps des projets qui était sans doute valide. Il y a quelques années s'avéreront complètement néfaste demain. Merci cher collègue. Qui est l'avis de la commission, madame la. Alors Alors l'avis de la commission est bien sûr défavorable. À la suppression de cet article, comme je l'ai dit lors de la discussion générale. Ce texte poursuit un objectif que nous pouvons tous partager. Il s'agit de permettre à un projet d'intérêt général déjà validé déjà validé soutenu par les collectivités territoriales et la majorité de la population de se poursuivre. Il n'est aucunement question d'aller à l'encontre des compétences des collectivités territoriales qui sont en attente de ce texte et ont déjà consenti en 2019 à la mise en compatibilité de leurs documents d'urbanisme. Au contraire, elle souhaite pouvoir faire évoluer leurs documents dans les conditions qui sont d'ordinaire permise en cas de déclaration d'utilité publique. Il n'est pas non plus question de réduire l'information du public. Je rappelle que le projet a fait l'objet d'une concertation publique sous l'égide d'un garant désigné par la commission nationale du débat public, de l'ensemble des consultations obligatoires chambre d'agriculture commune et d'une enquête publique en bonne et due forme. Il s'agit plutôt d'éviter au projet de repasser inutilement par l'ensemble de ces étapes. Alors qu'il n'a pas évolué d'un iota. Avis donc défavorable. Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre, de l'avis du gouvernement. Oui même avis monsieur le président sur le texte, le gouvernement a donné un avis de sagesse. Le Sénat va se prononcer dans quelques instants. Donc il me semble préférable que la vie de votre assemblée s'exprime à cette occasion et sur l'ensemble du texte. Je rappelle notre avis de sagesse défavorable pour cet amendement pour laisser la place au vote. Donc nous allons voter la commission m'a saisi d'une demande de scrutin public. Va être annoncé. Sur l'amendement. Pas sur l'article ensuite. Nous votons sur l'amendement de suppression avec avis défavorable de la commission et vite, ça laisse du gouvernement.

votants 265 exprimés, 264 pour 12 contre 252. L'amendement n'est pas adopté, je mets aux voix. L'article.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Je suis saisi d'un amendement numéro 2 qui porte sur le titre de la proposition de loi. Ces messieurs salement qu'il défend. Merci monsieur le président. Et bien sûr cette loi qui est franchement atypique au moins essayons d'être clair sur un point sur le titre. Alors je vais vous proposer de le compléter. Donc à 20 afin d'être précis dans l'intitulé du projet de loi et pour bien définir les moyens qu'il se donne pour atteindre l'objectif. Nous proposons de préciser que cette proposition de loi vise à contourner le droit de l'urbanisme dans le but de régulariser le lui de la communauté de communes du bas Chablais. Au moins ça aura le mérite de dire ce que ça veut faire voilà, je vous invite donc tout ça a changé ce titre je vous remercie de cette confiance. Beaucoup chers collègue David la commission s'il vous plaît madame là. Alors bien sûr l'avis de la commission est défavorable. La proposition de modification de l'intitulé du texte ne reflète ni son contenu ni son intention. Il n'y a pas de contournement du droit car il n'y a pas de volonté de faire échec aux compétences des collectivités, pas de volonté de supprimer des garanties de participation. L'ensemble de ces étapes ont déjà été ah a déjà été accompli avec succès au cours des dernières années, il n'y a pas de recul et pas d'évolution a posteriori du projet. c'est loin d'ailleurs d'être là pour la première fois que le la loi par dont traite de cas spécifique. Pour lever des obstacles ou proposer des simplifications. Il s'agit d'une mesure dérogatoire qui élève au niveau législatif, la déclaration d'utilité publique portant mise en compatibilité cette dérogation se justifie par l'absence d'alternative réaliste et l'intérêt général du projet. le vois cet amendement à monsieur dessus demande à exprimé son humble expliquer son vote. Oui, moi je pense que le l'amendement reflète bien le l'intention du du texte. Initial et je pense qu'on est en train de créer, ça a été répété par certains des des des intervenants. On est en train de créer un précédent assez dangereux. d'intervenir sur un tout un tas de documents qui ne serait pas conforme avec la loi et puis en plus j'ai entendu un des coauteurs de du texte nous expliquait que si on ne venait pas du territoire concerné. On n'avait pas non plus à se prononcer alors qu'il vient lui-même devant la représentation nationale nous proposer un texte, il faudrait désormais avaler tout ce qu'on nous raconte. Sans avoir à s'exprimer. Moi je suis assez inquiet aussi de ce qui a été prononcée dans cet hémicycle, puisque quand on nous explique une autoroute sera vertueuse pour l'environnement. Je suis quand même assez perplexe. La compensation, on sait que c'est devenu une vaste fumisterie. Mais j'ai bien compris que ça faisait partie du pilier qui nous rendrait vertueuse. Ce ce ruban de bitume. Mais un projet qui a été imaginé dans les années 80. Au moment où le président de la République nous dit qu'on ne remplit pas nos objectifs qu'on est largement en dessous, qu'il va falloir doubler les efforts. On a un ministre des transports qui lui veut faire du en même temps développer les infrastructures ferroviaires, les infrastructures routières tout ça tout en même temps. Tout ça n'est pas sérieux tout ça extrêmement inquiétant pour la suite pour notre. Pour notre avenir pour le climat. Moi je suis. Très inquiet, on est dans une, dans une forme de fuite en avant dans les projets routiers. Toujours plus, c'est très inquiétant, c'est qu'il y a des milliards de projets routiers encore dans les dans les cartons. Je des milliards d'euros à investir dans les projets routiers. Dans dans dans Il va falloir arrêter ça assez vite et se concentrer sur le report modal apporter des solutions réelles aux vrais problèmes réels des territoires mais qui ne passeront plus par ce mode de déplacement. C'est pour ça que nous voterons contre aussi ce texte, à la fin, merci. Madame Cukierman explique son vote. Très rapide, monsieur le président, monsieur Miss mes chers collègues. Moi je crois que nous devons éviter tout écueil. Sur sur ce texte là. Nous ne pouvons pas non plus nous dire autant que de besoin, qu'il faut décentraliser renforcer le pouvoir des élus locaux et compte il y a des projets. Forcément les stigmatiser et je crois que et. La question n'est pas de savoir de quel territoire nous sommes pas parce que de partout dans le territoire national, la question elle se pose. Oui moi je fais partie de semi-mais défend défendant le train mais nous savons aussi d'un point de vue pragmatique que le train ne pourra pas et ne passera pas partout. Et qu'aujourd'hui on a une vraie réelle problématique dans ce territoire là qui est d'abord l'urgence à désengorger la traversée d'un certain nombre de communes au quotidien. Et parallèlement et en plus, on le sait très bien dans cette partie là de de de de de la Haute-Savoie. Les différents modes de transport de transport se développe et donc travaillent en complémentarité. Donc, je crois, faisons vraiment attention et je le redis tout de même je crois faisons aussi parfois. Attention à ne pas donner le flanc à la critique d'un travail parlementaire qui ne serait pas sérieux moi je respecte, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette proposition de loi en revanche. Le sens initial de la proposition n'est pas de déroger au code de l'urbanisme, il c'est d'apporter une solution aux habitants d'un territoire. explications de vote sur le titre du texte monsieur seulement a demandé la parole. Oui, excusez-moi monsieur le président, c'est. C'est pas franchement sur le titre effectivement c'est plutôt je je le ferais tout à l'heure dans explication de vote à ce moment-là sur l'ensemble de la loi. Et merci madame la présidente, vous souhaitez intervenir sur le titre. Très rapidement, monsieur le président. Merci de me donner la parole, je voudrais dire à monsieur dessus que je comprends qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette proposition de loi qui une fois encore, n'est pas sur l'intérêt du projet mais sur une une. Une procédure mal. Mal conçus ou mal réalisé au regard de la complexité du droit de l'urbanisme. En revanche, je voudrais dire à monsieur dessus quand il nous dit qu'on veut faire ici avaler des couleuvres ou des mensonges. Je voudrais dire à monsieur dessus de respecter le travail de Madame la rapporteure madame la rapporteure. On essaie de vous faire avaler rien du tout, elle a travaillé, elle a fait les auditions avec nos administrateurs, et elle a fait un travail sérieux, donc je vous demanderai par respect du rapporteur de vous excuser sur ce point. les questions de d'ordre personnel, se déroule en fin de séance. Donc maintenant je consulte le Sénat sur ce titre. Quels sont ceux qui sont pour l'amendement qui modifie le titre. Quels sont ceux qui sont contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je dois mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi bien que Henry était tous soit adoptée et donc je recueille les demandes d'explications de vote sur le texte. Monsieur dessus monsieur le d'abord. C'est juste pour répondre. À la présidente de de la commission je je veux bien m'excuser si ça a été mal compris, ce n'était pas la rapporteure que je que je visais c'était plutôt les propos du co-, coauteur du texte qui nous expliquait que ne faisant pas partie du territoire, on devrait. Comprendre et avaler tout ce qu'on nous racontait mais je suis désolé c'est pas le cas. Moins il y a deux de mise en cause personnelle, le mieux on se porte quand même hein. Monsieur Salmon, veut s'expliquer le vote de son groupe sur la proposition de loi. Sur le fond de l'affaire. Il s'agit pas de stigmatiser quelques territoires que ce soit et des positions de certains élus. Simplement il faut s'. Il faut regarder les choses où elles sont aujourd'hui. Les alertes se multiplient. L'urgence est là. Eh bien je pense que dans ces temps d'urgence, il faut savoir prendre le temps de réanalyser des projets, même s'ils ont été validés. Il y a un certain temps. Aujourd'hui on doit regarder ça avec d'autres yeux. Je pense que sur de nombreux projets autoroutiers c'est un moratoire qu'il faut faire, il faut vraiment se pose des questions. On sait bien ce qu'on sait bien ce que ça donne chaque fois que l'on ouvre une une nouvelle route. C'est un appel d'air, c'est davantage de véhicules, il ne faut pas se voiler la face, et c'est pas parce qu'on mettra des véhicules électriques dessus que ça va régler tous les problèmes. Simplement on déplace on déplace les pollutions et on continue d'en créer. Et donc notre planète n'en peut plus et je pense que ce genre de projet n'a plus rien à faire en 2023. Je ne vois pas d'autres demandes d'explications de vote. Je vais donc mettre aux voix, la proposition de loi visant à régulariser le P. lui. De la communauté de communes du bas Chablais et nous avons une demande de scrutin public émanant du groupe j'ai. Du groupe Il va être procédé au scrutin public dans les conditions de l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Que personne ne nous demande de voter. Le scrutin est clos. Résultat, nous sommes 265 votants 246 exprimé pour la proposition de loi 234 contre 12. Elle était adoptée. Je suspends la séance quelques instants pour permettre aux autres orateurs de s'installer pour l'examen du projet. Du du projet. Un point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

en est reprise lors du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants. Monsieur le président. Présentée par Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier sur la demande du groupe les républicains. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Albéric de Montgolfier, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes.

Monsieur le président. Merci Monsieur le Ministre, mes chers collègues, monsieur le rapporteur général monsieur à la commission des finances. Nous allons maintenant examiner une proposition de loi qui n'a rien à voir avec AP lui intercommunal. Mais c'est une proposition de loi qui est portée par le rapporteur général Jean-François ici par moi même et qui je le précise est le résultat d'un long processus que nous avons engagé dès 2020 sur le thème de la protection des épargnants. Ce marathon si je puis dire, vu le nombre d'auditions. Je l'ai d'abord engagé en tant que rapporteur général dans un contexte qui était à l'époque fort différent d'aujourd'hui, puisque c'était un contexte de taux bas

La proposition de loi que nous avons à faut soit ils sont et moi-même déposé en mars dernier, se situe dans le prolongement Direct de notre rapport d'information publié au mois d'octobre 2021 et qui avait donné lieu à 17 recommandations de niveau normatif varier les 12 articles initiaux de la proposition de loi sont directement tirées des recommandations de nature législative de ce rapport. Au terme d'une quinzaine d'auditions. Ils ont été modifiées améliorées et complétées au stade de l'examen en commission par 20 amendements, dont huit portant additionnel. Je salue ici monsieur le ministre et les échanges constructifs que nous avons pu avoir avec bien sûr vos services mais également avec le ministère. Les autorités de supervision, que ce soit l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les constats que nous adressions il y a un an et demi dans notre rapport n'ont pas changé. Le marché de l'épargne est certes dynamique mais il se distingue également par la prédominance du marché historique de la banque assurance, ce qui nuit à la concurrence et par des frais qui sont plus élevés que la moyenne européenne. Ces constats sont d'autant plus d'actualité que vous le savez, l'inflation a atteint 5,2% en moyenne en 2022. Et cela devient un facteur supplémentaire d'érosion de l'épargne des Français.

regroupés dans 4 chapitres. Le 1er porte sur l'encadrement plus strict de certaines catégories de commission avec même la suppression des commissions de mouvement spécificité française. Le 2ème chapitre entend répondre aux épargnants. Leur permettant de faire un choix plus éclairé dans la sélection de leurs produits. Le 3ème chapitre comprend des dispositions destinées à lever les contraintes sur les produits d'épargne et à stimuler la concurrence, tandis que le dernier chapitre regroupe les dispositifs de nature à permettre de mieux encadrer le marché d'arrêter les acteurs du marché de l'épargne. Je concentrerai mon intervention sur le 1er et 4ème chapitre laissant rapporteur général le soin de présenter les autres chapitres. D'abord sur les frais, je le rappelais, alors même que la part de la performance capté par les frais et de plus en plus élevés à long terme, au détriment des épargnants. Les articles hein et de de la proposition de loi viennent soutenir un meilleur encadrement de ces frais. L'article 1er interdit les commissions de mouvement. Les épargnants doivent en effet s'acquitter en plus des frais de transaction de ces commissions et subissent à cet égard une double charge et ces commissions porte également un risque inhérent de conflits d'intérêts. Les gestionnaires peuvent être un effet inciter à faire tourner plus les portefeuilles. À faire plus d'achat ventes sans que cela se fasse uniquement au bénéfice de l'épargnant. Elles sont une spécificité veulent voir une âcre cuité française et nous nous félicitons que depuis de travaux l'Autorité des marchés financiers. L'AMF et modifié son règlement général pour les interdire à partir du 1er janvier 2026, depuis le dépôt d'autres textes. Cela a sans doute contribué de manière a servi de levier de négociation supplémentaires et nous avons donc obtenu gain de cause sur un sujet majeur c'est la raison pour laquelle nous vous proposons tout à l'heure d'entériner cette modification du règlement général de l'AMF en supprimant l'article hein je pense que nous avons en effet obtenu gain de cause, l'article 2 propose quant à lui d'introduire une définition de l'arbitrage et du mandat d'arbitrage dans le code des assurances. Pourquoi cet article. D'apparence si technique il y a cela de JT fication simple il faut opérer un rapprochement réglementaire entre les produits assurantiels et les produits financiers d'une part et il faut par ailleurs mettre fin à un certain nombre de pratiques hétérogènes. Après le passage en commission, il est désormais maintenant pleinement conforme au droit européen. Mais aussi plus tranchant puisque je lisais interdit les communistes perception de commission du mouvement par les mandataires j'aborde maintenant le chapitre IV et les autres étant abordé par Jean-François Bisson le chapitre IV qui compliquera les dispositions visant à mieux encadrer

Convaincus par les auditions que nous avons menée, que l'orgasme ne disposait pas des moyens nécessaires d'assurer sa mission. Il n'en demeure pas moins que le modèle actuel qui est basé sur un contrôle par les situation professionnelle et qui s'inspire de l'armée régulation qui est mis en place pour les conseillers notamment en épargne financier n'est pas optimale et suscite un certain nombre d'interrogations sur un risque de complaisance par exemple. J'avais évoqué ces risques devant vous. Lors de l'examen de la proposition de loi réforme relative à la réforme du courtage en assurance dont j'étais rapporteur et Jimmy tiens pour que ce modèle de co-régulation fonctionne il faut encore que les associations professionnelles elles-mêmes soient contrôlé et c'est le rôle de l'autorité de contrôle prudentiel et drôle, solution la CPR qui jusqu'à maintenant faisait très peu de contrôles. Les travaux que nous avons menée sur l'article 11 nous ont permis d'aborder d'arriver je pense à un compromis satisfaisant sur un sujet majeur, celui de l'encadrement des investissements défiscalisés dans le secteur locatif, alors vous savez en France on paye beaucoup d'impôts sans doute mais on a égal, on aime également beaucoup les réductions d'impôts parfois un peu trop et tous les ministres du Logement nous ont expliqué qu'ils allaient résoudre la question de la crise du logement en attachant leur nom à un dispositif fiscal alors là tout le Pinel, mais tous les tous les ministres de droite de gauche le Perissol et cetera ont inventé le boulevard le sens si on peut les citer. Ils nous ont expliqué que c'était des fugitifs, qui allait permettre définitivement de résoudre la crise du logement et il est forcé de constater que un certain nombre d'intermédiaires vendent ces produits d'épargne. Immobilière défiscalisé en oubliant parfois un peu de rappeler aux investisseurs, aux épargnants, le risque que cela comporte. On vous vend la réduction d'impôt, quand vous regardez les publicités vous voyez payer moins d'impôts. de de de de dire que c'est un investissement dans le terme qu'il y a des charges de remboursement on vous dit, rendement garanti. On vous dit risques locatifs zéro tout ça évidemment n'existe pas et aujourd'hui ce secteur n'est pas encadrée et vous avez sans doute voyez vu sur Internet des publicités pour investir dans des villes, parfois dans des quartiers

les investisseurs ne sont pas suffisamment averti des risques et parfois des offres frauduleuses qui minore ou qui font abstraction des des risques encourus. Les vendeurs se concentre en effet sur l'Avantage fiscal sans mentionner le risque pour le Patrimoine, il risque fiscal et je crois que nous pourrions Monsieur le Ministre, ne plus laisser ces pratiques perdurer. Nous proposons donc titre de cet article 11. Un encadrement plus strict de ces offres du travail des intermédiaires avec des exigences en matière de publicité qui serait renforcée pour indiquer l'ensemble des risques investissements avec une notice d'information qui devra être obligatoirement remis à la épargnants et avec un manquement surtout qui devrait qui pourrait être sanctionné par les agents de la DGCCRF de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la réflexion des fraudes qui pourront infliger des amendes administratives. Alors nous souhaitons plus loin nous avons examiné avec l'AMF la possibilité d'aller vers un contrôle plus accrue, il est en effet paradoxal. Je rappelais le montant des produits de des plans. En matière des ses 44.000 euros en matière d'épargne et sur l'investissement immobilier en évidemment sur des sommes qui sont beaucoup plus importantes et paradoxalement il y a moins de contrôles et donc le nous aiderons MatMut autrement de rapport pour évaluer les moyens nécessaires à la mise en place d'un contrôle systématique des offres de publicité des documents contractuels qui constituera une première étape, je l'espère vers un contrôle a priori de ces offres. je crois une tâche immense mieux réguler ce secteur en tous les cas, dans le sens de la protection des épargnants et c'est également le sens de l'article 12 qui vise à s'assurer que les acteurs du financement participatif sont bien soumis à des obligations des curative au titre de lutte contre le blanchiment. Voilà, je laisse à Jean-François Husson, puisque mon temps est écoulé le soin de vous présenter les autres aspects j'espère. Mes chers collègues que vous souscriraient assez de de loi qui vise à mieux protéger les épargnants dans un contexte de hausse des taux et et dans un contexte en tous les cas de recherche de rendements, c'est aussi le moyen de mieux protéger les Français, notamment en diminuant les frais je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant. Au rapporteur de la commission des finances Jean-François Husson qui a également 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Prenant à l'instant le relais de mon collègue Albéric de Montgolfier permettez-moi également et d'abord de saluer la qualité de nos échanges avec le ministère et les autorités de supervision, ainsi que l'importance de nos travaux complémentaires sur cette proposition de loi. Nous avons entendu de nouveaux acteurs avec qui nous n'étions d'ailleurs pas toujours en accord même si nous poursuivions le même but, protéger davantage les épargnants. Cet objectif il est au coeur des chapitres de étroit de cette proposition de loi que je m'apprête à vous présentiez. Sur les frais d'abord nous avons 2 moyens d'agir. Le 1er Albéric de Montgolfier. On a parlé avec l'article 1er, c'est celui d'interdire ce qui nous paraissent. Inopportun ou redondants. Le 2ème moyen d'action indirecte mais aussi très efficace consiste à garantir les conditions d'un choix éclairé pour les épargnants. En assurant une transparence accrue sur la performance des produits en tenant compte de tous les frais les épargnants seront alors en mesure de choisir les produits les plus rentables et adapté à leurs besoins. Quand nous parlons de ces informations, on ne fait pas référence à un document qui manqueraient de lisibilité ne n'en facilitant pas d'ailleurs la compréhension document que l'épargnant au mieux range rapidement dans un tiroir lorsqu'il est. Lorsqu'il rentre L'affichage du coup complet des produits doit conduire. À entretenir et à stimuler la concurrence entre les acteurs et à exercer une pression à la baisse sur les frais. L'article 3 imposent tout d'abord au distributeur d'assurance-vie et aux gestionnaires des plans d'épargne retraite de présenter lors de la constitution d'un contrat ou d'un plan. Les fonds indiciels côtés disponible. Pourquoi ces produits en particulier parce que ces fonds le plus souvent d'ailleurs en gestion passive. Présentent un niveau de frais généralement inférieurs au fonds en gestion active. Pour une performance nette en moyenne égale ou supérieure. Or, ces fonds ne sont quasiment jamais proposé à la souscription. Parce que trop peu rentable pour les distributeurs et les conseillers. Leur présentation pourrait donc entretenir une saine compétition et il est vraiment temps que les distributeurs se saisissent de ce sujet. Ils prennent le risque sinon de se voir dépassée par les nouveaux acteurs qui, eux, proposent des fonds indiciels côtés avec en plus une souscription sur internet. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment mieux pour les épargnants et je préférerais que les distributeurs que je qualifierais de traditionnelle qui ont la confiance des épargnants s'empare pleinement du sujet. L'article 4 permet quant à lui de remédier. Un obstacle que nous connaissons de longue date, à savoir l'impossibilité de disposer d'une information claire sur les frais totaux des produits financiers désormais l'ensemble des épargnants pourront accéder à une information lisible publiées sur les sites internet des établissements et par ailleurs les informations communiquées aux contrats contractants ne se auront plus seulement sur la performance annuelle mais sur la performance pluri-annuel des produits dans le même temps, le comité consultatif du secteur financier dans un format d'ailleurs rappelant celui de l'Observatoire des tarifs bancaires sera chargé de suivre les pratiques tarifaires de l'assurance vie et des plans d'épargne en actions, ouvrant la voie à une comparabilité objectif des produits. Je crois que Monsieur le Ministre partagera cet avis. Cet article est capital. Il constitue une véritable avancée au service de la transparence et de la bonne information des épargnants. Les unités de compte seront classées par performance nette. C'est plus lisibles pour chacun, à charge ensuite et c'est normal au conseiller de faire son travail pour constituer le panier de produits le plus approprié comme l'ont d'ailleurs souligné rappelé nos collègues en commission, peu de personnes peuvent spontanément comprendre ce que l'on veut dire par valeur brute en cas de rachat ou plus-values potentielles. Ce sont des informations, je dirais plus concrète dont ont besoin les épargnants. Je passe désormais au chapitre trois, notre proposition de loi relatif au développement à l'adaptation des produits d'épargne. Nous pouvons en fait ici distinguer 2 types d'articles. Ce qui lève les contraintes pesant sur certains produits d'épargne et ceux qui tendent envisager ou encourager une véritable concurrence sur le marché de l'épargne. Concernant les premiers rapidement l'article 5 propose un droit à l'erreur sur l'EPA, avec la possibilité. Pour l'épargnant de ne pas perdent l'Avantage fiscal s'il vient à corriger son erreur par exemple d'achat de titres non éligibles au PEA. En complément, l'article 5 bis vise à assouplir légèrement le Champ des titres éligibles OPA pour favoriser l'accessibilité des produits de capital-risque encore trop méconnu. Sur le développement du capital investissement. La commission a sur notre proposition, supprimer l'article 6, qui portait sur le dispositif Madelin dont nous avons eu l'occasion de débattre récemment dans le. Le cas du dernier projet de loi de finances. Preuve de notre bonne foi. Monsieur le Ministre, nous sommes d'ailleurs prêt à attendre les résultats de l'évaluation de ce dispositif avant de proposer de nouvelles mesures. Concernant l'encouragement de la concurrence sur le marché de l'épargne. J'en viens à cet instant un sujet. Qui nous est particulièrement cher et qui ne manquera pas, j'en suis sûr de susciter quelques débats. C'est l'article 7 et la transférabilité des contrats d'assurance vie. Il comporte 2 volets relatifs à la fois à la transférabilité interne d'une part et externe d'autre part, il s'agit d'abord de lever les obstacles au développement de la transférabilité interne que l'assuré pourra demander à tout moment à l'assureur ou un intermédiaire, lequel sera désormais tenu de réaliser le transfert dans les 2 mois. après le passage en commission cet article consacrent désormais un droit au transfert interne, sans possibilité pour les assureurs de s'y opposer, tout en limitant les frais pouvant être imposées lors de cette opération. Faire du transfert interne droit vraiment opposable est un progrès indéniable. Les dispositions que nous vous proposons permettront de donner leur pleine portée à ce que nous avions d'ailleurs voté dans le cadre de la loi pacte. Déjà et d'ailleurs à ce moment-là on nous prédisait que le transfert interne à les conduire à l'écroulement du marché de l'assurance vie. Et à une forte instabilité financière. Tout le monde s'y est opposée et nous voilà 3 ans plus tard à renforcer unanimement la portée ce dispositif. Sans surprise, j'ose le dire. Nous faisons face aujourd'hui au même qui dort avec la transférabilité externe. Le second volet de l'article sept autorise en effet le transfert externes des contrats d'assurance-vie avec portabilité de l'antériorité fiscale. À peine. Ses dispositions, a créé de vifs débats avant même que nous ayons eu le temps de présenter les garde-fous prévus pour l'encadrer. il convient. D'avoir une vision nuancée des conséquences attendues de cette mesure. Elle ne porterait que sur les contrats de plus de 8 ans et surtout elle pourrait améliorer la qualité des conseils prodigués aux épargnants. Ces derniers auraient d'ailleurs d'autant moins de raisons de quitter leur intermédiaire ou leur assureur, si ce dernier vient à leur proposer des produits plus approprié plus rentable que ceux souscrit initialement. Prenons un exemple des contraintes qui pèsent sur les épargnants. En l'absence de transférabilité. Personne n'avait entendu parler des produits verts il y a 10 ans maintenant de plus en plus d'épargnants veulent verdir leur épargne et soutenir la transition écologique. Monsieur le Ministre, allons-nous leur dire qu'ils sont prisonniers d'un produit souscrit il y a des années et qui ne peuvent pas réorienter leur épargne. Si c'est votre position, vous êtes has been. Notre objectif ici est donc simple éviter aux épargnants d'être captif et de susciter une plus grande concurrence ce qui encouragerait d'ailleurs en amont des pratiques de conseil plus active et plus adaptée aux besoins des assurés de la part des intermédiaires et des assureurs. Et d'ailleurs précisé qu'en cas de rachat du contrat l'assureur peut évidemment proposés à l'assuré des options de transfert internes pour conclure son renforcement de la transférabilité externe ou d'abus Thirion, qui a une transférabilité interne boiteuse. Et si vous me permettez de filer la métaphore. Je dirais que seul leur conjonction permettra à la liberté de choix de l'épargnant de marcher sur ses 2 jambes et de 2 exercer pleinement dans cette même optique, la commission introduit l'article 7 bis qui a institué à devoir de conseil dans la durée pour les intermédiaires et les assureurs. L'enjeu tu encore une fois d'adapter l'offre opposa à épargnants à l'évolution de son profil, c'est l'article 7 terre qui vise lui à prévoir exclut expressément une obligation de respect des engagements contractuels en cours d'exécution. Pour les 2 articles du chapitre III on aborde les sujets des plans tête bien que bien sûr, sans que cela ne doivent préempter le débat. Que nous aurons prochainement. L'article 8 enfin proroge jusqu'en 2026. L'incitation. Cal mises en place pour encourager le transfert de l'épargne des. S'ils ont un contrat d'assurance-vie. L'article 9 confie à la Caisse des dépôts, la gestion d'un fonds de fonds indiciels côtés qui seraient ensuite distribués dans les PER. Il s'agit tout simplement de proposer un produit peu chargé en frais aux épargnants. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous soutiendrez toutes et tous, notre démarche qui ne fait en fait que protéger les particuliers en améliorant développement encourageant et en soutenant le marché de l'épargne en France, le chemin est ouvert, ne perdons pas de temps, et sachons les uns et les autres être au rendez-vous de la responsabilité. Merci. Merci monsieur le rapporteur général et maintenant. Par le tout Ministre qui va relever le défi de la modernité. Monsieur le. Le président, monsieur le président de la commission des finances. Messieurs les les rapporteurs mesdames et messieurs les les sénateurs. Nous sommes réunis pour examiner la proposition de loi des sénateurs Husson et Montgolfier un texte qui propose de. Renforcer la protection des épargnants via une série de mesures articulée autour d'un triptyque information protection répression. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il contient, y compris après examen en commission plusieurs mesures que le gouvernement salut à vrai dire le le gouvernement accueille très favorablement cette. Proposition de de loi qui vient compléter un certain nombre d'évolutions récentes au bénéfice des épargnants, à l'exception. De 2 articles notamment qui vous feront peut être dire messieurs les rapporteurs que je suis un peu has been mais j'aurai l'occasion. À la fois à la tribune et et tout à l'heure dans le débat d'expliquer la position du gouvernement sur ces articles en matière d'information sur le contenu et les frais des produits financiers. Le gouvernement partage pleinement les objectifs de la proposition de loi exprimé en particulier dans l'article 1er et les articles 3 et 4. L'article 1er supprime les commissions de mouvement qui sont souvent peu transparente restreinte à un petit nombre de produits et qui altèrent la qualité globale de l'information sur les frais de gestion figurant dans la documentation commerciale. L'article 3, en créant une obligation de présentation des ETF produits simples et peu chargé proposés sur le contrat d'assurance vie ou sur le plan d'épargne retraite permettra de développer une classe d'actifs encore peu présente et incitera les gestionnaires d'actifs français à développer leur offre. Cette mesure est absolument fondamental, tant les ETF sont un moyen pour les épargnants français. D'accéder à des produits. Faible en coup. Mais dont la performance suit les les les grands indices et donc leur garantit une forme de de performance qui soit au minimum la même que celle des marchés d'actions. L'article 4 permet de poursuivre les efforts de la loi pacte pour renforcer la transparence des frais des contrats d'assurance vie et des plans d'épargne retraite cette transparence accrue permettra de stimuler la concurrence au sein du secteur et d'exercer une pression à la baisse par conséquent sur le niveau des frais pour stimuler le rendement de l'épargne. Par ailleurs, nous saluons la la création d'un observatoire de l'épargne, qui sera donc porté par le comité consultatif du secteur financier. Ces trois mesures sont de nature à permettre aux consommateurs de faire un choix mieux éclairé au moment d'allouer son épargne parmi les différents supports d'investissement. Le texte permet également d'encadrer certaines pratiques renforçant ainsi la protection des épargnants ainsi la création d'un mandat d'arbitrage en assurance-vie à l'article deux confère des garanties supplémentaires à l'épargnant. Dans un contexte où les pratiques du marché sont hétérogènes. Le gouvernement partage l'objectif poursuivi par les rapporteurs et proposera d'apporter des modifications concernant le Champ d'application les obligations du mandataire et la place des prestataires de services d'investissement. Le texte propose également de renforcer significativement le dispositif de contrôle des offres de vente de biens immobiliers dans le cadre de dispositifs fiscaux. Le gouvernement soutient cette proposition à l'exception de celle d'un rapport d'évaluation sur ces dispositions. ne semble pas utile. Compte tenu de la transparence donnée par la DGCCRF sur le bilan de ces enquêtes. Par ailleurs, les évaluations de ce type en matière d'effectifs sont très régulièrement demandées par le Parlement dans le cadre de travaux afférents au projet de loi de finances. Le Parlement a ainsi toute latitude à droit constant pour solliciter ces informations, le moment venu en matière répressive. Le gouvernement se félicite du renforcement des pouvoirs d'enquête de l'Autorité des marchés financiers par l'adaptation de ses compétences aux évolutions des offres de produits financiers et aux pratiques de marchés. La crédibilité de l'AMF est essentiel au maintien de l'intégrité du marché qui est le socle de la confiance des épargnants, dont la participation est nécessaire pour contribuer au financement de l'économie. Concernant la lutte contre le blanchiment. L'article 12 renforce les obligations déclaratives en matière de financement participatif sur une fraction des acteurs qui n'étaient pas encore couvertes le financement des parts sociales. Votre proposition permet de combler cette lacune. Je veux saluer au nom du gouvernement, les rapporteurs pour leur écoute et le travail préliminaire menée conjointement avec Bruno Lemaire qui a permis d'enrichir le texte et d'en renforcer sur certains aspects, l'ambition, je pense notamment au travail fructueux menée sur les dispositions concernant la transparence des frais. Ces travaux ont contribué à renforcer l'ambition du texte par exemple à travers la mise en place de l'Observatoire de l'épargne chargé de suivre l'évolution des frais de l'épargne assurantiel mais aussi des PEA et des PEA PME sur le régime de de contrôle des offres immobilières. Je remercie aussi la rapporteur pour la qualité des échanges et salue les avancées du texte adopté en commission est permise grâce à ce travail conjoint enfin je pense à la proposition des rapporteurs pour renforcer la protection des assurés, grâce à la clarification des obligations d'exécution. Des obligations contractuelles en cours de contrat. Cependant, le gouvernement conserve une divergence d'appréciation concernant l'article sept visant, entre autres, à mettre en place un droit à la transférabilité externes des contrats d'assurance-vie étant entendu qu'il accueille favorablement le renforcement proposée par les rapporteurs de la transférabilité interne de ces contrats d'assurance vie. La mise en place de la transférabilité externe constitue un risque significatif pour la stabilité financière et le financement de l'économie en période de remontée des taux, comme à l'heure actuelle les transferts obligerait les assureurs à réaliser les moins-values latentes en liquidant des obligations pour servir les demandes des assurés. La transférabilité externe créerait une situation de concurrence déloyale en bénéficiant à de nouvelles entreprises des entreprises en 30 ans, capacité d'investir dans des obligations à taux plus élevé qui pourrait ainsi capter les épargnants des assureurs établie et mettre en danger leur situation prudentielles les épargnants seraient les premiers perdants de la transférabilité externe, le rendement de l'épargne serait mécaniquement réduit car l'actif des assureurs s'orienterait vers des placements liquides et des obligations à maturité plus courte pour faire face à la demande accrue de rachat des épargnants. L'encadrement prévu par l'article est insuffisant pour limiter ces risques, la limitation de la possibilité de transfert au contrat de huit ans et plus est insuffisante car ces contrats de huit ans, représentent 70% du total des encours d'assurance-vie. Cette mesure est d'autant plus regrettable que, comme je le disais, le même article propose la mise en place d'un droit à la à la transférabilité interne. La loi pacte. Ouvrait cette possibilité là, la proposition de loi qui est soumise à votre examen. En créer un droit. Cette évolution constitue une piste prometteuse qui ira donc au bout de la logique de la loi pacte. à mon sens, que ces produits-là, les produits indiciels puisse se développer et dans l'intérêt général que les initiatives de la Caisse des dépôts ne soit pas redondantes avec celles du secteur privé afin qu'elle garde des marges de manoeuvre pour jouer un rôle contracyclique lorsque cela est nécessaire. Afin de répondre aux objectifs visés par la proposition. Stimuler le développement du offre de PER au niveau de frais contenu serait plus pertinent. Vous l'avez compris, ces 2 articles 7 et 9 seront les principaux points de discussion, que le gouvernement soumettra pendant l'examen que nous allons débuter. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre la discussion générale se poursuit avec la parole à Georges Patient. Pour le groupe RDPI et pour six minutes. Je le président. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Les frais encore pointé du doigt. L'accumulation des frais élevés peut dans certains cas amputé toute espérance de rendement.

Prononcer indique une fois de plus. Combien la question des frais notamment dans l'assurance-vie reste problématique. Le prix si dans Fougères préciser également. Que la mention des frais impliqués au plan épargne retraite et assurance vie désormais obligatoire depuis le 1er juin 2022. Sur les sites internet des établissements n'avait pas contribué à leur baisse. Bien au contraire. Si bien qu'une nouvelle recommandation des autorités aux professionnels sur ce point était attendue courant 2023. C'est dire que cette proposition de loi présentée par nos rapporteurs et auteur Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier. Arrive à point nommé dans cette quête dans cet appel à une plus grande protection des épargnants. Issu de leur rapport d'information sur la protection des épargnants dont elle traduit les principales recommandations de niveau législatif. On peut aisément concevoir que cette PPL fait consensus, à fortiori. Parce qu'elle reprend les conclusions d'une mission de contrôle sénatoriales transpartisane. Les rapporteurs ont mis l'accent sur un certain nombre de problèmes qui pénalise lourdement les épargnants français. Je citerai une concurrence entre entre acteurs limiter un nombre élevé d'intermédiaire ou encore un faible développement de la gestion passive. Ce structuration du marché de d'épargne se traduit aussi par un niveau de frais élevés qui pèsent sur la performance servis aux épargnants. Et certains des acteurs auditionnés ont tenu un discours particulièrement radical sur l'état du marché de l'épargne. Je pense notamment à la pratique des commissions de mouvement que l'article 1er propose interdire. Et qui a été vertement dénoncé par un certain nombre d'acteurs. Les épargnants subissent en effet une double facturation à chaque opération. Avec les frais de courtage et les commissions de mouvement. Chaque année ce sont 500 millions d'euros qui sont prélevés indument par les sociétés de gestion et les intermédiaires. Alors que ces pratiques sont interdites dans les autres juridictions européennes. Les rapporteurs ont déposé en commission 20 amendements sur leur propre texte. Tous les articles initiaux ont été réécrit et certains articles additionnels ajoutés. Signe que le dialogue des rapporteurs avec Bercy a été constructif. 3 articles sans néanmoins soulever des interrogations au sein de mon groupe. Le 1er concerne le droit à l'erreur fiscale. En cas de placement de titres non éligible sur un PEA ou un PEA PME. Que veut instaurer l'article 5, il n'y a-t-il pas là un risque d'inciter à placer des titres on en éligible sur un PEA, afin de bénéficier de ces avantages fiscaux. Tout en rejetant la faute sur le gestionnaire. Le second sujet porte sur l'article 7 et la transférabilité à tout moment de contrats d'assurance-vie entre assureurs. Je doute qu'une telle mesure conduisent à une réelle amélioration des tarifs des assurances vie pour les assurés. En revanche, elle pourrait s'avérer défavorables au financement de l'économie en contraignant les assureurs à préférer les placements de très court terme et sans risque, afin de pouvoir clôturer à tout moment en contrat. Enfin proposé un placement d'épargne retraite à l'article 9, en plein débat sur la. Sur la réforme des retraites est-ce. Opportun, même si la gestion confiée à la Caisse des dépôts serait peu chargée en fait. Aussi, si nous saluons le travail des rapporteurs qui dans l'ensemble va dans le sens d'une meilleure protection des épargnants. Nous espérons que la qualité de nos débats. Permettra de lever les doutes qui subsistent sur les sujets que je viens d'évoquer. Je ne saurais terminer mon propos sans faire mention des outre-mer. Tous les habitants d'Outre-mer doivent payer leurs produits financiers plus cher qu'en France métropolitaine. 10%. Quel est le surcoût que nos compatriotes ultramarins doivent pire leur banque en comparaison avec l'Hexagone. C'est ce que dévoile une étude menée par l'association des consommateurs CLCV. Contrairement aux tarifs bancaires, l'opacité des frais appliqué à l'épargne nous empêche encore d'avoir un état des lieux précis. J'espère que le comparateur officiel, les tarifs bancaires tenus par le comité consultatif du secteur financier. Ce rap-rapidement enrichie avec les données publiées

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur, le monsieur. monsieur. Les rapporteurs chers collègues nous examinons donc cet après-midi une proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants à l'initiative d'Albéric de Montgolfier de Jean-François Husson collègue que je veux remercier pour leur travail mené au nom de notre commission. Elle comprend de nombreuses mesures, souvent techniques que le groupe socialiste a. Soutenu la création par exemple d'une définition harmonisée de l'arbitrage en assurance-vie qui est une avancée positive alors qu'aujourd'hui les opérateurs disposent chacun de la leur, et ce dans une grande opacité pour leurs clients. L'instauration d'un devoir de conseil dans la durée pour les intermédiaires et les assureurs qui permettra d'adapter les offres proposées à l'assuré en fonction de l'évolution de son profil et de ses besoins. Cette obligation, qui s'appliquerait donc à l'occasion de toute opération susceptible susceptible d'affecter le contrat renforce ainsi la protection des épargnants. De même l'article 7 terre impose aux prestataires de services bancaires ou financiers, le respect de leurs engagements contractuels en cours d'exécution du contrat et l'article 13 renforce les pouvoirs du collège de l'autorité de l'autoroute en lui permettant d'asseoir ses injonction d'une astreinte. Nous avons toujours soutenu les mécanismes visant à assurer le bon fonctionnement des dispositions de contrôle et celui-là ne fera pas exception, idem pour la sécurisation du Champ de compétence de l'AMF pour les offre au public de parts sociales, comme les banques mutualistes ou les sociétés coopératives. Enfin, l'interdiction de la perception de commissions de mouvement sur le marché de l'épargne va dans le sens des mesures que nous avions défendu et adopté dans le cadre honneur de notre proposition de loi sur l'encadrement des frais bancaires. Je n'ai pas citer tous les articles. Mais je le dis au nom de mon groupe, la plupart d'entre eux vont donc dans le bon sens car il renforce à priori la régulation des marchés de l'épargne. en avons, nous l'avons évoqué en commission, nous avons regretté la présence de de mesures de nature plus fiscale en l'occurrence de des mesures de défiscalisation qui change la portée d'un texte au départ je pense davantage consensuel sur la protection des épargnants. Je me félicite donc que les rapporteurs du texte et de même proposé la suppression de l'article 600 commission. Même si c'est dans l'attente d'un rapport sur le sujet qui risque de ne pas nous rendent davantage favorable cela fait évoluer évidemment ne le regard que nous porte le groupe socialiste sur le texte d'aujourd'hui dans son ensemble. Il reste néanmoins quelques éléments qui relève, à notre avis davantage. De mesures fiscales que de protection des épargnants. Je pense à l'article 5 qui élargit l'Avantage fiscal attaché au plan d'épargne en actions, les PEA. Avec le garde-fous introduit en commission, cette disposition est basé sur un mécanisme préventif et correctif qui ne devrait cependant pas ou très peu créé de d'effet d'aubaine. Et surtout, l'article 8 proroge une disposition d'optimisation fiscale introduite dans la loi pacte pour un transfert de sommes d'un contrat d'assurance-vie vers un plan d'épargne retraite. En pleine manifestation même si nous sommes dans cette hémicycle contre la réforme des retraites est alors que. Partout dans notre pays. La mobilisation est très importante. L'adoption d'un tel dispositif ne paraît pour ainsi dire pas opportun et je leur dirais pas du tout de nous défendrons donc dans la discussion. Un amendement de suppression de cet article et j'ai bien noté l'avis favorable des auteurs du texte au retrait du dispositif afin de bien rester dans l'objet de la protection des épargnants. Mes chers collègues, vous l'aurez donc compris, nous ne sommes pas opposés à ce texte qui je viens va dans le sens des mesures déjà défendu par notre groupe sur les frais bancaires ou sur la capacité d'emprunt des personnes fragiles. Il participe à faire bénéficier les Français d'un peu plus de concurrence et de transparence en matière d'assurance vie. Et nous avons bien entendu les résistances exprimées par les assureurs, en en particulier sur la transférabilité externe argument d'ailleurs comme souvent repris presque mot pour mot par le gouvernement. cette situation montre bien qu'en la matière. Nous ne pouvons pas toutes à tendre de la bonne volonté des banques et de leur capacité d'autres ou de leur volonté d'auto- régulation et qu'il est nécessaire de légiférer pour rétablir un équilibre entre les Français épargnants et le système bancaire et assurantiel. D'autre part donc sous réserve de la discussion des articles et des amendements bien sûr la position du groupe socialiste sur l'ensemble de la proposition de loi devrait être favorable, je vous remercie. Merci, cher collègue, c'est maintenant. Pascal Savoldelli, qui prend la parole pour le groupe CRCE. Et pour cinq minutes. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mais mes chers collègues. Notre collègue Albéric de Montgolfier. L'auteur de la loi me questionnait avec humeur et humour à 14h en commission sur ma présence qui me demandait si j'étais gréviste. Je vais le rassurer. J'apporte mon total soutien aux grévistes et aux manifestations dans tout le pays. Signe que la démocratie sociale se mobilisent massivement lorsque ses intérêts fondamentaux sont menacés. Les retraites sont au coeur de notre modèle social. Et difficile de pas voir dans cette proposition de loi. Un agenda pour le moins troublant. Ce texte encourage par défaut quand même la retraite par capitalisation. C'est un projet politique cohérent. Que d'affaiblir la retraite par répartition ici par des exonérations de cotisations, la part des incitations à l'épargne de retraite individuelle. Excusez-moi mais votre complicité certes chaotique. En construction avec le gouvernement sur le projet de loi de retraites trouve dans ce texte des preuves supplémentaires d'une visée commune. Vous vous proposez de protéger les épargnants. Vous avez raison.

entre fin 2019 et fin 2020, les 5% les mieux dotés en Patrimoine. Écoutez-moi bien, ont augmenté de 21.000 euros leurs dépôts bancaires compte courant livrer des pas un compte en actions assurance-vie tandis que les 50% au Patrimoine financier le plus modeste non économiser que 800 euros sur l'année un grand nombre de n'a généré ni bas de laine 10 billets sous le matelas. Ils se sont tout simplement endetté que ceux qui n'ont pas des. Que ceux qui n'ont pas d'épargne financiarisé cessent de suivent nos débats. Ils ne sont pas concernés, la suppression par les auteurs eux-mêmes de la seule mesure de suppression des frais, des commissions de mouvement à l'article 1er État recul important. C'était le seul qui tendait au moins à lutter contres les gabegies des produits d'épargne financiarisé. Je m'excuse mais vous légiférer sous une autorité c'est vrai et vous l'avez dit en Corse l'après-midi sous une autorité sa salle des marchés financiers. En revanche, cette proposition de loi tente bel et bien de protéger les épargnants qui privilégie des plans d'épargne retraite et autres assurances vie pour se mettre à l'abri de leurs vieux jours ou plus certainement pour mettre à l'abri de l'administration fiscale, des sommes colossales. Je dis colossal. L'encours de l'assurance-vie s'élève à 2237 milliards en 2022. Les plans d'épargne retraite les PER, c'est 280 milliards d'euros. Bruno Lemaire qui a pas pu venir encore cet après-midi se félicite et la droite sénatoriale, l'encourage, je le cite le ministre-Lemerre quand il n'est pas obligé de parler à sa place le déploiement du PER est un succès majeur, ce produit d'épargne retraite permet aux Français de disposer d'un produit d'épargne avantageux pour préparer leur retraite. Enfin quelle ironie. Un succès tels que l'encours de 70 milliards du nouveau PER créé par la loi pacte provient pour soi dans 19% des anciens produits des plans d'épargne retraite. La loi pacte au moins eu le mérite de remplacer le nommer, plan d'épargne retraite populaire créé par François Fillon par un plan d'épargne individuelle qui dit là c'est vrai mieux son nom. Le rapporteur général et son prédécesseur ont décidé de supprimer l'article 8. C'était notre volonté également. Pas de prolongation du double Avantage fiscal sur la conversion des produits d'assurance-vie en plan d'épargne retraite. Vous évitez ainsi de mettre de l'huile sur le feu. Mais tout de même. Que tous ceux qui se mobilisent en ce moment même partout en France prenne le temps d'écouter un instant. Je me lance dans le conseil fiscal en citant Mariam Karoui ingénieur patrimonial au cabinet Haussmann Patrimoine, je la cite, nous recommandons principalement l'EPER à des personnes imposées à 41% vous m'avez bien entendu à 41% c'est la tranche d'imposition marginale de ceux qui ont près de 80.000 euros de revenus fiscaux de référence. Excusez-moi d'appeler ça une paille. Je reprends une question du média spécialisé option finance et je vous la pose, je cite, même si elle se développe l'épargne retraite restera-t-elle en conséquence un marché de niche réservée à une petite minorité de la population en mesure d'épargner fortement. Vous avez compris que j'avais une petite idée mais vous me direz si je me trompe. L'article 9 poursuit la même finalité de favoriser retraite par capitalisation par l'entremise de la Caisse des dépôts. Or la retraite par capitalisation. C'est déjà le chacun pour soi, alors même que la solidarité intergénérationnelle doit être sanctuarisée, alors même que l'épargne la plus sûre et la plus juste et la socialisation des salaires par les cotisations même alors même que depuis 90 les peurs alimentée. C'est incroyable, il y a eu des discours et des réformes alarmistes qu'ont fait croire au travers de ce pays qui ne n'aurait pas de retraite, c'est pour ça qu'il s'adonnent à des placements financiarisé dont ils ne connaissent ni les finalités sociales ni les finalités écologistes. Alors, mes chers collègues, nous voterons la moins près de la moitié des dispositions de cette loi. Par contre nous ne voteront pas le texte parce que franchement ce texte évacue le rendement social et écologique, je dis bien le chiffre et et vérifiable de 5727 milliards d'épargne populaire. Qui sont à nos yeux pas traiter dans ce projet de loi. Merci de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Michel Calvet. Qui a huit minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs généraux de la commission des finances, mes chers collègues. Il y a eu il y a peu de temps. La formule travailler plus pour gagner plus. Elle était bien connu, effectivement. Mais nos rapporteurs généraux ici en trouver une autre formule qui est payé moins pour gagner plus. c'est aussi pas mal parce que c'était le. Le, le titre de leur rapport. En 2021, sur. La protection des épargnants qui. 17 recommandations et le groupe de l'Union centriste tient bien sûr à féliciter. Albéric de Montgolfier et Jean-François Husson pour le travail qu'il avait ainsi été mené qui était important et qui aboutit ce jour à l'examen de la proposition de loi, enfin. Alors. Pascal Salomon Denis vient à l'instant de de citer les chiffres effectivement. Il y a dans notre pays. Un peu moins de 6000 milliards d'épargne des ménages. Le Ministre de l'Économie et des Finances ce week-end évoqué ses préoccupations quant à la dette de la France à l'aide de 3000 milliards, c'est-à-dire qu'on parle ici. En terme d'épargne de deux fois la dette. De la France, c'est dire qu'on est sur des sommes tout à fait considérable et si la dette constitue une préoccupation et nous partageons-nous au niveau du groupe de l'Union centriste. Les préoccupations du ministre de l'Économie et des Finances. À ce sujet, il faut effectivement que l'on trouve les moyens de réduire cette dette. Nous avons à côté. Une épargne qui est abondante Par rapport à ce qui vient d'être dit. Un instant je dirais que c'est pas un gros mot que de vouloir épargner. Je crois que c'est la volonté de beaucoup de nos concitoyens français. Ils le font bien sûr sur différents supports les supports de l'assurance-vie sont tout à fait significatif puisque il y a grosso modo un Français sur trois qui dispose d'un contrat d'assurance-vie un petit peu moins pour un total de l'ordre de 2000 milliards, c'est dire qu'il y a au-delà aussi. Des enjeux financiers extrêmement importants. Alors qu'-t-on observé. Notamment à à la lecture des rapports et et des conclusions des rapports qui ont été présentés par nos collègues. c'était une réelle opacité sur la réalité des frais que l'on paye au titre de cette épargne et cette situation n'est pas pour nous acceptable pour nous les membres du groupe de l'Union centriste est pas acceptable parce que il est légitime que tout ce qui est un Patrimoine qui est de l'épargne sachent combien ça leur coûte effectivement dès lors que cette épargne est d'autant plus confier à des interlocuteurs à des acteurs sur le marché et donc. On s'aperçoit finalement que c'est la plus grande opacité sur le sujet et il était nécessaire qu'il y ait une transparence cela fut fait d'ailleurs pour ce qui concerne les comptes bancaires courants de nos concitoyens hein qui dispose d'une information annuel sur l'état des frais qu'il paye, il était logique aussi qui liait la même chose. Pour ce qui concerne la part de l'épargne et je ne doute pas que les propositions qui sont formulées par les rapporteurs cet après-midi seront enrichies, des propositions des membres du groupe de l'Union centriste, moi-même et et Hervé Maurey. Nous avons déposé des amendements en ce sens permettant à notre avis d'enrichir. Les propositions de des rapporteurs. Alors parmi ces questions de frais, il y a bien sûr la question des commissions. De mouvement. Ce que l'on peut regretter, c'est que, c'est qu'il faille attendre 2026 pour. Que ces commissions de de de mouvement, cela a été dit par Albéric de Montgolfier dans son propos liminaire. C'est une singularité française. Et donc, il paraissait normal qu'elle soit supprimée. Nous aurions souhaité qu'on aille un peu plus vite parce que elle ne se justifie plus à notre sens Tiendront à la position définie par. Par les rapporteurs. Alors cette proposition de loi est également l'occasion d'évoquer d'autres frais qui sont payés par par les épargnants. Je pense en particulier à la proposition d'Hervé Maurey là encore sur ce qu'on appelle les frais sur succession effectivement là aussi on constate qu'il y a des pratiques totalement disparates souvent opaque et il importe que tout cela soit bien cadrée parce que il n'est pas légitime à notre sens que l'on profite de situations. Difficiles pour prélever une part des ressources. Des ménages, notamment les ménages les plus modestes, donc merci à à notre collègue Hervé Maurey d'avoir. Formulé des propositions en ce sens c'est extrêmement. Important et puis. Pour nous. Membre du groupe de l'Union centriste. Il y a la question de la transférabilité qui est aussi quelque chose d'important la loi pacte avait consacré cette transférabilité en interne. Pour nous en moi. Il n'y a pas de raison que l'on n'aille pas plus loin et que l'on n'encourage pas la transférabilité externe. Je crois que c'est une question de respect de la concurrence, c'est une question aussi de respect du choix des épargnants car il n'est pas tout de considérer qu'il paye par exemple trop de frais, mais s'ils ne peuvent pas changer de support. Constatant qu'effectivement, il paye trop de frais, cela paraîtrait anormal donc. Moi je dis que il est légitime que l'on puisse effectivement transférés des comptes je veux bien entendre Monsieur le Ministre qu'il y a quelques précautions à prendre Je souscris totalement aux propositions que le rapporteur général Jean-François Husson à formuler en ce sens tant dans le temps, on peut éventuellement aussi mettre des garde-refuge sur les sommes d'être transférés mais je crois qu'il est impératif que l'on puisse avancer sur cette transférabilité l'exemple qui a cité tout à l'heure sur. La transmission transférabilité interne qui avait été décrié au moment où la loi pacte avait été examinés montre la situation d'aujourd'hui montrent bien qu'il n'y a pas de raison pas de raison de s'inquiéter et qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le sens à la fois de la transparence et de la latitude laissée à nos concitoyens. Alors. Un autre sujet qui paraît important pour nous, membres du groupe de l'Union centriste. C'est bien sûr l'orientation de cette épargne. Il est d'abord légitime que le maximum d'épargne puissent être orientées vers l'économie. Donc nous avons à travailler pour que justement. Il en soit ainsi. nous considérons également, c'est le sens de quelques amendements que j'ai déposée. Qu'il est important que l'on prenne en compte les préoccupations d'aujourd'hui qui sont notamment la transition écologique et donc pour y arriver en sait que cela nécessite des moyens, si cela nécessite des moyens, il convient donc d'orienter autant que faire se peut, l'épargne vers ces investissements qui sont considérés comme essentiels pour l'avenir de Je vous invite messieurs les rapporteurs à reconsidérer votre position sur. Ces amendements destinés à orienter l'épargne vers. Les les la finance verte parce que il y a vraiment un enjeu d'avenir un enjeu d'accélération de cette transition écologique qui est bien entendu poser puis je voudrais conclure mon propos en. Remercions aussi le rapporteur Albéric de Montgolfier d'avoir introduit dedans la la question de la transparence sur les. Produits de défiscalisation de dans l'immobilier. Effectivement, on constate que bien. Beaucoup de nos concitoyens se fourvoie sur le sujet, il convient d'être beaucoup plus transparent. Merci de votre attention. Monsieur le président, Monsieur le ministre. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Passer la période budgétaire. La commission des finances retrouvent le temps de se pencher sur le sujet plus spécifique. C'est le cas avec cette proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants. Alors que l'inflation fait son grand retour dans l'actualité économique, 6% cette année environ après des années vous le dire, d'inflation faible voire nulle. L'épargne des Français est entré à une nouvelle zone risque. risque. L'le même conjugué à l'évolution parfois erratiques des valeurs boursières et tout de tirer encore bas malgré une nette remontée. Amorcée il y a un an Tan érodé la valeur des fonds placés en produits d'épargne rappelons. Que pas la moyenne des français est l'un des plus élevés des pays développés. Et ceux-ci de l'inquiétude collective face à l'avenir ou d'un pessimiste de se de se voir attribuer à notre peuple ou bien simplement dû au plus grave n'prévoyance ancré dans la culture nationale. En tout cas. On est loin du comportement des cigales. Quand vous souvent prêtée à nos concitoyens, il y a plus d'un siècle, la phrase était considéré comme le banquier du monde. Une population encore majoritairement rural. Habituer à économiser et dans l'État n'avait plus fait défaut sur sa dette. Depuis la révolution jouissait alors d'une. Puissance financière exceptionnelle, avec toutefois des des des communes historiques comme l'affaire des emprunts russes. C'est pas dans la première guerre mondiale où les nombreux scandales financiers. Qui ont émaillé l'histoire de la IIIe République, revenons au présent.

Sur longue période. Il est d'une assez grande stabilité autour de 15%. En comparaison aux États-Unis, le taux sur le long terme. Oscille autour de 6% seulement il y a en Allemagne et autour de 10%, seule la Suisse affiche un taux d'épargne supérieurs à la Laval. Un plus de la conjoncture actuelle. Les auteurs de la proposition de loi considère que le marché français de l'épargne souffrent de défauts structurels au détriment des épargnants. La majorité de l'épargne des Français et placé sur des comptes bancaires des livrets réglementés,

Faut-il pour autant se diriger vers une gestion de l'épargne à l'américaine, avec aussi les risques qu'une telle gestion comporte. Gageons que ce ne sont pas l'objectif des auteurs de cette PPL. Il est vrai en revanche que les différents frais liés à la gestion de l'épargne représente de du monde dans non négligeable pour les épargnants et souvent à six mois le colis. Je ne vois pas monétaire dans mon collègue Christian Billac en commission des finances. C'est l'année dernière. Il était important de revenir à une information claire et surtout personnalisés, adaptés aux beaux seins nus clients et si il faut plutôt il a une telle information sur la valeur nette des placements que sur la valeur brute et autant d'informations sur les frais potentiel que sur les plus values potentielles qui veut donner la moins des chiffres avancés par les auteurs de la PPL, je cite. Un particulier faisant le choix de commencer à épargner. Très tôt pour sa retraite pourrait voir la performance de ces placements 40 ans capter à plus de 55% par les vrais quand c'est où ces chiffres. Comment s'explique-t-il. Les chapitres sur l'encadrement des fruits et de la meilleure transparence apparaisse comme une bonne mesure pour des opérations dans l'épargnant. Soit même pas connaissance. J'aimerais me dérangent le bien fondé. L'article 5 bis. des fonds en paiera des fonds de placement à risques. J'aimais aussi réserves sur les dispositions de l'article 16. Et elle va introduire une commission et qui supprime le délit d'entrave aux enquêtes et contrôle de l'Autorité des marchés financiers pour les remplacer par une simple sanction administrative. que cette qui prolonge une mesure déjà votée dans la loi pacte. Assurera une tragédie transférabilité complète de l'assurance vie serait un réel progrès dans la mesure où il donnerait une lib liberté bien supérieur à l'épargnant dans la gestion de ses placements. Conclusion, les membres du aider lui se salue la qualité du travail accompli par les auteurs du texte. Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier et devrait se prononcer par sur pour savoir rédemption. À moins que des modifications importantes ne nous soit apportée en cours de séance. Si cher collègue. La parole est à madame Christine Lavarde. Pour le groupe des Républicains. Et elle dispose de 4 minutes. Merci Monsieur le Président. Alors sans trop de surprise, mon propos va se concentrer sur l'article 7. En effet il y a 4 ans jour pour jour dans cet hémicycle j'ai défendu un amendement qui visait à autoriser la transférabilité externes des contrats d'assurance-vie alors à l'époque le ministre-Lemerre s'y était opposé et il m'avait proposé de retravailler ensemble sur la concurrence entre les produits d'assurance-vie alors j'attends toujours l'invitation. 4 ans plus tard. Heureusement le Sénat lui a continué à travailler. je voudrais revenir sur 2 sujets déjà la transférabilité interne au sein d'une même entreprise. Assurance vie, sorte de pis-aller, qu'on nous avait accordé à l'issue de la commission mixte paritaire. Alors j'ai bien entendu cet après-midi et que le gouvernement soutient pleinement toutes les démarches qui visent à conforter ce principe. Alors il existe encore un certain nombre de freins de difficultés qui sont rencontrées au quotidien par les acteurs concernant la transférabilité interne en effet la moindre faille la moindre imprécision législative est utilisé par les assureurs ou les courtiers. Pour ne pas donner droit aux demandes des clients parce qu'ils sont en quelque sorte toujours réticents à cette transférabilité les amendements qui ont été adoptés en commission des finances à l'initiative des rapporteurs vont dans le bon sens. Moi il me semble qu'il y a encore un certain nombre de points qui pourraient être précisés. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé 2 amendements en ce sens mais surtout le gouvernement par la bouche du ministre Barrot vient de nous dire cet après-midi à qu'il continuait à s'opposer à la transférabilité externes et 2 arguments sont souvent exposés sur lesquels je voudrais revenir. Alors déjà la transférabilité externe par les sorties qu'elle entraîne empêcherait le bon financement de l'économie. Alors je voudrais juste vous rappeler, Monsieur le Ministre qu'aujourd'hui les compagnies d'assurance, elles sont obligés de respecter un certain nombre de ratios qui sont fixées par le code des assurances, elles doivent aussi respecter la directive européenne Solvency toi. Donc vous voyez bien il y a que ce c'est ce cadre-là. cadre-là. Qui impose les différents ratios et la nature, la proportion d'actifs que doivent détenir les les compagnies d'assurance et donc la transférabilité externe, elle n'aura absolument aucune conséquence sur ses différents ratios et elle ne viendra pas limiter les investissements en actions. Enfin, vous nous avez redit à l'instant que la transférabilité externe parce qu'elle déclencherait des sorties et des entrées amènerait les assureurs à devoir gérer des conditions de marché qui ne leur font pas forcément toujours favorable. Alors je voudrais juste quand même vous rappeler ici de l'ordre de grandeur des mouvements qui existe déjà en 2021 nous avons eu 148,6 milliards de versements en assurance-vie, nous avons eu 126,2 milliards de rachat. Donc là vous voyez bien que c'est des mouvements avec des qui entraîne des conséquences sur la gestion de portefeuilles des assureurs. Je prends aussi le rapport de France assurance de France assureurs pardon qui nous donne les chiffres de la transférabilité sur 2021, 657.000 contrats ont été transférés en 2020 et 2021 pour un montant de 21,9 milliards d'euros et au 1er semestre 2022 le mouvement poursuit son et son essor 128.000 transfert de contrat pour 4 5 milliards d'euros. Tout ça a bien évidemment a rapporté au volume d'encours de l'assurance-vie qui a été rappelé 1000 mi-. 1874 milliards d'euros. Alors juste pour vous le dire dans le cas de la transférabilité interne. Les fonds du contrat du contrat à sont vendus et réinvestit ensuite dans le contrat bé pour la part en euros compréhension et aujourd'hui j'entends pas. Les assureurs se plaindre de ses problèmes de transférabilité je les entends pas non plus se plaindre quand ils doivent gérer des mouvements de rachat de la part de leurs clients. Alors pourquoi aujourd'hui et c'est des choses qui existent depuis longtemps le transfert habilité externe qui va pas entraîner du jour au lendemain des mouvements de déstabilisation d'une importance telle je rappelle toujours l'encours total 1874 milliards entraînerait des craintes de la part du gouvernement. Si c'est juste à nous dire que vous avez peur que des compagnies d'assurances en difficulté puissent être mise à mal par des clients qui auraient peur alors pourquoi doit-on sauver des assureurs zombie. C'est la question, je vous pose. Est Madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe des Indépendants. Et pour. Cinq minutes.

Et constaté pardon fin juillet par la Banque de France de l'épargne accumulée par les Français depuis le début de la crise sanitaire. C'est plus que le montant du plan de relance. C'est plus aussi que le montant des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Le phénomène est désormais bien connue. Avec les mesures de restrictions sanitaires, la consommation a chuté, alors que les mesures de soutien au pouvoir d'achat ou préserver les revenus des ménages. En conséquence, l'épargne a explosé et atteint des sommets sans précédents. Mais ce que révèle l'étude de la Banque de France, paru en septembre dernier, c'est que ce phénomène perdure, alors même que les restrictions sanitaires ont été levées. Cette sur épargne Covid nous rappelle que les pagnes constitue d'abord un moyen de se protéger, surtout quand l'avenir est assombri par les incertitudes. Or, ce qui a changé depuis mars 2020 c'est que notre pays a renoué avec l'inflation alors que la plupart des économistes pensaient que ce phénomène ne nous concernait plus du tout. L'inflation constitue aujourd'hui la principale menace pour l'épargne des Français elle lancèrent en effet dans un étau. D'une part parce que les prix augmentent la fraction de la consommation dans le revenu des ménages augmente augmente aussi ce qui mécaniquement diminue la fraction affecté à l'épargne. D'autre part, la hausse des taux d'intérêt qui accompagne l'inflation ne suffit pas à compenser l'augmentation des prix. On le voit avec le taux du Livret A, récemment rehaussé à 3% bien en-deçà du tout de l'inflation en conséquence l'épargne de nos concitoyens a tendance à s'éroder. C'est pourquoi je tiens à saluer la proposition de loi présentée par nos collègues Albéric de Montgolfier et Jean-François Husson, pour protéger les épargnants. Leur travail a été engagée bien avant l'envolée de l'inflation. Dont, dont je fais part notamment avec un rapport d'information qui a été publié en octobre 2021. D'où la proposition de loi présente reprend les cours les recommandations d'ordre législatif. Il s'agit pas d'un texte de circonstance. Mais les circonstances actuelles, le rendre encore plus pertinent. Si la plupart des articles, y compris les nombreux qui ont été rajoutés en commission semble très technique. Ils apportent des mesures bienvenu pour les épargnants. C'est notamment le cas pour l'article 7 qui garantit une réelle transférabilité des contrats d'assurance vie. Une telle mesure devrait rendre le marché plus concurrentiel et donc améliorer les prestations de gestion de ces produits. Elle donne également davantage de liberté aux épargnants en leur permettant de choisir l'option qui leur convient le mieux. Nous l'avons vu encore récemment avec la résiliation à tout moment des contrats d'assurance-crédit. Les Français se sont emparés de cette nouvelle liberté. Ils le feront désormais aussi à leur Avantage pour faire jouer la concurrence en matière de contrats d'assurance-vie. Dans le même esprit. Je tiens aussi à saluer l'assouplissement des critères d'éligibilité des quotas. FCPR au PEA. Cela favorise le financement capital-risque notamment pour les jeunes entreprises innovantes. Et tout ceux qui financent notre économie particulièrement. Par les temps qui courent est encourager. La proposition de loi porte également plusieurs mesures d'encadrement et de régulation. Elle vise à protéger les épargnants contre des pratiques qui pourraient les induire en erreur. Cependant, certaines de ces mesures risquent de manquer d'efficacité car on le sait bien, mes chers collègues, les opérateurs et notamment les banques trouvent toujours un chemin pour les contourner. C'est ainsi que le bien connu, s'agissant de la régulation bancaire certaines pratiques soulèvent des indignations. Le législateur légifère et les banques finissent par contourner ces interdictions sous le vent, toujours de nouvelles indignation. Dans ce cas, il est à craindre que la régulation des pratiques bancaires ne soit un travail à la Sisyphe jamais. Toujours à recommencer. Dans le registre des pratiques bancaires peu recommandables. Mes chers collègues. Il en est une qui a soulevé l'indignation du public, grâce notamment à une publication du magazine, l'UFC Que Choisir que nos concitoyens connaissent bien. Il s'agit du prélèvement de frais bancaires sur le compte des défunts. Je vous proposerai un amendement pour. Encadrer très strictement ces pratiques. Cet amendement reprend en partie une proposition de loi que j'avais déposé sur le sujet. Voici près d'un an. J'espère que notre assemblée pourra légiférer sur ce point, afin d'envoyer un message fort pour mettre un terme à ces pratiques qui ajoute de l'indignation à la peine des familles qui écornent la confiance que les Français peuvent avoir dans leurs institutions bancaires. Vous l'aurez compris, notre groupe soutiendra cette proposition de loi. Qui va dans le bon sens et je vous engage, mes chers collègues à voter pour les amendements que nous proposerons je vous remercie. Merci, cher collègue, c'est parfait pour le timing maintenant, la parole est à Monsieur Daniel Breuiller pour cinq minutes également. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la commission. Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Tout d'abord je voudrais saluer les travaux de contrôle du, du Sénat et de sa commission des finances, sous l'impulsion de nos collègues de Montgolfier et Jean-François Husson. Le groupe écologiste soutient les mesures qui visent à accroître la transparence dans tous les domaines et singulièrement dans le domaine bancaire et à amoindrir les frais d'épargne la double charge pour les pour les épargnants et particulièrement inique et votre proposition de loi en interdisant notamment la perception de commissions de mouvement tend à répondre à cette problématique, comme la transparence accrue sur les investissements immobiliers absolument nécessaire. Toutefois, nous ne partageons pas votre vision et vos propositions sur les contraintes du marché au chapitre trois, quand vous voulez notamment encourager les épargnants à mobiliser leur épargne au profit des entreprises. Cette thèse néo-classique de la hausse de l'épargne qui bénéficie toujours à l'économie n'est pas la nôtre, parce que pour être efficient qu'il faut qu'elle soit orienté vers la transition écologique de l'activité économique et sans doute aussi vers l'économie sociale et solidaire. Plusieurs amendements l'évoque plutôt que sur la financiarisation de cette épargne la période d'inflation que nous traversons frappe de plein fouet les petits épargnants et je pense bien sûr aux 55 millions de détenteurs d'un Livret A et plus particulièrement à tous les foyers modestes qui ont un encours inférieur à 1500 euros. Ce sont eux, effectivement, qu'il convient d'abord de protéger ils sont nombreux et nombreux The à avoir d'abord et déjà dû renoncer à une partie de leur épargne pendant les confinements, quand effectivement les plus aisés d'entre nous augmenter considérablement leur épargne les plus modestes étaient souvent contraints de la consommer. La limitation des frais et la transparence sont donc nécessaires pour ces personnes modestes car la réduction des inégalités doit toujours demeurer la la priorité. Nous sommes là au coeur du problème, il est indispensable de rétablir une fiscalité juste sur les revenus des épargnes accumulées, ce Patrimoine ne dort pas, il génère des revenus supplémentaires pour les ménages les plus aisés, mais encore plus pour les établissements financiers. depuis la mise en place de la flat tax à 30% en 2018, ses revenus sont moins taxés que ceux du travail. Je profite de ce texte pour rappeler à cette occasion que notre groupe est opposé et souhaite la même imposition pour le travail que pour les revenus financiers. Je souhaite enfin parler un instant de l'impact social et environnemental des comptes bancaires et de l'importance de réguler les activités des banques. Objet de la proposition de loi ce sujet soulevé par Oxfam France en 2020, démontrait combien notre argent mis en banque finance potentiellement de projets polluants en France comme à l'international et révélé l'empreinte carbone colossales, des banques françaises. Les activités de financement et d'investissement des 6 principales banques françaises représentent près de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Il est donc urgent de réguler les banques françaises Oxfam France recommande d'ailleurs de créer un Label en transition qui pourrait venir éclairer et définir un degré d'alignement d'un portefeuille avec l'accord de Paris sur le climat, nous soutenons bien évidemment cette initiative concernant cette proposition de loi, elle est bienvenue sur la protection des épargnants et d'exigence de plus de transparence et ne répond peut être pas suffisamment aux enjeux de justice fiscale, sociale et environnementale que nous défendons. Nous avons un doute notamment sur la question de la transférabilité externe mais j'écouterai avec intérêt les débats et les réponses. Cette proposition introduit à l'article 8, un lien au débat en cours sur la retraite que nous ne pouvons souvenir soutenir et je salue l'avis favorable donné à l'amendement de retrait de cet article. ce texte m'a contrarié non pour son contenu mais parce qu'il m'a imposé de rentrer trop rapidement de la manifestation contre une réforme de retraites que je juge injuste, inefficace et inutile. Malgré cela, nous serons attentifs à l'écoute des argumentaires et prendrons notre décision vue du traitement des amendements présentés. Merci cher collègue. La parole maintenant monsieur Vincent Segouin pour les républicains. Et dispose de 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'assurance vie est aujourd'hui le placement préféré des Français, on l'a dit avec 45% des ménages qui possède un contrat en assurance-vie presque 50 millions de contrats individuels répertoriés pour un total de près de 2000 milliards d'encours. La durée moyenne de détention d'un contrat en assurance vie, et de 12 ans qui permet au gestionnaire du secteur bancaire et assurantiel d'accompagner de dettes des États et le développement des entreprises sur le long terme. Cependant, avec la chute des taux d'intérêt la meilleure rémunération des fonds euros est passé de 5,3% en 2000 à 0,8% en 2022, a subi d'importantes conséquences poussant les gestionnaires orienter les épargnants vers des unités de compte de la rémunération est plus attractive mais aussi plus risqué. Ces unités de compte sont des investissements confiée à des gestionnaires de fonds avec des orientations ciblée sur les actions, obligations nationales, européennes, internationales, comme les fonds verts ou j'en passe. La rémunération des épargnants et donc aujourd'hui plus aléatoire moins sûrs moins linéaire car plus risqué mais sur le temps long plus favorable. De même, il apparaît plus éthique d'investir sur de la valeur d'entreprise et de la croissance que sur de la dette des États. Mais il est vrai que les frais de gestion peuvent venir sérieusement diminuer les rémunérations. La proposition de loi de mes collègues Husson une Montgolfier met en évidence une opacité des frais qui pénalise les épargnants à premier un rapport était sorti en 2021 et a permis certaines avancées de la part des gestionnaires, et de là mais l'AMF sur la transparence des frais avec de nouvelles obligations pour le 1er janvier 2026, on en prend acte. Après ce 1er chapitre sur l'encadrement des frais. La proposition de loi de nos collègues propose aussi la transparence de la performance des produits. Qui est une condition clé pour assurer un choix éclairé pour les épargnants et stimulante pour la concurrence. Ces quatre premiers articles sont donc particulièrement dirigée vers les épargnants afin de leur garantir une information claire et transparente pour guider au mieux leur choix. Cependant, je m'interroge sur l'ensemble des obligations imposées aux gestionnaires dans les lettres annuel. Je reste convaincu qu'on ne remplacera remplacera pas le Conseil la confiance parle des obligations et des devoirs qui rendent l'information trop lourde et 2 hommes de moins en moins lisible pour les épargnants. Mais l'Arctique de cette proposition de loi. Qui m'apparaît le plus important et dont la mise en place pose question à l'ensemble des acteurs et sans doute l'article 7. Il a pour objectif de permettre une véritable transférabilité, interne et externe des contrats d'assurance-vie au delà de huit ans. De transférabilité externe est actuellement impossible. Les épargnants doivent racheter leur contrat au risque de perdre l'Avantage fiscal à qui au au-delà des 8 ans. La transférabilité interne est aussi compliquée et dépend du bon vouloir des gestionnaires en cas de refus trop souvent l'épargnant rachète et ne remplace plus forcément les sommes sur l'assurance-vie qui est pourtant censée le suivre tout au long de sa vie. Prenons un exemple. Vous avez un souscrit un contrat d'assurance-vie il y a 8 ans chez un gestionnaire de Patrimoine qui a placé dans une compagnie. Le gestionnaire de Patrimoine n'est plus là aujourd'hui et la compagnie a été racheté par une autre compagnie qui ne souhaite plus avoir de réseau physique. Votre situation change et vous souhaitez faire le point. Il n'y a plus personne. Vous allez voir, donc un nouveau conseiller qui vous avise de renforcer les versements sur l'assurance-vie pour préparer vos prochaines étapes de la vie, il aura alors l'obligation de vous conseiller de le faire sur le contrat existant car il bénéficie dit de l'antériorité fiscale de 8 ans. C'est une obligation voulue par l'autorité de contrôle et les législateurs qui entrave dorénavant le choix d'épargnants. Certes, le législateur a souhaité rendre répréhensible des actes commerciaux qui désavantage des clients mais attention aux limites de ses lois. L'absence de transférabilité empêche donc l'épargnant de faire les bons choix et d'opter pour les conditions qui correspondent le mieux à sa situation personnelle et à ses objectifs. C'est pourquoi je suis favorable à transférabilité, à la condition que la durée minimum de 8 ans soit respecté. J'entends cependant la crainte des gestionnaires qui s'inquiète du nombre de rachat et de l'obligation de garder une réserve pour répondre à ces demandes. J'entends aussi leurs réserves. Quant à. La part des parents qui ne pourront plus placé pour répondre au rachat. Avec un chers collègues de performance qui diminue. Vous avez perdu. Au final ce suis désolé mais je ne crois pas aux risque majeur que cela puisse entraîner et la transférabilité apportera plus de confiance aux épargnants qui pourront changer de gestionnaire ou d'intermédiaires en conclusion, comme le groupe LR, je suis favorable.

monsieur le président, Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues. Aujourd'hui nous débattons de la concrétisation législative du long travail de nos rapporteurs généraux. Monsieur de Montgolfier monsieur Husson sur un sujet structurant tant pour le pouvoir d'achat des Français que pour le financement de l'économie. J'adresse mes remerciements aux deux rapporteurs pour cette belle opportunité mon intervention portera sur 2 points. D'abord le modèle de rémunération des produits d'épargne qui fait l'objet de débats, tant au niveau européen qu'au cours des travaux de la mission d'information qui a précédé cette PPL. Pour moi, au coeur de la protection des épargnants le conseil financier doit demeurer accessible au plus grand nombre d'épargnants et ne doit pas être réservé aux seuls ménages qui peuvent s'acquitter d'honoraires. Le modèle de commissionnement actuel doit être préservée. Les risques sont contrôlés par nos régulateurs nationaux aujourd'hui un épargnant trouve normal d'être conseillé par un salarié de la banque ou de l'assureur puisqu'il a choisi et qui lui vend le produit. À l'inverse, celui qui ne peut pas se payer une prestation de conseil réalisera ses investissements seul devant son écran sur des plateformes plus ou moins encadrés qui leur orienteront vers des produits à la mode comme certains cryptoactifs pour ne citer que cet exemple. Le 2ème point ses portes pour l'assurance-vie comme beaucoup de mes collègues. Depuis 18 ans ici au Sénat, nous avons fait progresser le placement préféré des Français. D'abord sur la déshérence des contrats d'assurance puis sur l'information des assurés. J'ai modestement contribué, nous avons réussi à faire évoluer au bénéfice des assurés. Malgré la frilosité des assureurs et sans jamais fragilisé ce secteur clé de l'économie française, quoi qu'on disait à l'origine et l'assureur. C'est pourquoi je crains messieurs les rapporteurs que la transférabilité total prévu dans la PPL même avec les garde-fous proposés n'ait des conséquences sur le financement à long terme de nos entreprises. La transférabilité réduira forcément l'horizon des investissements et orientera l'épargne sur des actifs. De plus court terme et moins risqué pour pouvoir faire face à des sorties facilité et donc importante, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une voie médiane. Ahan qui dynamisera l'assurance vie sans la dynamiter avec un des amendements qui porte à 12 ans la transférabilité externes car seulement un tiers des contrats d'assurance ne serait seraient concernés. Je tiens aussi à conclure pour me réjouir de la richesse de vos travaux en commission et sur le renforcement de la transférer par habilité interne qui ouvrira de nouvelles opportunités pour l'assurer et je ne vois pas comment et pourquoi les assureurs pourraient s'y opposer. Merci beaucoup cher collègue et. Nous terminons la discussion générale avec monsieur Jean Rey vont Hugonnet qui a également trois minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Aujourd'hui l'épargne des Français atteint des sommets et plus que jamais, il nous faut veiller à la protection des épargnants. Cette épargne se heurte pourtant à un manque de transparence notamment sur les frais et les produits disponibles. Le nombre élevé d'intermédiaires participe également à une forme d'opacité entretenue par une concurrence insuffisante. Tout ceci tire vers le bas les performances servis aux épargnants qui finance, pourtant, ne l'oublions pas. L'économie réelle de notre pays. Nous avons donc besoin de comme ils ont besoin de nous. Notre responsabilité. Est aussi de protéger le pouvoir d'achat des ménages, surtout en ce moment. En sécurisant les revenus complémentaires issus des placements de nos concitoyens. L'interdiction des commissions de mouvement. Le référencement des produits indiciels à Bakou. L'amélioration de l'information disponible sur les frais de l'assurance-vie ou encore une réelle transférabilité de celles-ci constituent autant de pistes évoquées par nos éminents collègues Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier il y a quelques mois dans leur rapport d'information intitulé la protection des épargnants de points payer moins et gagner plus. Voilà un véritable objectif. La proposition de loi qu'ils ont déposé à l'issue de ce travail en profondeur traduite au niveau législatif les juste recommandations qu'ils ont formulées. À cet égard la transférabilité externe des contrats d'assurance-vie apparaît comme le point faisant l'objet du plus important débat. Pour s'y opposer. Évidemment, les banques et assurances mettent en avant un risque prudentiel et systémique. Ce qui n'a rien d'étonnant venant d'elle. Pour autant, comme l'ont précisé les rapporteurs. Elles n'ont rien pu prouver avec des simulations et des chiffres. Nous sommes d'ailleurs preneur. Ici, la représentation nationale, Monsieur le Ministre. Nous sommes preneurs de ces chiffres et puis évidemment si Bercy pouvait nous en fournir serions bien heureux. Alors Monsieur le Ministre, nous aimerions tout simplement savoir si vos services sont en mesure d'éclairer le débat sur ce point, je vous remercie de votre écoute. Merci cher collègue. Cela clôt la discussion générale. Et nous passons à la discussion du. Texte de la commission et nous commençons avant l'article 1er. Un article additionnel fait l'objet de l'amendement 35. Monsieur Savoldelli vous pouvez le défendent l'amendement 35. Monsieur le président. Je vais même vous faire une bonne proposition. Je vais vous proposer défendent les deux en même temps ça vous va ça. alors adopté. Ouais ça serait bien, mais ça ne sera peut-être pas le cas. Donc monsieur le président, monsieur le rapporteur général mes, mes chers collègues vous porter l'ambition je cite de renforcer la protection des épargnants. Mais là aucune disposition de ce texte ne concerne les livrets réglementés. Pourtant 87 millions de livrets de ce type sont ouverts pour un encours total de 846 milliards d'euros. Vous les connaissez tous hein. Le Livret A, le livret de développement le le LEP et Et pour vous en convaincre. Je vous lis un extrait des observations de la Cour des comptes. Je cite bénéficiant de la part de l'état d'une garantie sur le capital et d'une rémunération évoluant en fonction de l'inflation. Pour le système financier. Elle constitue une ressource stable et contribue à transformer les dépôts des épargnants en emplois d'intérêt général de long terme, fin de citation de la Cour des comptes. Ces deux amendements propose d'élargir les bénéficiaires du livret d'épargne populaire et de rendre sa présentation obligatoire aux épargnants éligible. Il est emblématique de ce qu'est un produit d'épargne protecteur c'est-à-dire rémunérateur car indexés sur l'inflation sécurisant par des dépôts garantis liquide et avec une fiscalité avantageuse. Alors que les clients les plus aisés bénéficient de remises commerciales, ce qu'on appelle des ex-tourne et des supports défiscaliser les clients les plus modestes subissent la double peine, plus de frais et une épargne moins ruiné artiste pourtant comme pour les aides sociales le non recours au livret d'épargne populaire et massif. L'Observatoire de l'épargne réglementée a établi son rapport. 21% des individus éligible détiennent à et le P. alors que les personnes éligibles non détentrice du livret d'épargne populaire la moitié détient un livret A pourtant moins rémunérateurs. Donc l'ambition de ces deux amendements devrait devrait devrait être de rester de populariser les produits d'épargne réellement populaire est réellement utiles à l'intérêt général. Merci de votre attention.

Je vais être appelé aussi ce que ça représente par personne l'encours moyen l'assurance vie c'est autour de 30.000 euros donc ça concerne évidemment des millions de Français et pas uniquement les plus riches et avec. À peu près 12.000 euros pour l'PER donc voilà dans les enjeux. Donc ça concerne notre position loi ne s'adresse pas qu'elle est pas des plus aisées. C'est ça concerne les pertes de l'ensemble des Français. Alors c'est vrai que sur le livret d'épargne populaire et c'est l'objet de de ces deux amendements notamment le premier le 35 qui vise à élargir. La possibilité de diffusion. Il y a un sujet puisqu'il y a 18 millions. De Français qui sont éligibles au livret d'épargne populaire. Mais la réalité c'est qu'il y en a que seulement 8.500.000 qui souscrivent alors. Le, le sujet est réel et l'enjeu plutôt je réponds entre également à l'article l'amendement 34. L'enjeu, plutôt que d'augmenter les plafonds c'est peut-être de mieux diffuser ce livret d'épargne populaire. Alors il y a je crois une information qui est donnée par la DGFIP chaque année. La direction générale des finances publiques. Je ne sais pas comment elle pourrait être mieux diffuser peut-être être sur l'avis d'imposition, elle regarde simplement. Si on est éligible est à l'épargne populaire ou les le P. et les l'administration fiscale, la DGFIP est censé informer le contribuable. De son éligibilité à l'épargne populaire. Faut-il aller au-delà qu'me repose l'amendement 35, ça peut à mon sens poser hein ça me difficultés notamment la question de la confidentialité des informations. Ça veut dire que c'est le banquier, c'est la banque qui devrait aller regarder. Les prestations sociales, les revenus donc avec un problème de peut-être de secret et. À mon sens, il vaut mieux en rester au dispositif existant, c'est-à-dire

Donc si tu demande de retrait et peu de se peut-être que pourra nous donner sans doute peut-être d'autres pistes pour a notamment sur l'avis d'imposition, mieux informer les contribuables sur le deuxième homme. Moment élargir

Monsieur le Ministre. Et bien gouvernement sur ces deux amendements. Merci monsieur le le président mais non j'aurais pas de meilleur argument que. Que ceux déployés par par le le rapport le rapporteur, si ce n'est pour dire que. La campagne la 3ème campagne d'information sera lancée dans les semaines qui viennent. Suite à l'augmentation du taux, que les précédentes campagnes ont porté leurs fruits puisque celle de l'année dernière a conduit 1,3 millions de de de Français éligibles au au LEP à à y souscrire permettant de de réduire un petit peu le, l'écart entre comme l'a rappelé le rapporteur. C'est des ceux qui sont éligibles et ceux qui ont déjà souscrit ce produit qui est effectivement destiné. Aux Français les plus modestes, donc une demande de retrait et à défaut un avis défavorable.

Moi je vous dis très simplement en en a vous accepterait pas ces amendements. Mais je veux rappeler quand même qu'ils avaient qu'une vocation c'est favoriser l'épargne populaire. Et l'intérêt général et et Albéric de Montgolfier. Vous, vous parlez des banques. Je pense tout le monde a fait la même expérience autour de lui la même que moi pour plus qu'un autre. J'ai beaucoup de gens. Notamment c'est des retraités qui sont appelés par les banques. Pour leur dire qu'ils ont atteint le plafond. Pour leur faire prendre un autre produit. Et beaucoup dans les banques. Provoque un un mensonge pour obtenir d'autres ouvertures. En disant aux gens, vous avez éteint le plafond il faut passer à autre chose, sauf que vous le savez tous, ici, j'ai des gens que vous avez rencontré comme moi c'est les intérêts qui les ont amenés à dépasser le plafond. Donc c'est pour ça qu'à un moment législateur aussi, je pense qu'il a une responsabilité sans être intrusif mais faut quand même qu'il joue son rôle pour encourager l'épargne populaire. Voilà donc si on vote pas ces amendements, c'est quand même au final on ne veut pas encourager les l'épargne populaire, merci.

L'abstention n'est pas adopté ces même sur le 34. Même vote. Nous passons à l'article 1er nous avons premier amendement un amendement de.

fait un travail utile. Depuis 2020, en insistant sur le caractère un peu spécifique, un peu incongru, des commissions de mouvement commissions de mouvement, je le rappelle ce sont les commissions que les gestionnaires perçoivent en vendant et en achetant des actions et évidemment, plus on fait tourner un portefeuille par définition plus on touche des commissions de mouvement c'est parfois dans l'intérêt de l'épargnant, mais pas toujours. On peut comprendre qu'un certain nombre de gestionnaires soient tentés de multiplier ces mouvements qui génère des commissions et donc c'est la raison pour laquelle on avait beaucoup insisté c'est la commission là les commissions. Le mode de rémunération, c'était la commission Irène scandaleux en soi. Tout travail mérite salaire. En revanche, ces commissions ne sont pas forcément justifiées. Encore une fois, par l'intérêt de l'épargnant. Et c'est la raison pour laquelle nous avions dès le début proposé de les de les supprimer assisté. Je crois que notre assistance apportée puisque le règlement général de l'AMF prévoit à partir du 1er janvier 2026. Faut attendez adaptation l'interdiction totale des commissions de mouvement donc on va pas. Rajouter une disposition qui est me semble-t-il satisfait et dans un souci de simplification et d'éviter peut-être une loi trop bavarde. Nous proposons la suppression de l'article premier donc satisfaits par la modification du règlement général de l'AMF qui interdit ces commissions. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le le président. Je salue l'esprit constructif des rapporteurs. C'est un avis favorable pour cet amendement. Ah. Demandes de paroles donc voit cet amendement de suppression qui est pour. Qui est pour. Voilà. Contre. Il est adopté, il fait tomber les autres et donc la l'article 1er est supprimé après l'article 1er.

Comme Monsieur Calvez. On a déjà fait la promotion, je serais rapide sur présentation de de cet amendement qui vise à encadrer, enfin les frais sur les comptes bancaires de personnes décédées qui aujourd'hui sont souvent très élevées, quand bien même. Les opérations pour des personnes vivantes sont sont gratuites et des des opérations équivalente. Ils sont opaques et ils sont très hétérogènes et donc j'avais déjà interpellé le gouvernement sur ce sujet le ministre de l'Économie m'avait répondu dans une question écrite il y a 2 ans que tout ça allait se régler que des mesures allaient être prises et malheureusement on en est toujours au même point et c'est pour ça que j'ai proposé cet amendement qui reprend en grande partie la proposition de loi que j'ai commise. L'année dernière et qui vous propose donc il y a une gratuité des des frais bancaires pour les comptes dans le inférieur à 5000 euros et de là ces frais soit plafonné à 1% du compte dans la limite d'un montant fixé par un arrêté ministériel. M. Paoli-Gagin. Il est défendu, monsieur le président. C'est exactement le même. Monsieur le rapporteur. qui montrait d'une part une très grande hétérogénéité de de frais parfois des niveaux assez élevés et notamment pour la succession, les plus modestes et on a, on va beaucoup parler de concurrence, notamment à travers la transférabilité sur. Dans ah externe là malheureusement lorsque survient un décès, il y a pas de me citer de mettre en concurrence les la banque vous imposer unilatéralement des frais qui peuvent être très élevé pour des petites successions et donc c'est la raison pour laquelle à travers ce dispositif d'encadrement je crois ce qu'on remédie à situation qui est

monsieur le président. Le gouvernement partage le le sentiment la légitime d'injustice que. Les frais bancaires de succession peut faire naître dans certaines situations qui touche nos concitoyens Dans un moment particulier et profondément intime de leur vie. C'est la raison pour laquelle. Le gouvernement suite. Oh diverses interpellations qui lui ont été adressées à souhaité trouver la solution la plus efficace possible et c'est pour cela qu'une démarche de négociation d'un accord de place engageant pleinement les banques. Au-delà des des exigences légales est en cours. C'est cette même démarche qui avait été engagé pour plafonner les les frais pour les publics fragiles en 2019 et qui a porté ses ses fruits qui s'est montré efficace en reposant sur un engagement volontaire de de chaque banque. Cette méthode a pu prévenir tout risque de contournement du du cadre législatif que à l'époque, nous aurions pu mettre en oeuvre. Dans cet esprit, le gouvernement réunira les banques en février afin de finaliser les travaux avant le passage en séance de cette proposition de loi et je vous propose, monsieur le sénateur. Si vous retiriez votre amendement. Que à cette occasion là vous puissiez contribuer aux travaux. J'ajoute que sur le le fond de l'amendement. Ce que nous espérons c'est de parvenir à un accord de place. Sur lequel les le le plafonnement des frais puisse être inférieure à 1% des sommes du compte qui pourrait très vite représenter des frais bien plus importants que ceux aujourd'hui pratiqués.

donc il y a pas besoin de de temps de parole pour ça. Madame Goulet a demandé la parole, avant qu'on vote. Oui, monsieur le président, Monsieur le millésime, chers collègues, nous on va voter cet amendement et Monsieur le Ministre, ça va vous aider à négocier. Voilà donc je pense que c'est un amendement de bon sens on va le voter et puis ça vous aidera comme je viens de le dire à à négocier exactement dans le même sens. Pardon de dire vous dites nous partageons. Nous sommes d'accord avec tout, enfin on vous demande de le retirer. Sincèrement, à un moment il faut que le débat parlementaire ait du sens. Si vous dites que vous voyez les banques en février. Ben vous avez le soutien du Sénat pour amplifier vos négociations avec les banques vous devriez au contraire dit que non seulement vous êtes favorable mais que vous regrettez de ne pas l'avoir vous-même présenté. Expliquer son vote.

aurait cette position parce que nous dire attendez attendez on, on, ça va se régler tout seul, c'est ce qu'on me dit et ce qu'on m'écrit depuis maintenant. 2 ans Le le pardon. La réponse du gouvernement dans une question écrite c'était le gouvernement demeure à ce titre, déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagés en février 2021 et ensuite j'ai eu un courrier un courrier de Bruno Lemaire. Ben disons que tout ça serait réglé d'ici le début de l'Automne 2022. Donc permettez-moi, Monsieur le Ministre de penser qu'il faut peut-être que l'on légifère et comme l'on dit, mais mes collègues ça ne pourra qu'être utile à à au gouvernement s'il veut arriver à un accord encore meilleur que ce qu'on propose aujourd'hui. Alors. Monsieur le Ministre. de la profession bancaire, sur la base d'un accord de place et si aujourd'hui 4 millions de Français peuvent bénéficier d'une offre qui limite les frais d'incident bancaire à 25 euros par mois et pour certains d'entre eux à 20 euros par mois et à 200 euros par an. C'est sur le fondement d'un accord de place et sans qu'aucun ne un amendement n'a été. Adopté auparavant. C'est vous dire notre détermination à faire. À faire converger les choses et à obtenir que dans ce type de situation, un plafonnement puisse se trouver qui sera, je l'ai dit, nous l'espérons en tout cas inférieur à 1%. Merci, monsieur le Président notre groupe votera cet amendement. Enfin faut prendre, faut, faut pas être dans la démesure. On on parle des frais. Bancaires sur la clôture d'un compte de moins de 5000 euros en cas de succession. quelle est la valeur de ces frais. Franchement. Non là là vraiment quand on voit les échelles des chiffre qu'on a, dont on a parlé auparavant dans notre diversité ici dans l'hémicycle. C'est un amendement responsable. Donc nous nous le voterons. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le sénateur, je vous rappelle que ce plafonnement va concerner également les les très hauts patrimoines que vous dénonciez tout à l'heure à la à la tribune, c'est, c'est votre. Droit que de défendent le plafonnement des frais pour ce type de public mais vous l'assumerai. On doit pouvoir voter calmement sur ce sujet qui est pour ces amendements. Bon ça va vite, qui est contre. Il y a pas d'abstention. Ils sont adoptés. Nous arrivons à l'article de et tout ça va bien se passer. Le gouvernement a quelques amendements. C'est le gouvernement qui commence avec le 31 puis le 45 mais un par si vous voulez bien. Allez le ministre l'amendement 31, en quelques mots. Merci Monsieur le Président c'est un amendement qui prévoit plusieurs modifications pour clarifier le le Champ d'application de l'article en 1er lieu la gestion pilotée par horizon du plan d'épargne retraite est exclu d'une partie du Champ d'application du dispositif dans la mesure où ce mode de gestion définis par voie législative et réglementaire prévoit déjà une sécurisation progressive de l'épargne à l'approche de la date de liquidation du contrat. Le 2ème point. Il s'agit de préserver le cas des mandats dits familiaux ou la gestion de l'épargne a confié est confié à un proche et il est précisé que cet encadrement ne concerne que les mandataires agissant dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnel. En dernier lieu, c'est le 3ème point les opérations ponctuelles déterminé lors de la souscription de l'adhésion, qui ne s'apparente pas un mode de gestion habituel du contrat sont exclus du Champ d'application de cet article. Favorable. Je le mets aux voix qui est pour. Compte. Il est adopté. Nous passons 45 mêmes process le plus le gouvernement le défend. Merci monsieur le président. l'interdiction des rémunérations différenciées en fonction des supports dans le cadre du mandat d'arbitrage se traduirait par une interdiction des rétrocessions telles qu'elles sont conçues aujourd'hui si un plus grand encadrement de certaines rétrocessions est nécessaire. Celui-ci doit faire l'objet d'un examen approfondi et d'une étude d'impact exhaustive vu les implications potentielles sur le modèle de distribution français qui offre une gratuité du conseil et une accessibilité des ménages à l'épargne financière depuis un large réseau d'agences. Bien l'avis de la commission. Favorable, favorable également donc on revote qui est pour. Contre. L'abstention, il est adopté et enfin le 32. Monsieur le ministre. Un amendement du gouvernement numéro Vous avez un petit tableau qui vous permet de voir arriver les amendements avant que je les appelle. le ce 3ème amendement a pour objet de permettre aux prestataires de services d'investissement des délégataires d'opérations relevant du mandat sous le contrôle du mandataire, les prestataires de services d'investissement pour ainsi plus aisément faire bénéficier les épargnants de leur expertise en matière d'allocations de portefeuilles tout Enak encadrant les pratiques de délégation.

donc ce sera David sagesse pour s'assurer vraiment de cette compatibilité. Entendu. Donc à mon. Le ministre d'ajouter une précision. Oui pour peut être apporter un complément de réponse. Cette évolution est pleinement compatible avec le droit de l'Union européenne et permet simplement de limiter les effets de l'encadrement des mandats sur les pratiques d'un marché où les prestataires de services d'investissement interviennent déjà. Vous maintenez votre avis de sagesse. Donc, amendement du gouvernement avec avis de sagesse de la commission qui est pour. y a-t-il des contre. L'abstention. Il est donc adopté nous votons maintenant sur l'article de ainsi. Qui est pour. pour. Abstention, et l'article de ainsi modifié est adopté sur le trois, nous avons un amendement 24 du gouvernement. Oui, monsieur le président. Un amendement qui supprime la référence au fonds de fonds indiciel de la Caisse des dépôts et et. Qui est prévue à l'article 9. sommes le gouvernement est opposé à la création de cette. De ce fonds de fonds indiciels et et par conséquent propose de le retirer de cet article. 3. Monsieur le rapporteur. Un avis défavorable puisque c'est contraire à l'avis de la commission. D'accord donc. Un amendement du gouvernement avec avis défavorable de la commission je consulte le Sénat qui est pour. pour. Entre. Plus qui s'abstient. Donc il n'est pas adopté, je passe au vote sur le trois non modifié, qui est pour l'article 3.

merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre ce Monsieur le président de la commission des finances. Messieurs les rapporteurs chers collègues concernant cet article 4. Qui vise au renforcement de la transparence sur les frais attachés aux produits d'assurance vie et d'épargne retraite, il s'inscrit. Dans le chapitre 2 qui est consacré au thème, permettre à l'épargnant de faire un choix plus éclairé des 2 rapporteur Jean-François Husson, Albéric de Montgolfier rapport d'octobre 2021 et qui concerne bien entendu les enjeux financiers. Particulièrement important pour les ménages, comme pour le financement de l'économie en rappelant, selon le rapport des de nos deux rapporteurs, l'encours des placements des ménages ont valeur de marché au 2ème trimestre 2022 s'élève 5727 milliards d'euros. Cet article 4 qui fait référence également à la loi pacte concernant le renforcement de la transparence des frais. Ceux qui Qui a été aussi largement développé par le rapporteur et et nos collègues qui sont intervenus. Rôle de suivi. Au qu'au comité consultatif du secteur financier. Concernant le suivi des pratiques tarifaires de. Différents produits. Financiers et enfin aussi également renforcer l'information sur les frais qui sont accessibles aux épargnants. À toutes. Les étapes et y compris également pour les contrats conclus auprès des ou. Auprès des mutuelles voilà con donc je soutiendrai également cet article IV merci. Alors sur cet article que nous avons l'amendement 33 présenté par Monsieur Maurer qui a la parole. j'ai j'ai zappé le 49 qui est un amendement de rectification rédactionnelle du rapporteur. Avis favorable du gouvernement donc je consulte sur cet amendement rédactionnel qui est pour.

Monsieur le rapporteur. Mes, mes chers collègues. Cet amendement vise à améliorer l'information et la transparence sur les produits d'assurance-vie et de capitalisation. La loi pacte a déjà prévu la publication d'un certain nombre d'informations mais, aujourd'hui, de toute évidence, cela n'est pas suffisant et donc cet, cet amendement vient compléter la rédaction de l'article IV en proposant des informations complémentaires, la communication d'informations complémentaires et en prévoyant également que un, un arrêté du ministre de l'Économie viendra prévoir les modalités de publication de ces informations de telle sorte à ce qu'il y a une, une espèce de de normalisation des informations et d'homogénéité, parce qu'aujourd'hui j'invite mes collègues à faire l'exercice. Quand on va sur des sites qu'on essaie de comparer tel ou tel produit. C'est tout juste impossible parce que les données sont parfois impossibles à trouver ou qu'elles sont présentées de manière extrêmement différente d'un d'un produit à l'autre Cet amendement vise à y remédier. Qui est l'avis de la commission. Favorable, le gouvernement. C'est une demande. De retrait à défaut défavorable car l'équilibre qui avait été trouvé en commission. Nous paraît. comme le disait le sénateur c'est loin tout à l'heure, il convient de ne pas noyer l'épargnant sous une somme d'informations sans quoi on perd le bénéfice de la mise en transparence de ces informations et donc on souhaite le gouvernement souhaiterait qu'on puisse rester sur la rédaction de la commission. Donc nous avons un avis favorable de la commission est défavorable vous demande de retrait du gouvernement. Monsieur Moret. En forme de boutade mais peut-être pas tout à fait au ministre que je vais finir par penser comme monsieur Savoldelli qu'il est là uniquement pour défendre les sociétés d'assurance et les établissements bancaires parce que là encore on a un amendement qui est destinée à apporter plus de de lisibilité. Plus de transparence et nous explique que c'est que c'est pas bien, donc c'est assez, c'est assez surprenant. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur ni Bruno Lemaire ni moi-même ne ne ne pouvant être soupçonné de servir les intérêts des assureurs. Regardez, regardez le contenu de la loi pas qu'aujourd'hui vous avez vous vous venez augmenté d'un certain nombre de propositions complémentaires. C'est une loi qui a été adopté il y a 4 ans et dont Bruno Lemaire été l'artisan et dont j'ai été moi-même le le rapporteur pour sa dimension financière. Il nous nous sommes posés ces questions là pendant dans le cadre de la loi pacte et nous sommes venus à la même conclusion qu'il convient effectivement de mettre l'information en transparence pour permettre à l'épargnant de naviguer et de faire son choix en pleine connaissance de cause, mais que si vous donnez à l'épargnant. Trop d'informations en même temps vous perdez le bénéfice de cette transparence. Monsieur le Ministre, je vous comprends pas, vous vous venez dire quasiment à l'instant. Si on donne trop d'informations pour participer à la transparence et à la connaissance des produits, on perd. On perd le bénéficiaire l'assuré enfin je suis désolé, les bras m'en tombent. on s'est tous mobilisés dans le cadre de la discussion du projet de loi pacte. La question n'est pas de savoir si c'est Bruno Lemaire, si c'est vous. Si c'est nous, c'est pas le sujet, le sujet on veut mieux protéger les épargnants et donner la transparence de l'information. Vous savez ici, on est un certain nombre à penser que plus on gagnera en compréhension et en connaissance des mécanismes de l'épargne et de l'économie, plus on amènera les Français à adhérer et à épargner. C'est le seul objectif comprenez-le. Je pense qu'il faut sortir d'une forme de posture qui vous met un peu en décalage dans en ce début de débat.

une fois n'est pas coutume. Monsieur le rapporteur général, mais là je, j'avoue que je bloque sur le sujet parce que. On a tous à peu près un contrat d'assurance-vie avec des unités de compte et on dit de recevoir le rapport annuel et ça représente 12 pages. 12 pages d'informations, il y a eu un test qui a été fait. C'est grosso modo 12% d'assurés qui regarde ces 12 pages. Donc. Franchement, on arrive à un moment un degré d'administration d'administratif

Le Sénat a donc vu l'avis favorable du gouverneur de la commission sur cet amendement est l'avis défavorable à défaut de retrait du gouvernement ne pouvons nous prononcer qui est pour cet amendement. Qui est contre. Y a-t-il ou abstention. Adopté ensuite nous avons un amendement 50 du rapporteur. Qui a la parole. Oui qui vise simplement donc Retenir les mêmes dispositifs. De la compétence du CCSF pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et à Y a-t-il des contre. À l'abstention, il est adopté. Et nous avons un amendement rédactionnel. 51. Même avis du gouvernement qui est pour cet amendement. Une double avis favorable. Contre. Abstention. Il est adopté. Donc sur l'article quatre avec ces modifications. Qui est pour l'article IV. Qui est contre. Ah l'abstention il article IV est ainsi adopté après l'article IV. Nous avons un amendement

à l'épargnant. Ce sera Sam sans. Un grand nombre de pages. Il faut rechercher la simplicité et que l'épargnant puisse réellement appréhender la réalité des coûts qui le supporte. Qu'est l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Le ministre.

qui est évoqué dans le l'amendement de Monsieur Kenneth est une instance de coordination de ces 2 autorités qui n'a pas la capacité de, de contrôler les obligations pesant sur les entreprises. L'amendement 3 donc une compétence au pôle commun, bien au-delà de ce pourquoi il est pensé et qui ne sera pas en capacité d'honorer. Pas de retrait. Donc. Je mets aux voix cet amendement qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission et d'un avis défavorable à défaut de retrait du gouvernement qui est pour.

de ce que je pourrais appeler moi de dévoiement de l'Avantage fiscal qui est dévolu au plan d'épargne en actions. D'ailleurs, vous l'écrivez vous-même dans votre rapport. Je cite jusqu'au début des années 2000 le et son avantage fiscal était quasi intégralement réservé au financement de l'économie française soit on à l'action d'actions cotées en France. Et aujourd'hui 75% des titres ne doivent plus provenir de France. Mais de l'Union européenne ou d'un état de l'Espace économique européen. Donnera un exemple. Pas très probant. C'est par exemple ça peut venir du Liechtenstein par exemple par exemple. Ce même pays que le juge Renaud Van Ruymbeck considère comme un exemple parfait de l'évasion fiscale au coeur de l'Europe. Friands de sociétés offshore. Je crois que ce sujet connu quand même par tous les collègues de l'hémicycle. En 92, à la création du PEA. Les seules actions cotées admise était celle émise par les établissements de crédit appartenant au secteur mutualiste et coopératif, Crédit Mutuel, Banque Populaire Caisse régionale du Crédit agricole notamment aujourd'hui, c'est un produit d'épargne qui est capté par les grandes entreprises cotées et d'après les données collectées par le CSA pour l'AMF. Plus de 60% des supports détenues au sein d'un PA ou d'un compte titres seraient des actions des 120 plus grandes s'entreprise française. Donc qu'est-ce qu'qui a quoi on parle on irait à créer un droit à l'erreur. Qui s'apparente à un droit à la fraude pour des titres inéligible interro portefeuille alors que les possibilités d'investissement sont extrêmement larges. Donc la rédaction de ce qui sort de la Commission nous semble exonérer de toute responsabilité. Ce qu'on appelle le gestionnaire de plan. Donc un ciblage sur les revenus déjà élevé et le produit proposé procède donc d'un ciblage très étroit en termes de définition des bénéficiaires potentiels qui discute pas les comportements spéculatifs. Je vous cite, ceux de votre famille politique ces mots date de 1992 mais il nous semble toujours d'actualité. Aujourd'hui, 70 pour 177 pour des PO a ouvert, ont fait l'objet de versement de moins de 15.000 euros, soit 10 fois inférieur au plafond. Alors qu'est l'avis de la commission sur cet amendement de suppression monsieur rapporteur général. Une possibilité d'améliorer le dispositif autour du PA. On l'a évoqué d'ailleurs y compris dans les échanges en commission. C'est je dirais, c'est l'objet même éventuellement sur ce sujet de la navette donc un avis défavorable. L'avis du gouvernement. C'est un avis favorable sur sur le sur l'amendement. Considérant que, même si le travail doit se poursuivent pour améliorer le fonctionnement du PEA et du PEA PME que la la la la mesure proposée dans l'article 5 n'est pas souhaitable en l'état. donc. Nous avons à nous prononcer sur un amendement. De monsieur Savoldelli objet dans la ville défavorable de la commission est favorable du gouvernement qui est pour.

5. Abstention. Une est adopté. Il y a ensuite un 5 bis sur lequel il n'y a pas de d'amendements. Qui est pour l'article 5 bis. Et contre. Qui s'abstient. Il était adopté. Après l'article 5 bis. Nous avons un article additionnel qui est un amendement 52 Dieu monsieur de Montgolfier. qui, qui propose en fait sur des. Fins de vie de fonds de capital-investissement de passer non pas. La fin de vie à 10 ans mais à 15 ans parce que dans certains cas, on s'aperçoit que, et on le cite notamment les biotechs. On a besoin. De davantage de temps pour retrouver de la rentabilité. Y a-t-il des contrats. On ne voit pas à l'abstention, il était adopté l'article 6 a été supprimée en commission. Ensuite nous avons un article. Additionnel. 2 amendements identiques, le 1er et les posée par monsieur Bachere qui a la parole à ballon. Allez-y, chers collègues, monsieur. La rédaction actuelle des activités susceptibles d'être reconnus d'utilité sociale n'évoque pas explicitement la préservation du Patrimoine naturel et historique. Chacun sait le rôle que ce Patrimoine joue dans l'attractivité de la France et particulièrement pour le tourisme. Sa valeur historique et culturelle. Son impact économique ne sont plus à démontrer. Le sites naturels et historiques constituent également des espaces protégés propice à la biodiversité largement répartis dans toute la France. Il joue un rôle important. Dans l'attractivité des territoires ruraux. Faute de rentabilité. La préservation du Patrimoine et peu propice au développement d'une activité de marché. Son insertion dans l'économie sociale et solidaire permettrait l'émergence d'acteurs qui la prendrait en charge dans le cadre de la lucrative IT limiter évidemment de C'est pourquoi il convient donc d'ajouter la préservation du Patrimoine à l'énumération de l'article 2 de la loi, donc de l'économie sociale et solidaire qui est également reprise à l'article 3332 tiré 17 tirer un du code du travail. Monsieur Blin vous descendez le même amendement. à l'essentiel, l'amendement est défendu. Néanmoins, je voudrais insister sur l'évidence qu'il y a à considérer. Les activités immobilières des foncières patrimonial comme une activité. D'utilité sociale. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons leur faire bénéficier des avantages prévus pour ses us. Et donc les les intégrer formellement à ce à ce dispositif est. Supprimée la dérogation qui existe de façon générale pour les activités immobilières concernant les dispositifs d'investissement dans les PME et permettre à ce que cette activité qui s'intègre qui dans l'économie de marché puisse être soutenue, compte tenu de son utilité culturelle et et patrimonial. Qui est l'avis de la commission monsieur avis. Un avis favorable. Je voudrais d'abord dire que. C'est une finalement c'est une ouverture supplémentaire. En direction des des entreprises d'ailleurs. Donc je rappelle qu'elles sont eux aussi agréé par le ministère de la culture et qu'elles ont pour objectif de mettre en valeur le Patrimoine bâti mais pas seulement le Patrimoine naturel, et je pense que le fait de proposer cette ouverture sur des dispositifs. Qui sont. Finalement. Non lucratif enfin des, pour les entreprises à but non lucratif, c'est aussi un élément particulièrement important et intéressant, qui s'inscrit dans la droite ligne d'un certain nombre d'avancées que nous avons soutenu au travers des précédents débats budgétaires. monsieur le président. Le gouvernement partage l'objectif de soutenir. La la la la restauration et l'entretien du Patrimoine culturel, il soutient l'idée selon laquelle 10 ans après sa création, il convient de faire un bilan et peut-être de faire évoluer dispositif et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il remettra comme le comme il comme le Parlement lui a demandé un, un rapport sur le dispositif et ZUS. Au mois de septembre 2023. Il est donc trop tôt, sans doute pour. Légiférer dès aujourd'hui sachant qu'il existe. D'autres dispositifs identifié de soutien à la restauration du du Patrimoine comme le le dispositif Malraux par exemple mais que, qu'en tout cas s'agissant de la réforme du dispositif ASUS, il convient d'attendre son évaluation qui va donc intervenir 10 ans après sa création. Donc, avis défavorable. Donc. Nous avons 2 amendements identiques, objet d'un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement. Je les mets aux voix qui est pour. Qui est contre maintenant. Y a-t-il abstention donc ils sont adoptés. Nous passons de l'article 7. Et nous commençons par un amendement de suppression numéro 21 de monsieur Savoldelli. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mais mes chers collègues. Notre groupe considère que c'est un Arctique. Qui pour nous est une fausse bonne idée. Alors évidemment quand il s'agit de permettre à l'épargnant de renforcer sa capacité à décider sur la base d'informations rationnelles et transparentes. Quel distributeur d'sur 11 villes choisies sur la base de ces informations, il pourrait privilégier un autre assureur en conservant le bénéfice fiscal. La durée de conservation mais pourrait être rattrapé en quelque sorte par une offre alléchante de sa compagnie d'assurance actuel. En, en somme, vous allez me dire franchement ça vaut le Savoldelli. Vous pouvez pas contre une concurrence saine dans un marché sans voilà sauf que moi je vous dis, c'est que vous considérez dans cet article que l'épargne est un marché comme les autres et là il y a problème de de de de penser. Ça m'évoque une citation de Paul Valéry, quand on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, on dit rien car les mêmes choses ne se reproduise jamais. Et d'ailleurs on ne peut jamais connaître toutes les causes. La loi pacte la assurance emprunteur dans une certaine mesure la PPL courtage en assurance. À chaque fois une réponse. Libérer le marché de ces entraves en octroyant les droits aux consommateurs supposée éclairer. Sauf si c'est l'angle mort de cette proposition de loi strictement focalisées sur l'épargnant enfin l'épargnant assez aisée. Jamais vous ne considérez à quoi sert l'épargne et c'est ça, c'est une des questions d'ailleurs qui nous a amenés sur notre vote. L'épargne sert à quoi. L'épargne ne peut pas être considéré comme seulement et uniquement un Avantage fiscal. Ce support l'épargne doit être un support par rapport à des objectifs sociaux, économiques, écologiques et quand on voit tous les enjeux qu'on a devant nous et des problèmes de financement qu'on a il faut traiter cette question là et là bas cette captivité des épargnants n'est pas rattaché à un objectif, j'irai dire d'émancipation et au regard des des enjeux. C'est pourquoi nous pensons que cet article est toujours une fausse bonne idée. Et nous demandons la suppression de l'Arctique. D'une forme d'épargne. Non c'est pas tout à fait pareil qui est là le l'épargne assurantiel. Ce qui m'étonne, mais enfin au moins aujourd'hui. Alors qu'. Un certain nombre de Français manifestent dans la rue. notamment qui partage pour un certain nombre de vos idées. Je vois que vous êtes finalement avec France assureurs et Pascal Savoldelli, main dans la main pour un même combat. Honnêtement ça manque pas de sel. ça obéit exactement au même objectif. Or, or ce qui est important. Là c'est de permettre finalement à l'épargnant une de 2 éléments. Le 1er de recouvrer une liberté.

Avec un consentement évidemment éclairé choisir d'autres solutions. J'ai pris l'exemple tout à l'heure effectivement de on va l'appeler d'une épargne assurantiel Verdi. Mais. Vous le savez très bien, il y a une dizaine d'années on nous on nous promettait le paradis avec l'assurance vie heureux croissance échec. 4 ans plus tard, on nous a dit c'est le 2ème temps ça va être magique, échec. Heureusement que lui qui a eu d'autres solutions parce que sinon vous êtes avec une formule complètement prisonnier. Donc l'idée c'est de redonner de la capacité de la fluidité et de comment dirais-je, de libérer un peu le marché. Alors rassurez-vous Monsieur le Ministre. Christine Lavarde à juste raison a donné. Le petit montant. Au regard du montant très important. Et je parle de petits montants, qui a fait l'objet de transférabilité interne. Nous n'avons pas ici vocation je crois personne à vouloir déstabiliser le marché, l'économie française, c'est pas notre objectif, notre objectif c'est de faciliter la capacité des Français. Ah non seulement épargné mais à changer de modèle et éventuellement de support c'est ça qui est important parce que c'est la manière de financer l'économie et c'est le plus important pour nous. Favorable, l'amendement de monsieur Savoldelli. D'accord. Monsieur le Ministre, c'est aussi votre avis. Je suis. Hé non Monsieur le Président, c'est un avis favorable à cet amendement. Pourquoi est-ce que. Je peux y aller. Pourquoi est-ce que les Français font confiance à l'assurance vie. Pourquoi est-ce qu'il préfère. Le ministre s'il vous plaît. Jusqu'à présent nous avions une séance courtoise. Pourquoi est-ce que les Français. on fait de l'assurance vie leur produit d'épargne préféré. Pourquoi est-ce qu'ils investissent dans l'assurance-vie. Plutôt que dans des fonds d'investissements classiques ou non de la détention directe d'actions. Pour 2 raisons principales, la première c'est que c'est un capital qui leur est garantie en tout cas s'agissant du fond euros et la 2ème c'est que contrairement aux fonds d'investissement. Monsieur Salvodelli n'a, n'a pas tout à fait tort, il y a. Dans les raisons pour lesquelles les Français apprécient l'assurance vie, un principe de mutualisation au travers du temps. Je m'explique. Monsieur Husson. Avait ouvre un contrat d'assurance-vie en 2010, à un moment où les taux d'intérêt sont relativement élevés. Monsieur de Montgolfier investi dans un contrat d'assurance-vie en 2020 au moment où les taux sont à zéro. Le principe de mutualisation et de partage dans l'assurance-vie fait que le contrat d'assurance vie va délivrer va offrir au second, celui qui est entré sur le marché au moment où les taux étaient à 0, une moyenne entre les taux élevés et les taux à 0, si bien que nous allons partager avec celles et ceux qui investissent à nos côtés dans le même contrat d'assurance vie auprès du même assureur hé bien le même taux, quel que soit le moment où nous sommes entrés dans le contrat, c'est ce qui fait que les taux de rendement des contrats d'assurance vie ne varie pas aussi brutalement que les taux mais permet une forme d'assurance au travers du temps qu'on aura un rendement à peu près décent. Et la transférabilité externe. De de l'assurance vie. Elle est mauvaise pour les épargnants. Elle est mauvaise pour l'économie française et surtout elle est injuste. Elle est mauvaise pour l'économie parce que si la transférabilité. Fonctionne alors les épargnants et c'est normal changeront plus souvent d'assureurs s'ils changent plus souvent d'assureur. Cela veut dire que la durée d'investissement, ce qu'on dit la duration dans le jargon va se rétrécir pour l'assureur et donc l'assureur aura une capacité moins grande à investir dans la transition écologique investir au capital des entreprises et Donc moins de financement de l'économie française et moins de rendement en moyenne pour les assurés. Mais la transférabilité externe, elle est surtout injuste. Elle est injuste parce que si vous ouvrez la transférabilité externe de l'assurance vie. Si vous permettez à monsieur Husson est à monsieur de Montgolfier de sortir de l'eau. Contrat d'assurance-vie qui va le faire en premier qui sortira en premier de son contrat d'assurance vie pour aller chercher un contrat nouveau nouvellement offert par un autre assureur, parce que la période des taux est plus favorable avec des taux plus élevés, hé bien c'est celui des 2 qui a la meilleure connaissance financière c'est celui des 2 qui qui est probablement le plus sophistiqué et donc le plus aisée et qui restera. Dans le contrat d'assurance vie moins favorable que celui qui vient d'être créée sur le marché. Hé bien, celui des 2 qui est un peu moins sophistiqués et vous voyez que je n'en homme, aucun des deux. Que c'est celui qui est un peu moins sophistiqués et qui sans doute à une épargne moins importante et Et enfin. Je, je voudrais dire aussi que la transférabilité existent déjà. Grâce à cette proposition de loi la transférabilité interne sera désormais. De droit. Et ça c'est une. C'est une bonne chose, puisque effectivement il y a aujourd'hui des contrats d'assurance-vie relativement nouveau qui offrent des unités de compte verte. Si je suis rentré il y a 10 ans dans mon contrat d'assurance-vie qui n'offrait pas d'unités de compte verte je peux solliciter mon assureur. La loi pacte me le permettez mais mon assureur avait jusqu'à présent le droit de me dire non. Avec cette proposition de loi le transfert sera de droit. Mais si vous voulez-vous transférer votera sur votre contrat d'assurance-vie vers un autre assureur, c'est possible. Vous sortez vous rachetez votre contrat. Et vous entrez dans un nouveau en accumulant progressivement l'Avantage fiscal qui est la condition de cette mutualisation, à travers le temps qui fait que les épargnants au sein des contrats d'assurance-vie ça sur les uns les autres. Donc, avis favorable à l'amendement de suppression. Alors monsieur le rapporteur général. Juste pardon monsieur le Ministre, moi je on ne va pas faire de de vente. À domicile ou en agence. Il y a juste. Vous êtes mis en porte-à-faux. Alors là je vois France assureurs Pascal Savoldelli, Monsieur le Ministre. Donc c'est c'est une alliance. Tout à fait improbable mais surtout. En. Donnant un avis favorable à la suppression vous supprimez même la possibilité de la de la transférabilité interne. Alors je ne comprends plus rien. Le gouvernement est favorable à la transférabilité interne et aujourd'hui il est compte non mais honnêtement je pense que vous savez plus où vous habitez à cette heure-ci. Je rappelle que le disque. D'un amendement de suppression qui est préalables. Tous les autres amendements dont. Nous pouvons engager toute la discussion de l'article avec tous les amendements sur l'amendement de suppression c'est comme on veut. Madame Lavarde demande la parole Oui, j'ai écouté attentivement les explications magistrale du ministre et je voudrais lui poser de questions. Aujourd'hui, la loi ne m'interdit pas d'avoir de contrats d'assurance vie. Donc, si un des contrats est mauvais. Rien ne m'interdire de sortir mon argent pour aller l'investir dans un autre contrat donc autant dire que dans les faits c'est comme si je faisais de la transférabilité. Sauf que j'ai eu la possibilité à un moment d'ouvrir de contrats d'assurance-vie j'ai eu la possibilité de. Est ce que tous les Français peuvent ouvrir de contrats d'assurance-vie et comme j'ai eu la possibilité de l'ouvrir. Je me donne ensuite les moyens d'avoir une meilleure rentabilité d'aller vers un assureur peut être plus novateur qui pratique d'autres techniques. La personne qui n'a pas eu cette possibilité à un moment d'ouvrir de contrat elle elle reste point est lié son ancien son ancien assureur. Ça c'est ma première question, ma 2ème qu'seront il y a un certain type de contrat vous vous supposez que les contrats sont majoritairement investis en fonds euros et marginalement en unités de compte. Ça c'est tout votre raisonnement, mais quelqu'un qui a un contrat 100 pour en unité de compte, tout ce que vous venez de nous démontrer sur la mutualisation des taux ne tient pas donc pourquoi pour ce contrat-là on pourrait pas avoir une transférabilité. Voilà juste de questions que je vous pose à l'issue de votre argumentation. Nous nous prononçons sur l'amendement de Monsieur Savoldelli qui est un amendement de suppression du ministre. Et qui a donné lieu à un avis défavorable de la commission un avis favorable du gouvernement qui va compléter son appréciation. Oui simplement précisé qu'effectivement la vie sur l'amendement de Monsieur Salvodelli est défavorable car comme je l'ai dit à la tribune et comme je l'ai dit à l'instant, le gouvernement est évidemment favorable à la à la au renforcement de la transparence de s'agissant ensuite des réponses à Madame aux questions de madame Lavarde. C'est la, la transférabilité existe déjà ce que fait l'Avantage fiscal c'est qu'qui pousse l'épargnant ou il encourage l'épargnant à rester un peu plus longtemps dans le contrat d'assurance vie. À quoi cela sert-il à à réaliser cette mutualisation au travers du temps qui fait que on peut servir à l'épargnant une moyenne des taux et que. La la la rentabilité que vous tirez de votre contrat d'assurance-vie ne dépend pas. Du niveau des taux au moment, vous y êtes rentrés et s'agissant des des unités de compte alors. Les unités de compte sont effectivement moins concernée par le la la démonstration que je faisais tout à l'heure, vous avez néanmoins une plus grande latitude de choix et d'arbitrage entre les unités de compte proposer au sein du contrat du du du catalogue proposé par par par votre assureur, mais il convient de rappeler que une une une partie majoritaire du stock de l'assurance vie, même si les flux ont évolué ces dernières années et constitué du fonds euros c'est-à-dire de la dimension mutualisant de l'assurance. Je sais quoi. Explique son vol sur l'amendement de suppression. Oui, Monsieur le Ministre. La transférabilité, on parle d'une transférabilité au-delà de 8 ans. Donc ce que vous venez de démontrer sur la règle fiscale pour maintenir des contrats sur un long terme cette règle fiscale elle est elle est maintenue puisque on ne parle pas d'une transférabilité dès le premier dès la première année on parle seulement au bout de 8 ans, donc je ne vois pas quel est le problème. En plus il y a un 2ème point. Sur l'EPER. Les, les compagnies d'assurances étaient. Fermés sur le le la transférabilité des des À l'époque en disant il y a un risque systémique et cetera et cetera. Pourtant, l'EPR est devenu favorable puisque six vend si bien aujourd'hui c'est parce qu'on peut liquider sous forme de capital afin. Donc il y a intérêt de transformer les anciens contrats en nouveaux contrats et quand on fait le résultat quand on voit le résultat des transformations c'est seulement 10% des contrats et de l'épargne, qui ont été transférés sur le nouveau support. Donc vous voyez qu'on est vraiment loin du risque systémique, qui peut être décrit par l'ensemble des acteurs. Messieurs Savoldelli demandé la parole. Mais moi les ministres. Je débat des idées. Qu'il développe je les traite pas d'has been. Et s'agissant de nos collègues. Jamais. Je leur fais des remarques personnalisés, individualisés. Des fois on a des mots vifs. On a des des échanges. Passionnés mais toujours courtois et respectueux. Et on fait jamais des amalgames où il y a pas lieu d'en faire donc moi je vais vous redire très simplement, sur quoi vous allez voter. Peut être que je suis dans l'erreur et c'est le, le vote qui va décider. Mais moi je vous ai attirer votre attention sur la captivité des épargnants et par là même l'Avantage fiscal attaché qui sont quand même intrinsèque lié à la durée de détention. Longue a même pour l'assurance de placer les montants collectés par ces fonds et là où je m'interroge. Mais vous pouvez me dire que c'est une erreur. C'est qu'est-ce qu'il faut continuer à inciter à tout moment le client quel qu'il soit. peut-être que je suis un has been puisque je n'ai pas d'assurance vie. Vous pourrez vérifier. C'est de montrer aux clients qui puissent renforcer ses investissements en unité de compte sans garantie de capital et au détriment de la dette publique française. Vous voyez donc, on peut ne pas être d'accord mais c'est un amendement responsable. Voilà qui doit être traité avec. Par une contre-argumentation opposable mais avec respect. Parce que moi j'ai pas envie qu'un exode des épargnants français. Voilà. Et c'est pas franchouillard. Ces câbles a Croque il a des grands investisseurs il y a des fonds internationaux énorme qui peuvent nous capter des investissements des Français et des Françaises et qui empêche que s'asseoir injectés dans l'économie française. Vous voyez ça hein c'est c'est une voilà je pense un sujet responsable je m'excuse.

très rapidement, réponse à à monsieur le sénateur segments simplement dire que c'est 70% des contrats qui ont plus de de 8 ans et que l'EPER. Pour l'EPER. c'est intéressant parce que l'incitation fiscale est encore beaucoup plus forte que pour l'assurance-vie puisqu'elle vient dès l'année 2 versements et la raison pour laquelle on met une une incitation. Plus forte, c'est parce qu'on exige une durée de d'investissement encore plus longue que pour l'assurance-vie puisque c'est vrai qu'on peut sortir en capital mais au moment de la retraite, sauf cas particulier et que donc se justifie un Avantage fiscal très fort mais ça ça permet de valoriser le les abattements de l'assurance-vie comme une incitation à rester le plus longtemps possible dans le contrat. Bien monsieur le rapporteur, pardon messieurs. Besoin de faire une longue comparaison j'ai juste un élément pour Pascal Salvodelli à qui appartient l'épargne sur l'assurance-vie pas l'assureur. Elle appartient à l'assuré. Ouais mais son argent lui appartient. C'est c'est son argent, et ce serait le seul chose un des rares domaines je n'en vois pas d'autres ou après un engagement initial de 8 ans on serait captifs et seule l'assureur pour essayer de votre sort. Moi je prends un exemple qui m'a un peu choqué, qui est venu je crois dans le débat du PLF à l'initiative de Christine Lavarde. La question, membre de la vente une condamnation ING qui a été vendu à Boursorama.

donc on l'a voulu, en matière d'assurance vie, on a voulu en matière d'assurance emprunteur. On a voulu prendre en matière de. D'assurance dommages, dans les autres domaines on peut et c'est normal, changer là il y a une règle comme assez longue après 8 ans, ce serait le seul domaine où on serait captifs alors et ça l'impression que l'argent n'appartient pas à l'assuré à l'épargnant. Mais à la compagnie d'assurance et on a parlé à l'instant de finance verte par exemple, il y a des compagnies qui n'en proposeront pas si le si le l'assuré souhaite aller vers d'autres produits, libre à lui de pouvoir changer. Donc c'est un minimum de liberté qu'on doit pour l'argent qui partir non pas la compagnie mais qu'elle retient l'assuré, y compris je dans le cas de vendre une compagnie d'assurance, c'est un exemple qui m'avait un peu. Alors. Alors. Sommes-nous suffisamment éclairé donc je mets aux voix l'amendement de suppression de monsieur Savoldelli. Qui finalement a fait l'objet de 2 avis défavorable qui est pour. D'accord. Qui est contre. Il y en a un peu plus. Et qui les abstentions. Il est pas adopté. Donc nous allons pouvoir commencer avec le premier amendement de madame Lavarde qui porte le numéro 4 rectifié la la parole. depuis la promulgation de la loi pacte ils se posent. Enfin, il existe 3 situations lors d'une demande de transfert interne alors soit un accord automatique de l'assureur pour un transfert au sein du même courtier c'est notamment le cas depuis l'engagement déontologiques des assureurs pris en juillet 2021 un refus systématique de certains assureurs pour un transfert entre 2 courtiers ou 3e cas une acceptation de certains assureurs si et seulement si le courtier d'origine et d'accord. Alors tout ça est un peu bizarre et ça donne le sentiment. Que la loi pacte n'est pas vraiment appliquée, en tout cas telle que l'a voulu le législateur et je vais d'ailleurs à l'appui de cet argument, vous citez à la page 73 du rapport de France Stratégie hein sur l'application de la loi pacte qui dit que donc le rapport du Sénat. Il s'agit du rapport de Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier note que les demandes de transfert se heurte à la séparation entre les assureurs, qui gère le contrat et les courtiers qui en assure la distribution en pratique les transferts de contrats avec un changement de distributeurs ont pu se révéler complexe pour les assurés. Donc là l'adoption de l'amendement que je propose permettrait en fait de mettre fin à cette situation différente. Suivant si le transfert a lieu à l'intérieur du même courtier ou entre différents courtiers qui sont toujours dans la même. Chez le même assureur et donc en fait de permettre à tous les épargnants, d'être sur un pied en quelque sorte. Sa vie à écrire dans le dur de la loi, quelque chose qui a été, il me semble, voulue par le législateur en 2019. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur général. une, une demande de retrait parce que le. Le texte de la commission permet de dire que le, l'amendement est déjà satisfait. Et et je veux simplement peut-être apporter une précision supplémentaire parce qu'il pourrait y avoir avec l'amendement une une Une part de confusion puisqu'il ne mentionne pas par exemple le cas où la transformation et réalisée directement auprès de l'assureur sans intermédiaire, ce qui peut donc amener une complet ce qui pourrait

Merci. Nous passons à l'amendement 12 de Monsieur épais. Oui, merci Monsieur le Président. Les assureurs mettent du temps à concrétiser les transferts de. De compte et donc le texte propose de leur donner de mois pour cela. Et cet amendement de le réduire à un mois. Commission. Un tant que j'appellerai incompressible. Quelques éléments peut-être pour éclaircir ou éclairées plutôt. La vie vous prenez. Une demande qui arrive. Dans un mois de mai habituel avec énormément de pont, vous aurez à vous avez à peu près une dizaine de jours pour répondre. À la demande. Je rappelle qu'avant de faire droit dans ce délai de 2 mois. Heureusement d'ailleurs ça la la la la compagnie à la faculté de faire une contre-proposition donc je pense que déjà de respecter le délai dit incompressible de deux mois est une bonne formule. Je pense qu'elle suffit largement qu'elle se justifie d'ailleurs dans le. C'est pas excessivement long. Pour la même si la personne maintient qu'elle est une contre-proposition ou pas. Je pense que c'est un délai qui est raisonnable, qui est d'ailleurs la plupart du temps. Le délai on l'avait vu, ah bon dans un certain nombre de disposer de dispositions sur les résiliations et cetera ça permet d'avoir le temps logique pour une éventuelle négociation. Alors. L'avis du gouvernement. Même avis. Monsieur. Cannet vers retire son amendement. Nous passons à l'amendement 6 bis de Madame gageure. Monsieur le président, il s'agit ici de préciser la rédaction en fait du dispositif relatif à la transférabilité. Il est proposé en fait de décider pour le cas où un intermédiaire d'assurance est impliqué dans ce transfert hein que l'intermédiaire est tenu de transmettre sans délai cette demande à l'entreprise d'assurance pour préciser en fait. Sur qui pèse la charge des risques en fait qui est impliqué au terme. de responsabilité en fait dans le transfert et ensuite que les frais encourus ne peuvent être supérieur à 1% pour l'assurer pour éviter des frais qui soit composée Audi Audi transfert. Et l'opinion de la commission. C'est un avis défavorable, alors. Je pense que l'amendement pourrait. Créer finalement une une insécurité juridique 2 éléments la précision selon laquelle le l'intermédiaire est tenu de transmettre comme c'est précis sans délai la demande de l'assurée à l'entreprise de de d'assurance finalement pourrait faire naître une insécurité juridique et peut être des contentieux fréquents sur ce qu'on appelle le délai. Et puis. La précision selon selon laquelle les frais encourus à l'occasion de ce transfert ne concernerait que l'assuré paraît superfétatoire puisque le texte évoque justement des droits acquis on aura un doute quant à la rédaction. Celui-ci ne pourrait finalement que profite à l'assuré puisque si les frais totaux encourus lors du transfert sont bien inférieurs à 1% des droits acquis, la part supportée par l'assuré sera alors forcément inférieure ou égale à ce total. L'avis du gouvernement et même la même Paoli-Gagin. Retire son amendement. Nous passons à l'amendement 3 rectifier le madame Lavarde. Merci. Alors cet amendement. Évoque le 3ème usage du courtage. Alors je suis désolé, c'est un petit peu technique mais c'est un usage qui est fréquemment invoquées par les assureurs ou les courtiers pour freiner les transferts prévus par la loi pacte alors ce 3ème usage en fait. Il prévoit que le courtier d'origine a droit à une commission tant que dure le contrat, même en cas de changement de courtiers et l'assiette des commissions Mon Repos sur les primes qui ont été apportées durant la gestion du courtier porteur alors je vais aller très très vite, mais il y a eu une directive sur la distribution d'assurances qui s'applique depuis le premier octobre 2018, et qui revient à remettre en cause le 3ème usage du courtage pour tous les contrats qui sont postérieurs à cette date en fait, la question se pose pour tous les contrats antérieurs donc au premier octobre 2018. Et donc pour ces contrats, on se retrouve dans les cas de figure que j'évoquais quand je parlais de l'amendement précédent pour pour certains il y a pas de problème et puis pour d'autres. On est face. À un frein qui est liée notamment à ce 3ème usage du courtier du courtage pardon alors mercredi en commission des finances a été adopté un amendement qui vise en fait à aligner un peu le fonctionnement de l'assurance vie sur le fonctionnement du père avec la fixation d'une grille pour les frais en fait, cet amendement il vise un peu à faire la même chose, c'est-à-dire à aligner le fonctionnement de l'assurance vie sur le fonctionnement du père pour ce qui concerne le 3ème usage du courtage. Alors l'avis de la commission. que non effectivement pour un certain nombre de contrats, c'est ce qu'on appelle l'indemnité entre guillemets compensatrices, c'est-à-dire c'est le montant en général d'une année de commissions. Liées au contrat. Ce que, ce que je crois c'est que ça relève plutôt des pratiques. Des compagnies de ce que j'appellerais un peu le, les règles de bon fonctionnement ou le règlement intérieur et je pense, pour le coup qu'il devrait plutôt y avoir. De comment dirais-je. Des consignes et un accord entre assureurs à partir du moment où une demande est formulée. On l'a fait rentrer dans un délai de maximum deux mois. La question en fonction de la date de souscription du contrat de ce qui pourrait être dû à un intermédiaire parce que effectivement il perd à la demande de son assuré. Le contrat de doit à mon avis pouvoir hein, faire l'objet de la petite, comment dirais-je indemnités qui lui revient mais sans que ce soit nécessaire de l'inscrire dans la loi parce que c'est plutôt des règles de bonnes pratiques. À défaut d'un accord de place mais on va pas aller jusque-là, Monsieur le Ministre. Donc un avis défavorable défavorable. L'avis du gouvernement de fumisterie. Le le point hé hé bien pris on va saisir le CCSF sur ce sujet donc demande de retrait à défaut défavorable.

donc c'est un retrait. Merci cher collègue. Ensuite nous avons quatre amendements identiques. Que nous commençons par celui du gouvernement qui est le 29. le cet amendement pour obliger de supprimer la possibilité ouverte par l'article 7 de permettent la transférabilité externe tout en préservant la transe militer la transférabilité interne de l'assurance. Pardon. Je me suis mal exprimé selon dans amendements en discussion commune mais ils ne sont pas identiques, donc j'appelle maintenant le 2ème amendement le numéro 16 de Madame Procaccia. Oui merci. Je me réjouis de voir que monsieur. De Montgolfier a bien été ah tiens à son attention attirée par l'amendement que j'avais présenté. Au PLF et et qui demandait simplement de réduire va d'accepter la transférabilité dans les cas très précis et en l'occurrence. vous avez cité le cas d'ING quand une banque. Fournissait de l'assurance vie. Clôture tous ses comptes en France les transferts vers un autre opérateur, es transfert en même temps l'assurance vie. Sans aucune hein enfin en simple information tous vos contrats. Vous avez le droit de prendre de ne pas transférer vos comptes dépôts vos comptes livrets vos comptes épargne CEL et cetera par contre vous êtes dans l'obligation d'accepter le transfert de l'assurance vie alors qu'on me dise. Que l'assurance-vie et déstabilisé. Ici, on permet un transfert dans des cas qui sont des cas exceptionnels, combien de fois en disant cela s'est-il produit. Je sais que bientôt il y aura HSBC qui va se rapprocher. Je ne sais pas. Quel sera le corps le sort des contrats d'assurance vie proposée par HSBC. Ce que je peux vous dire c'est que le nouvel opérateur qui s'appelle Boursorama le communique bien en disant, nous sommes le gestionnaire de votre nouvelle de votre assurance vie et absolument pas, nous sommes l'opérateur réel et. Generali donc je demandais en matière d'assurance vie et de transférabilité d'autoriser dans ces cas précis, le ministre de. Des finances sur le banc, m'avait dit tenez moi au courant s'il y a. Si vous avez des informations complémentaires, je lui ai écrit en lui donnant des éléments et la communication qui est faite sur ce sujet. Donc je pense que c'est bien moins important que la transférabilité totale mais ça irait quand même davantage dans le sens de ce que voudrait le ministère le ministre ici au banc. Madame Procaccia puisque nous sommes en discussion commune il nous attendons ce que vous présentiez vos 2 autres amendements. Je ne les avais pas dans le bon ordre. Pardon. Donc on va commencer par le sous-amendement de madame Lavarde.

c'est ah rendent parfaitement opérationnel. Les amendements, 16 et 18. Que je rejoins parfaitement parce que je pense que le cas exposées par Madame Procaccia et j'entends que le gouvernement et compte la transférabilité externe. Il va peut-être falloir quand même aussi prendre le cas ses clients liés qui eux non Riancho Asie quand ils sont dans un cas aujourd'hui de transférabilité interne et donc c'est juste à une correction sémantique pour utiliser le terme d'intermédiaires d'assurances, qui est-ce qui est visé plutôt que entreprises d'assurance. Alors nous poursuivons la discussion commune de cette fois-ci, c'est l'amendement 18 de Madame Procaccia qui n'a pas de sous-amendement. Voilà, merci Monsieur le Président. Eh bien j'ai évoqué dans la discussion générale. Le fait que je m'interrogeais sur la transférabilité après 8 ans sachant que la plupart des contrats d'assurance ont une durée de 8 ans et je propose je me doute. Contre l'avis de la commission. Des finances mais je propose que cette transférabilité soit possible après 12 ans, après 12 ans, j'ai regardé des tableaux c'est 12 c'est 12 à 15% enfin c'est ou 20% maximum des contrats d'assurance vie et non pas 70% des contrats d'assurance vie. Il y a et donc maintenant vous pouvez. Votre amendement 17. Et le dernier dans la discussion commune et qui sera accompagné d'un sous-, amendement qui a déjà été défendu. Un amendement de repli. Pour adapter la transférabilité externe. Vers des situations où l'assuré voit son contrat se transférer vers un autre opérateur. Il crée une exception à la condition de durée l'externe pour la transférabilité externe donc amendement de repli de souplesse. Parce que dans le cas que j'ai cité le gestionnaire théoriquement ne change pas mais le client. Doit quand même gérer son contrat et c'est la raison pour laquelle en suspendant la la condition de durée, on offre une transférabilité plus aisée. Et donc madame Lavarde ajoute aussi un sous-amendement qu'elle a déjà expliqué pour cet amendement là. Donc maintenant la Commission va donner son avis sur cet ensemble en commençant par le 29 du gouvernement. Voilà donc ce un avis défavorable sur l'ensemble des amendements. Le 29, ce n'est pas une surprise. Le gouvernement le sait je vais rentrer un peu plus en détail sur 18 16 17. Dans le 18, comme. L'amendement le propose finalement en passant la durée d'assurance vie de 8 à 12 ans on va à l'encontre de l'objectif visé, qui est plutôt de donner de la souplesse. À l'épargne de la fluidifier. Je vais quand même vous donner un élément. Vous avez des, des réseaux pour lesquels la duration moyenne. Alors on a, on a dit et 12 ans et de l'assurance vie, je dis bien des réseaux hein. C'est 19 ans. Alors c'est des réseaux avec intermédiaire ce qui démontre. Que le Conseil. À mon avis a une utilité et je fais l'observation, en considérant que c'est avant les éventuelles améliorations sur le conseil qu'on nous propose, dans cette proposition de loi. Donc derrière les moyennes on peut vraiment dire beaucoup de choses sur l'amendement les amendements, 16 et 17. Dans l'affaire. ING pour faire très bref ING en fait c'est un changement de distributeur. j'ai posé la question dans les auditions et en fait, l'assureur vie est resté le même. Non non mais le, l'assureur vie puisque c'était dans les deux cas, c'était la même compagnie d'assurance C'est la raison pour laquelle on propose toujours la transférabilité enfin on soutient nous la police militaire, une transférabilité externe au-delà dès 8 ans. Voilà, on reste dans la même dans et donc. Un des risques d'adopter un de vos amendements en plus dans le 16. C'est que finalement. On aurait une une durée. Uniquement lorsque l'assurance vie est géré par une entreprise d'assurances que le client n'a pas forcément choisis, ce qui veut dire que on priverait de liberté on écraserait le texte que nous proposons de la commission. Donc, avis défavorable sur l'ensemble des amendements et retrait des 46 et 47. Les sous-amendements. Alors maintenant l'avis du gouvernement sur les autres amendements que le sien, c'est-à-dire le 16 le 18 et le 17. Et si c'était dans l'ordre ce serait précieux. Monsieur le Ministre.

Difficile de s'y opposer. Même si ce que le gouvernement souhaiterait c'est le renforcement. Prévu par la proposition de loi de la transférabilité interne sans ouverture à la transférabilité externe y compris dans des, dans le le le cas qui est, qui est cité où on comprend bien. Que lorsque même le distributeur change au fond on voudrait changer mais dans ce cas précis celui d'ING. L'assureur comme l'a dit le rapporteur n'a, n'a pas changé donc avis de de sagesse du du gouvernement sur ces amendements qui viennent restreindre la transférabilité etc. J'ai donc appelé les différents amendements. Nous commençons par l'article l'amendement 29, qui est celui du gouvernement qui a donné lieu à un avis défavorable de la commission, quels sont ceux qui sont pour. Contre.

Donc le sous-amendement de madame Lavarde numéro 46. L'amendement numéro 16 qui est pour. Madame Procaccia pour le sous-amendement chaleur. Remercie madame Lavarde qui apporte une précision. De professionnels que je ne suis pas.

oui. Donc. Sur cet amendement sur ce sous-amendement qui. Ont fait préfigure l'amendement. Nous avons des amis des enfin un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement qui est pour.

Même dispositif c'est-à-dire avis défavorable du gouvernement de la commission, autant pour moi et de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. L'abstention. N'est pas d'adopter et ce que je peux. Réputé que c'est le même vote sur les amendements 18 sous-amendement 47 et amendements 17. On est tous d'accord, ils ne sont donc pas adopté. Alors on va voter sur l'article 7 finalement pas modifié. Qui est pour. Qui est contre. Tiens donc il était adopté. Je peux mettre aux voix pour le même prix. L'article 7 bis nouveau sur lequel il y a pas l'amendement qui est pour. Abstention donc il est adopté. Je vais suspendre la séance. Et elle sera reprise à 21h. 30. Et on fait un prix. Pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.